La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Nous n'avons pas reçu d'observation, il y en a-t-il en séance. Je n'vois point il est donc adopté sur les réserves d'usage. Madame la première ministre, mesdames et messieurs les Ministres, chers collègues, notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement notre séance et retransmise en Direct sur Public Sénat et sur notre site internet, chacun sera attentif au respect des uns et des autres et à celui du temps de parole et je donne immédiatement la parole au président Jean-Claude Requier pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci monsieur le Président Madame la première ministre après la crise des gilets jaunes et la pandémie de Covid 19 qui a mis à l'arrêt, le monde durant 2 amené notre pays est confronté depuis plusieurs mois un nouveau choc économique majeur avec l'explosion des coûts de l'énergie et puis largement, de très fortes hausses de prix des matières premières et de l'alimentation, cette accélération de l'inflation en partie frappent désormais toute notre économie et le quotidienne de nos compatriotes à Jeanne Brown de fortes tensions sociales dans de nombreux secteurs, les revendications de revalorisations salariales sont bien sûr légitimes dans un contexte inflationniste auquel nous étions plus habitués, nous devons Ramtane dans ce qui demande une répartition plus juste de la valeur ajoutée, à laquelle il contribue et une rémunération digne de leur travail, la solidarité doit aussi continuer à s'exercer envers les plus fragiles dans ce climat social tendu le dialogue et la négociation doivent demeurer les outils, la sortie de crise, en particulier dans les raffineries et ou les transports publics, les revendications sont connus et ont pu s'exprimer, elle ne peut cependant plus justifier un blocage indéfini notre économie, au risque de pénaliser des millions de personnes et d'entraîner le pays dans une boucle de récession, nous savons la pris la première ministre a la volonté d'autres gouvernements à oeuvrer pour le pouvoir d'achat et de niveau de vie des Français, nous nous comptons aussi sur la responsabilité des entreprises pour répondre sur le long terme, aux attentes des salariés voilà dire ministre comment comptez-vous maintenant à agir pour répondre aux attentes de nos compatriotes. Je sais que vous êtes élue dans un département où la voiture n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour le travail pour le quotidien. Et je sais votre attends votre attention particulière à tous nos compatriotes qui veulent vivre de leur travail, qui s'inquiète face à la montée des prix qui subissent de plein fouet les tensions d'approvisionnement dans les stations services et craignent le blocage du pays. Monsieur le président, Wauquiez ses préoccupations, ce sont aussi les nôtres. Certains cultivent les inquiétudes et veulent l'échanger en colère. Nous, tout comme vous, monsieur le président, nous voulons y répondre apaiser le pays et rassembler les Français aussi pour protéger nos compatriotes face à l'inflation, nous avons pris des le précédent quinquennat des mesures fortes avec un bouclier tarifaire dès octobre 2021. En juillet, vous avez voté des textes d'urgence en faveur du pouvoir d'achat et, plus récemment, j'ai annoncé la prolongation des bouclier tarifaire et le maintien jusqu'à mi-novembre, de la remise de 30 centimes sur les carburants, ce sont les mesures les plus protectrices d'Europe et nous avons l'inflation la plus basse de la zone Euro. Mais je car je garde une conviction, une conviction que nous avons en commun sur bon nombre de ses rangs une conviction partagée par nos compatriotes, le pouvoir d'achat durable viendra du travail alors concernant particulièrement les salaires, hein, vous le savez, notre pays dispose d'un système unique au monde de revalorisation automatique du SMIC, de ce fait, le SMIC a augmenté de 8 % en un an, c'est-à-dire plus que l'inflation qui est autour de 6 % cette augmentation doit conduire en conséquence à une revalorisation des grilles salariales dans les différentes branches professionnelles, la dynamique est lancée puisque depuis le début de l'année, plus de 500 accords de branche sur les salaires ont été signés, mais au-delà, je l'ai dit, je le crois et je le répète : les entreprises qui le peuvent doivent augmenter les salaires, elles le doivent d'autant plus dans le contexte d'inflation et elles ont une responsabilité particulière, si elles ont réalisé plus de profits, malgré le contexte pour y parvenir, des négociations doivent se tenir dans les branches et dans les entreprises, et elles doivent avoir lieu rapidement, car j'en suis convaincu, la seule solution vient toujours du dialogue social. Le blocage, le refus de la discussion, par une minorité ou la grève préventive ne sont jamais les solutions et je pense ici à tous les Français qui rencontre encore aujourd'hui des difficultés pour trouver du du carburant, heureusement, la situation s'améliore, mais nous serons mobilisés jusqu'à un retour à la normale, je vous remercie. ont besoin de se déplacer, de voitures et les voitures sauf électriques comme Bowen désastre il faut approvisionner les stations services dans cette phrase là, la voiture est indispensable et contrairement au centre-ville et qui la bannissent sans lui fera son usage est apprécié, et le terme bagnole n'y ait pas un gros mot. Merci monsieur le président. Je vais donner la parole à notre collègue Daniel Breuiller pour le groupe écologiste solidarité territoires. Monsieur le Président Madame la première ministre ma question est simple travail on nous pour rien. Conseil national de la refondation travail transpartisan dialogue de Bercy autre gouvernement démultiplie les annonces et les rendez-vous dit de concertation, mais en même temps vous laisser planer depuis plusieurs mois, la menace du recours éventuel potentiel à l'article 49 3 de la Constitution et cela sur les sujets essentiels de la vie des Françaises et des Français, les retraites, l'assurance-chômage, le projet de loi de finances, cette conception de la démocratie et déroutante, surtout dans ce contexte de crise multiple et d'inquiétude grandissante des citoyens comme des collectivités, les mobilisations contre la vie chère et l'inaction climatique ou pour la hausse des salaires, montre bien les attentes de nombres de nos compatriotes, les députés ont en responsabilité face au besoin de justice sociale et écologique largement amendé le projet de loi de finances, c'est le rôle des consensus ont été trouvés, par exemple, pour que ma prime rénovent finance davantage des rénovations globale que des petits travaux ou encore pour taxer à 35 pour 100 des super-dividende je pense également au crédit d'impôt pour le reste à charge de tous les résidents en Ephad Madame la première ministre alors que vous choisissez d'écourter les débats au moyen du 49 3, prenez vous l'engagement de présenter au Sénat le projet de loi de finances, enrichi par le travail parlementaire de nos collègues députés, pouvez-vous nous assurer que nous ne travaillons pas pour rien et nous confirmer que nos amendements sénatoriaux non pas également vocation à disparaître dans les poubelles de tri présidentielle ou bien nous préciser le cas échéant, s'il faut désormais soumettre nos amendements directement au président de la République. Pour vous répondre, la parole est hein. Monsieur Véran, porte-parole du gouvernement. des mois, désormais celle de la concertation de la main tendue de la volonté farouche de travailler en commun et d'arriver à trouver au-delà des clivages politiques traditionnels des voix des chemins de crête pour pouvoir travailler ensemble au à l'intérêt général pour notre pays, il en est ainsi, avec l'examen du budget, vous l'avez souligné, c'est le 8ème jour du débat à l'Assemblée nationale sur la partie du projet de loi de finances, les débats sont riches, ils sont passionnants passionné évidemment certain consensus ont pu être retrouvés et le gouvernement par la voix de la première ministre a déjà annoncé que, quel qu'en soit l'issue, il s'engageait à reprendre un certain nombre d'amendements qui avait permis d'enrichir le texte venant des majorités et des rangs des oppositions madame madame la sénatrice, vous dites tous si je devais fait faire le compte à l'heure à laquelle je vous parle, nous en sommes à 8 milliards de sur, dépend si nous devions tenir compte de la totalité des amendements, des oppositions telle qu'adoptée en première lecture, 8 milliards qui ne sont pas financés 8 milliards qui correspondrait ou à de la dette supplémentaire pour notre pays, ou à des impôts supplémentaires pour les Français. Or. Or, si le chemin du dialogue est réel et si la volonté de trouver des compromis, je le redis et permanente, nous ne rogne auront pas sur un certain nombre de principes qui sont chers au président de la République à la première ministre et à cette majorité, de hausse d'impôts, il n'y aura pas de hausse de la dette, nous ne détricote rompt pas l'ensemble des mécanismes qui ont permis à notre pays de retrouver son attractivité et sa richesse en 5 ans, et nous n'iront pas, nous nous réunirons pas les engagements qui ont été pris par le président de la République lors de la dernière campagne présidentielle et pour lesquels il a été élu, je vous remercie. Monsieur le Ministre, retenez nos propositions comme les taxation des superprofits la démocratie sans dialogue social et sans Parlement, ce n'est plus tout à fait la démocratie. La parole est maintenant. Au président Claude Malhuret pour le groupe. Les indépendants. République et Territoires, monsieur le président.

ouvriers bloqués dans les que des stations service, infirmière en panne et leurs patients qui attendront artisan au chantier suspendu le syndicalisme trash, c'est ça : des salariés payés le double de la moyenne qui empêchent les autres de travailler et qui en plus prétendent les défendre à tous ceux tentés de croire à cette arnaque, je voudrais rappeler ce dicton, on finit toujours par payer le joueur de pipeau, le comble du cynisme, c'est quand on apprend que ces grèves n'ont rien à voir avec le pouvoir d'achat, mais que ces règlements de comptes à CGT chorale les durs de la fédé chimie mécontent que Martinez, fidèle à sa conception de la démocratie est nommé tout seul sa successeur qu'il trouve trop molle déclenchent la grève pour le déstabiliser pour les faire taire, il en rajoute dans la radicalité sur le dos des Français, comme toujours, personne n'est dupe et l'Automne chaud que nous promettent les agents d'ambiance de l'agit-prop piétine les grèves sont condamnés par une majorité de Français, la journée d'hier fut un échec comme le fut dimanche la marche des gros shows marxiste de la Nupes, emmenée par le Che Guevara de Nation, Bastille. la prochaine étape est encore plus obscène la récession guette la planète, le prix de l'énergie mais des usines à l'arrêt, les Français vont avoir froid cet hiver, mais la même CGT pour la plus grande joie de Poutine empêchent la maintenance des centrales nucléaires qui nous permettrait de surmonter l'arrêt du gaz russe Madame la première ministre, vous avez commencé de prendre les réquisitions qui s'impose, pouvez-vous nous assurer que vous-poursuivrait toutes les mesures nécessaires pour que 90 % 90 par Sun, pardon ne puisse interdire à la moitié de la France de se déplacer et que quelques centaines d'autres ne puissent empêcher nos concitoyens de se chauffer au coeur de l'hiver. Pour vous répondre, la parole est à Madame la première ministre. Merci monsieur le. Président, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Maluret. Le conflit social chez Total et Esso, a des répercussions dans tout notre pays, et touche le quotidien de millions de Français. Comme vous, Monsieur le Président Maluret j'entends et je partage les préoccupations de nos concitoyens, qui craignent de ne pas avoir de carburant pour aller travailler, que leur aide à domicile ne puisse pas passer, qui craignent de devoir renoncer à retrouver leurs proches pendant les vacances de la Toussaint. Pour eux, nous devions agir fort et vite, en lien avec le président de la République, le gouvernement est totalement mobilisé et je réunis quotidiennement une cellule interministérielle de crise pour coordonner l'action des services de l'État dès les premiers jours de la grève, nous avons pris des mesures pour augmenter les livraisons de carburant dans les stations service, nous avons notamment libérer des stocks stratégiques de l'État, nous avons augmenté les importations nous avons autorisé l'ouverture des dépôts et les livraisons le week-end, ces mesures ont eu des effets importants sur les livraisons de carburant et ces derniers jours, elles étaient jusqu'à 2 fois plus importante qu'en temps normal, mais les inquiétudes des Français, compte tenu des inquiétudes des Français face face au risque de pénurie, nous avons assisté à une augmentation de la demande plus forte que cette augmentation des livraisons aussi, il était essentiel de sortir du conflit social, je me suis impliqué personnellement pour que le dialogue social et lieu chez Esso et chez Total et dans ces 2 entreprises désaccord ont pu être signé avec des syndicats représentant une majorité des salariés. Quand il y a un accord majoritaire, le travail doit reprendre une minorité ne peut pas, ne doit pas bloquer le pays, c'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au préfet de réquisitionner les personnels nécessaires au fonctionnement dans certains dépôts aujourd'hui avec la fin du Golfe conflit social chez Esso et l'ensemble des mesures prises par le gouvernement, la situation continue à s'améliorer nettement au plan national, ce matin, 20 % des stations étaient en rupture sur au moins un produit, elles étaient 30 % ce week-end, et peut être plus précisément parce que la situation peut être contrastée par territoire, je voudrais souligner que la situation s'améliore sur tout le territoire dans Les Hauts de France, on était à 55 % de stations en rupture, il y a une semaine, nous sommes aujourd'hui à 15 % en Île-de-France avec le débloquer, pardon, la situation se s'améliore également avec lui 8 points de moins sur le nombre de stations et et dans votre région en Auvergne, Rhône-Alpes le déblocage du dépôt de Feyzin permet des améliorations sensibles depuis hier matin, nous sommes passés de 36 % à 26 % de stations en rupture, je sais que la situation est encore difficile pour beaucoup de nos compatriotes, mais la dynamique est là et je veux une nouvelle fois appelé les salariés grévistes à reprendre le travail, il est inacceptable qu'une minorité bloque un pays et de notre côté, Monsieur le Président, nous continuerons à agir jusqu'au retour à la normale, je vous remercie. La parole est maintenant président Bruno Retailleau pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président Madame la première ministre depuis dimanche dernier, la France est sous le choc, le là, une jeune fille de 12 ans. A été sauvagement agressé et les morte agressée par une ressortissante algérienne qui n'aurait pas dû être sur le sol français depuis dimanche, des voix s'élèvent pour que d'autres, de voir se taisent pour imposer le silence. Pour bâillonner le débat. Mais l'essence même de la démocratie, mes chers collègues précisément questionnement, c'est le débat, le meurtre de Lola me rappelle un autre meurtre qui m'avait touché personnellement. Le meurtrier à l'époque était depuis plus de 10 ans en situation irrégulière, il était sur le sol de France. Il avait été frappé par 3 OQTF, il n'était pas expulsé, il a incendié la cathédrale de Nantes, il n'était pas en prison. Il avait une santé précaire mental, il n'était pas un hôpital psychiatrique et vous voudriez Madame le 1er Ministre que nous nous Dion, ce sont les Français qui réclame des comptes et il faut l'admettre le désordre migratoire peut tuer si cette algérienne avait pas été sur le sol français le là aurait été encore en vie, j'ai une double question à vous poser : la première, reconnaissez-vous des défaillances de l'État. Une part de responsabilité, la seconde, que dites-vous aux Français pour que ces tragédies et ces drames ne se reproduisent plus. Pour vous répondre, la parole est à Madame la première minute. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, Retailleau. Je crois qu'en politique, quelles que soient les circonstances, nous devons toujours faire le choix de la dignité. Une jeune

une jeune fille de 12 ans a été tué dans des conditions effroyables, une famille, des amis, des voisins. Un collège sont en deuil et tout le pays, partage leur émotion. C'est pour les parents de Lola, que je veux avoir mes premiers mots. Le président de la République a eu l'occasion de les recevoir hier. Et de leur dire toute l'émotion et la solidarité de la nation et je souhaite à nouveau dire à cette famille. Au nom du gouvernement et j'en suis sûr en votre nom à tous, notre plein soutien. Et Monsieur le Président, Retailleau, savez-vous ce qu'ont demandé les parents de Lola du respect. La paix pour la mémoire de Lola et qu'on les laisse faire leur deuil dans la dignité. Nous le leur devons et je le dis franchement : je crois que la dignité nous commande de ne pas exploiter la douleur indicible d'une famille de ne pas utiliser la mort d'une enfant à des fins politiciennes. Ce que nous devons à la mémoire de Lola et à toute sa famille, c'est la justice, une enquête a été immédiatement lancé les services de police ont pu identifier et interpeller des suspects en quelques heures, 2 personnes ont été. Es mis en examen par les juges d'instruction et l'une d'elles se trouvent en détention provisoire, l'enquête se poursuit aujourd'hui pour déterminer précisément les faits. Et il y a une autre chose à laquelle je crois profondément, monsieur le président, c'est à l'indépendance de l'autorité judiciaire. Je ne dis donc pas d'autre commentaire à faire, laissons les enquêteurs travailler, laissons la famille de la faire son deuil en paix, nous leur devons justice ils l'auront, et c'est la République qui la rendra je vous remercie. Madame la première ministre, vous vous trompez en réduisant la mort de Lola, un simple fait divers, je pense, vous voyez que la politique se diminue quand elle refuse le débat, je pense que la politique ne peut pas se contenter de pleurer sur les conséquences, elle doit en dénoncer aussi clairement les causes, elle doit affronter la réalité pour que ces meurtres ne se reproduise plus, Madame la première ministre que vous êtes une responsable public chaque responsable public doit avoir le courage d'affronter la réalité et doit protéger les Français, avec une politique, il ne s'abandonne pas justement aux laxiste et au laisser-faire migratoire, vous devez prendre des décisions, toute de suite pour aujourd'hui pour demain. demain. La parole est à notre collègue Loïc Hervé pour le groupe. De l'Union centriste. Monsieur le président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou plutôt à monsieur le Ministre délégué en charge de l'industrie, le Mondial de l'auto a été l'occasion d'annonce politique d'importance pour continuer d'accompagner la filière vers sa transformation qu'il s'agisse d'un entretien du président de la République dans Les Échos ou des propres déclarations du ministre Bruno Lemaire. Toute la filière automobile française des nos dans d'ordre aux sous-traitants et Fleurot qu'il nous faut savoir préserver malgré les contraintes considérables auxquels l'ensemble de cette filière se trouve confronté, qu'il s'agisse du coût de l'énergie, de la compétitivité ou d'énormes le virage de l'électrification va nécessiter en soit des évolutions majeures de l'outil de production, après les différentes vagues du plan de relance, de nouvelles aides sont prévues. Dans mon département, de la Haute-Savoie, singulièrement dans la vallée de l'Arve, l'industrie du décolletage est au coeur de ces enjeux et avec quelques outils mais surtout une myriade de PME qu'il faut accompagner une par une avec les meilleures chances d'être aidés, monsieur le Ministre, pouvez-vous garantir que les aides pourront bien aller aux entreprises qui le mérite, comment envisagez-vous de garantir l'accès équitable à ces aides pour toutes les entreprises sans qu'elle n'ait l'obligation implicite d'avoir recours à des cabinets, chasseur de primes dont les rémunérations sont indécentes et qui a montré moins de risques d'autant le volume des aides versées, je vous remercie. Monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, le Loïc Hervé, cette question est, vous l'avez dit tombe bien puisque nous sommes la semaine du Mondial de l'automobile, le 1er et le seul salon en Europe cette année, le 1er depuis 4 ans auquel est adjoint également le salon Equip Auto, donc on a toute la filière, les constructeurs et les équipementiers, réunis à la porte de Versailles sur vos moments perdus, je vous engage à y aller, parce que c'est toute l'industrie automobile française qui brillent, vous l'avez dit, le gouvernement a accompagné cette filière dans un moment difficile, la Covid France relance pour l'industrie automobile, c'est environ 750 millions et pour votre département que nous avons visité avec Bruno Lemaire il y a quelques semaines, la filière de la vallée de larmes, vous y a été là, la filière du décolletage, ça a été le 1er département accompagné avec 54 millions d'euros d'argent public qui ont conduit à 125 au total 1000000 d'euros d'investissements pour accompagner la filière, on va continuer, on va même accéléré, j'irai plus loin que ce que vous disiez vous disait l'objectif, elle est de préserver la filière non, l'objectif, il est de la développer, de s'assurer que l'industrie automobile qui va prendre le virage de l'électrification le fasse en toute souveraineté en réindustrialiser nos territoires et en développant ses filières qui en ont bien besoin, vous l'avez dit, pour cela il faut annoncer il faut accompagner toute la filière, y compris les petits sous-traitants qualificatif que j'apprécie pas beaucoup parce qu'ils sont petits par la taille mais extrêmement important dans la filière et notamment chez vous, en s'assurant que les 5 milliards d'euros, dont 1 milliard d'euros dédié à la sous-traitance qui sont au sein de France 2030 destiné à accompagner la filière puisse aussi toucher les petites et moyennes entreprises, je ne suis évidemment pas là pour choisir à la place des empreintes entrepreneur quel cabinet de conseil vont choisir ou pas pour demander telle ou telle aide mais ce que je peux vous dire, c'est que nous souhaitons que les appels d'offres quoi simple que les appels d'offres soient accessibles et qu'on puisse même sur le terrain, organiser un accompagnement public des entreprises pour qu'elle puisse remplir ses appels d'offres, on s'appuiera notamment sur les chambres de commerce et sur les pôles de compétitivité pour que les entreprises, pardon, petite, moyenne ou grande puisse profiter à plein de France 2030 merci. dans la vallée de la et Haute-Savoie ça reste quelque chose de très important, apprenons de ce qui s'est passé ces dernières années avec les 3 vague du plan de relance et morale ont l'octroi des aides pour que toutes les entreprises et la capacité d'avoir des aides merci. La parole est à notre collègue Marie-Noëlle Lienemann pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste avait la parole. Monsieur le Ministre de l'industrie en quelques semaines, 2 fleurons de notre industrie aéronautique et spatiale passe sous pavillon américain, deviennent propriété de la même société High Co, la société Excelya qui intervient dans l'aéronautique, le spatial, l'armement, mais aussi dans le médical, qui plus est, cette société devrait bénéficier du programme, France 2030 la société Trade, spécialisée dans la technologie des tests et analyses des effets de radiation sur les matériaux et composants électroniques fondamental pour la recherche spatiale, les avions de haute altitude et l'armement, entre autres, comment ne pas voir qu'il s'agit là de secteurs de haute technologie, essentielle pour l'autonomie stratégique de la France et qui concourent à notre souveraineté industrielle, comment pouvez-vous laisser faire ça doit-on revoir le sinistre scénario consécutif aux décisions d'Emmanuel Macron, avec la vente des turbines Arabelle essentiel pour les centrales nucléaires à l'américain General Electric pour devoir aujourd'hui les racheter au double du prix de vente 100 récupérer les licences, perte d'emploi, d'argent, de savoir-faire, vous auriez dû vous en souvenir, alors Monsieur le Ministre, pourquoi n'avez-vous pas déclenché le décret Montebourg qui permet au gouvernement de contrôler les investissements étrangers en France dans les secteurs-clés :

d'abord peut être rappelé le ce que vous appelez le décret Montebourg qui est en fait la procédure investissements étrangers en France, qui a été à la fois élargie et renforcée dans le mandat précédent, en accord d'ailleurs entre le Sénat et l'Assemblée, j'étais à l'époque, président de la commission d'affaires économiques et rapporteur général de la voix, et beaucoup travaillé sur ce sujet nous avons élargi les secteurs concernés, nous avons aussi renforcer la procédure de contrôle du Parlement sur ses investissements étrangers en France, une fois par an, vous avez un rapport qui vous êtes envoyé qui vous permet d'avoir la liste nombre d'investissements concernés et ceux qui ont fait l'objet d'autorisation sous conditions, je vous rappelle qu'en 2021 328 dossiers ont été soumis à la procédure dite Montebourg investissements étrangers en France et sur ces 328 124 124 pardon est autorisée, dont 67, sous conditions, aller plus loin, suppose de mettre en cause le secret des affaires et, parfois, le secret de la défense nationale et c'est pour pallier ce défaut que dans le cadre encore de la loi pacte nous avons voté une disposition particulière qui fait que sur des cas particuliers, les présidents des commissions des affaires économiques du Sénat et de l'Assemblée, les rapporteurs généraux du budget peuvent, sous le coup du sucré, du secret, pardon, examiner des cas particuliers mais vous comprendrez bien que pour les 2 raisons susmentionnées je ne peux commenter en détail des cas particuliers comme ceux que vous mentionnez, sachez, pour autant que, que ce soit pour la société Trade et pour la société Extelia vous mentionnez, évidemment, nous avons à coeur les intérêts stratégiques de la nation, la souveraineté industrie un industriel et les enjeux de secrets d'enfance quand nous examinons ces dossiers et nous l'avons fait et nous continuons à le faire, merci mes chers collègues, nos concitoyens ne comprennent rien, vous êtes ministre, enfin votre ministre monsieur le maire de la souveraineté industrielle on voit partir 2 fleurons, on sait que ces fleurons en particulier que Célia on sait qu'il a eu un débat et que vous n'aviez pas dans un 1er tour de table, trouver les actionnaires français, c'est pas un secret d'État, c'est dans tous les journaux de France et de Navarre, donc aujourd'hui, moi ce que je vous demande, on aimerait vous croire, mais on voit s'accumuler la perte de souveraineté industrielle du pays, pouvez-vous nous donner la garantie que l'État se maintiendra, ex-Elia et Trade à capitaux majoritairement français. La parole est à notre collègue. Michel Dagbert pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes qui avec. Merci monsieur le Président Madame la première ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail du plein emploi et de l'insertion, monsieur le Ministre, si depuis 2004, les départements assurent avec le concours de l'État, le versement de l'allocation au profit des bénéficiaires du RSA, l'exercice de cette compétence a été et demeure au coeur de bien des discussions entre départements et gouvernements successifs, les départements sont aussi en charge de l'accompagnement social et ou professionnels de chaque bénéficiaire cette politique publique participe, et c'est heureux, à la cohésion sociale du pays, sans remettre en cause la détermination des élus départementaux le professionnalisme de leurs équipes et tout en leur reconnaissant un certain nombre de réussite, il est à noter que, malgré la baisse significative du chômage, une longue liste de propositions d'emploi restent non pourvus les secteurs concernés sont diverses, serveurs de cafés restaurants, agent d'entretien Atsem Aide à Domicile Aide ménagère, voire même professionnels de l'animation socio-culturelle de quoi réinterroger légitimement l'adéquation entre les parcours d'insertion proposée et la réalité du marché de l'emploi, je sais, Monsieur le Ministre que quelques départements se sont portés volontaires pour une expérimentation, celle-ci fait craindre à une importante association du secteur social, une réforme qui, selon elle, s'apparente à un retour du servage n'ayant aucun doute sur la volonté qui vous anime en la matière, pouvez-vous, Monsieur le Ministre, devant mes collègues de la chambre haute, préciser les contours de cette évolution des politiques d'insertion et nous en donner le calendrier. On vous répond : la parole est au ministre du Travail, le pleine emploi de l'insertion, monsieur. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Dacbert vous l'avez dit pendant la campagne des élections présidentielles, le président de la République, alors candidat à réinterroger les modalités et la réussite du modèle et de l'outil qu'est le RSA RSA héritier du RMI, créé en 1988 avec cette volonté et c'est une fierté notre modèle social d'accorder et d'apporter un concours minimum un revenu minimum à celles et ceux qui se retrouvent sans revenus aujourd'hui les résultats en matière d'insertion d'intégration professionnelle de retour à l'emploi ne sont pas des résultats satisfaisants, ils ne sont pas satisfaisants parce qu'un rapport des cours de la Cour des comptes l'a montré au 1er semestre de l'année 2022, 7 ans après l'entrée dans le RSA 42 % des bénéficiaires sont encore bénéficiaire du RSA de manière permanente ou de manière discontinue, mais extrêmement régulière de la même manière, 7 ans après l'entrée dans le RSA, seuls 3 bénéficiaires sur 10 ont retrouvé un emploi, et seul un sur 10 à retrouver un emploi stable, ça nous oblige et ça nous oblige à agir, nous pouvons continuer à croire ou à penser que la société serait quitte de son devoir de solidarité, une fois qu'elle aura attribuer une indemnité d'un peu moins de six cents euros à une personne dépourvue de revenus, la conviction du gouvernement, la conviction que je défends devant vous et que la société sera quitte de son devoir de solidarité le ce qu'on leur a permis le retour à l'emploi parce que l'emploi, le travail et l'élément de d'émancipation, d'autonomie, de dignité et la capacité à retrouver un revenu, comment nous allons nous le faire, nous allons le faire avec un accompagnement plus intensif des bénéficiaires du RSA et je le dis tout net devant vous, il n'a jamais été question ni de travail gratuit ni de bénévolat obligatoire, il s'agit de formation, il s'agit d'accompagnement, il s'agit de de remobilisation collective et individuelle, mais il ne s'agit ni de bénévolat obligatoire ni de travail gratuit c'est important à souligner parce que ça ne correspond pas au modèle qui est le nôtre, le président de la République l'a dit, le RSA est un droit inconditionnel pour tous ceux qui sont privés de revenus, le devoir de la puissance publique de toute la puissance publique et de garantir une offre d'insertion et de formation adaptée personnalisée partout sur le territoire et de ce que ces de concision sont remplies, il y a une logique de droits et devoirs, pour faire en sorte que ceux qui en bénéficient s'inscrivent dans ces parcours de retour vers l'emploi et d'insertion par l'emploi. De la parole maintenant notre collègue Monique Lubin, pour le groupe socialiste. écologiste et républicain. Merci monsieur le Président Madame la première ministre le prix du gasoil dépasse les 2 euros le litre, les tarifs des différentes sources d'énergie augmente considérablement les produits de première nécessité, tels que les pâtes ou le beurre revoient leur prix augmenter de 22 à 47 %, la liste est longue, de tout ce qui concourent à la vie quotidienne des Français, dont une partie d'entre eux n'aura pas d'autre choix que de se priver, dans les semaines à venir et nous savons tous ici, qui seront les premiers à sacrifier des biens pourtant indispensable à ce que l'on qualifie de vie décente, vous répondez primes aléatoires défiscalisation et des socialisation d'heures supplémentaires, rachat de RTT et autres mesures qui finalement n'implique que les salariés eux- mêmes, mais vous refusez obstinément de satisfaire notre demande, surtout celle des salariés d'initier un grand débat sur les salaires, les salariés ne demande pas l'aumône, ils veulent vivre de leur travail, vous ne cessez de rappeler la valeur travail, souvent d'ailleurs pour stigmatiser ceux qui en sont privés, nous vous répondons pas de valeur travail sans travail de valeurs et la valeur d'un travail se mesure, entre autres, à l'aune de sa rémunération depuis 2008, les salaires des 10 % les mieux payés ont augmenté 3 fois plus vite que ceux des 10 % les moins rémunérés, est ce que le travail du patron d'une grande enseigne vaut 300 fois le travail de sa caissière, il est temps de parler du partage de la masse salariale dans les entreprises quand mettrez-vous Hanovre une conférence nationale afin de poser enfin tous ces sujets et soutenir par là même tous les salariés de France. On vous réponde, la parole est au ministre du Travail, monsieur Olivier Dussopt. vous auriez pu faire le constat avec nous que nous sommes le pays en Europe qui, par mesures mises en place le bouclier tarifaire sur les questions énergétiques, les aides que nous apportons aux ménages a permis de réduire l'inflation le plus possible, nous sommes autour de 6,5 % c'est beaucoup, c'est plus que ce que nous avons connu depuis 1985 mais c'est bien souvent, presque la moitié de ce que connaissent nos voisins européens et c'est aussi la démonstration que la politique que nous menons protège les Français, vous nous appelez M. finalement à une augmentation de salaire, nous avons une conviction, c'est qu'une augmentation générale des salaires ne se décide pas par la loi, cela relève du dialogue social, j'y reviendrai, nous avons eu notre conviction, c'est que l'augmentation ou l'indexation du SMIC vous avez parfois appelez de vos voeux dans les débats ne concernent finalement qu'une partie des salariés alors que notre position est de nourrir de pousser au dialogue social, la première ministre l'a dit tout à l'heure, nous engageons nous encourageons les branches et les entreprises, au dialogue et dans le cas du dernier projet de loi de financement rectificatif : vous avez voté le Parlement a voté des mécanismes permettant d'accélérer l'ouverture des négociations dès lors qu'un des niveaux de rémunération conventionnelle serait inférieur au SMIC, il faut ajouter à cela des outils que vous n'avez pas mentionné, vous avez parlé de défiscalisation, vous avez parlé des socialisation, vous avez oublié de dire les efforts que nous faisons pour améliorer le partage de la valeur, faire en sorte que les intérêts, les accords d'intéressement soit plus facile, faire en sorte que les primes que vous qualifiez d'aléatoire et qui bénéficie à des millions de Français soient elles aussi plus facile à verser, je peux vous assurer que celles et ceux qui peuvent en bénéficier sont heureux d'en bénéficier, bien plus que les mots vous prononcer pour les décrire ou pour les qualifier, vous avez dit que depuis 2008 et d'ailleurs cela interroge sur la responsabilité des uns et des autres, tout ce confondu de sur cette même période, il y aurait un écart croissant qui s'est creusé grâce aux outils de redistribution dans notre pays dispose, l'écart entre le 1er et le dernier décile ne s'est pas creusé, il ne s'est pas creusé parce que nous avons un système redistributif qui permet de compenser les écarts entre les revenus primaires et nous nous devons aussi en en faire une fierté dans quelques semaines, j'aurai l'occasion sous l'autorité de la Première ministre d'ouvrir une négociation interprofessionnelle sur le partage de la valeur, ça serait une première et j'espère que l'énergie que vous mettez à critiquer la politique du gouvernement, vous pourrez l'utiliser à meilleur escient en accompagnant ces discussions.

notamment sur les aides mais tout ce que vous venez de nous dire, visiblement, n'est pas entendu par la majorité des salariés qui ont besoin de cette conférence salariale pour que tous les employeurs de France à la mesure de leurs moyens et de la taille de leurs entreprises soutiennent et leur pouvoir d'achat, mais je constate que vous êtes plus prompt à dégainer le 49 3 pour mettre fin à un débat budgétaire pourtant absolument riche comme l'a dit tout à l'heure, Monsieur le Ministre, Véran qu'a organiser ce que les salariés demandent de leurs voeux depuis un petit moment maintenant. La parole est à notre collègue Anne Chain Larché pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, mes chers collègues, ma question s'adressait à Madame la première ministre ah vous entende madame tout va bien, alors que les Français le constatent chaque jour la France devient le pays de la pénurie, pénurie de médicaments, pénurie de carburant pénurie des transports, confronté à la grève, pénurie d'électricité annoncée pour cet hiver et face à ces pénuries on fait le terrible constat que le gouvernement n'a rien anticipé, il aura fallu plusieurs semaines avant de réquisitionner une partie du personnel de quelques raffineries, résultat : les Français font la queue pendant des heures devant les rares stations service ouvertes, la grève s'étend aux centrales nucléaires 11 central sur 18 été touchés hier, cette grève, si elle se poursuit, pourrait provoquer une terrible pénurie d'électricité RTE prévoit d'ailleurs, je cite, des conséquences lourdes cet hiver, si la grève se poursuit : qu'attendez-vous pour protéger les Français des pénuries dans ces secteurs stratégiques vous faudra-t-il, comme pour les raffineries attendre plusieurs semaines pour agir, allez-vous enfin réquisitionné toutes les raffineries allez-vous réquisitionner le personnel des centrales nucléaires, allez vous mettre en place un service minimum dans les transports comme le prévoit la proposition de loi de Bruno Retailleau, voté au Sénat, la situation exige du courage et 10 mesures fortes mais on avez-vous. pour avoir la chance de partager avec Madame la première ministre un certain nombre de rencontres avec les différents présidents de groupe, dans le cadre de la réforme des retraites, je peux vous assurer que les partenaires sociaux qui ont a participé je peux vous dire madame la sénatrice que les partenaires sociaux qui ont a participé aux négociations salariales dans les différents secteurs ne se pose pas la question de savoir si Madame la première ministre et de la force et du courage, il ne constatent-ils vide et je peux témoigner des efforts qu'elle met elle-même à à propulser et à promouvoir ce dialogue, je voudrais revenir sur 2 aspects de votre question, 2 aspects de votre question, le 1er concernant les centrales nucléaires comme dans l'ensemble des secteurs nous encourageant la négociation et, aujourd'hui, l'entreprise doit ouvrir un cycle de négociations et nous espérons que ce cycle de négociations sont aussi de nature à dissuader cette grève à l'empêcher et à permettre un bon fonctionnement vous nous interrogez c'est le 2ème point de votre question sur la question des réquisitions, je suis désolé de vous rappeler, Madame la sénatrice, que dans le cadre de du respect des droits constitutionnels, nous sommes évidemment respectueux du droit de grève que la jurisprudence en matière de réquisition est clair que les réquisitions doivent être proportionnées, justifié par un impératif d'urgence ou de troubles à l'ordre public et respectueuse de l'exercice du droit syndical, c'est ce que nous avons fait en veillant à ce que les réquisitions auxquelles nous avons procédé, pour ce qui concerne les raffineries s'inscrivent parfaitement dans ce cadre, c'est ce qui a d'ailleurs permis aux tribunaux administratifs de Lille et de Rouen, de considérer que les décisions prises par le gouvernement était conforme à la loi et qu'elle pouvait ainsi s'appliquer, nous pouvons nous affranchir des règles du droit et parfois même des principes constitutionnels, sauf que cela n'existe pas et que ce serait la meilleure façon d'être, dans dans l'inefficacité avec des décisions qui serait immédiatement censuré par La Tribune, la justice administrative. Madame marché. Mais Monsieur le Ministre, l'impératif et là, il faut agir et agir vite, chaque jour de grève, ce sont plusieurs milliards d'euros perdus pour l'économie française qui viennent creuser encore plus la dette abyssale, la vérité c'est que votre gouvernement est débordé, débordé par ses contradictions débordé par son arrogance débordé par son déni de la réalité par son incapacité à ressentir une quelconque empathie vis-à-vis des Français qui galèrent toujours et toujours plus dans notre pays où règne excusez-moi la chienlit. La parole est maintenant à neutre. Collègues Rachid Temal pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, permettez-moi ici d'être pour quelques instants, le porte-parole des régions, des départements, des interco des villes et des villages, d'autres pays, ces ces collectivités qui encore une fois, sont très largement impacté par l'inflation et qui voient leurs coûts, multiplié par 8 à cette date, rappelons quand même que ces collectivités représentent 70 %. De là son public entre pays et donc ce soir le ravissement ça des pans entiers de notre économie qui s'effondreraient et des emplois qui seraient détruits. Rappelons qu'ici sont donnés sur ces bons, là nous sommes tous à travailler au quotidien avec les élus, avec les associations d'élus, nous l'étions d'ailleurs, nous-mêmes, nous étions d'ailleurs dans le Val-d Oise, ce week-end avec mes collègues ici présents et qu'est ce qu'on constate chez les élus locaux que nous rencontrons d'abord pour la première fois il n'arrive pas à boucler leur budget, c'est une première, ils nous disent qu'ils sont aujourd'hui dans l'obligation de s'interroger sur la fermeture de service sur la suppression de poste et on ne peut qu'imaginer les Français qui, dans quelques semaines, quelques mois, iront à l'dans leur piscine dans leur gymnase et trouveront porte Close parce que il n'y aura pas pour les cocotiers, les moyens d'ouvrir, de les financer, alors Monsieur Miss, la question est relativement simple. Qu'entendez-vous modifié dans votre projet de loi de finances 2023 sur les collectivités pour qu'enfin elle s'est lycée puisse fonctionner dignement et répondent au service public, je vous remercie. On nous répondent la parole les au ministre de la transition. écologique la cohésion des territoires Monsieur Béchu. Monsieur le Président Madame la première Ministre Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, tu es mal. Les élus que vous avez croisé dans le Val-d Oise, les membres du gouvernement les députés, les sénateurs des autres groupes les rencontres aussi et personne ne peut nier que ce retour de l'inflation, à des niveaux que nous n'avons pas connu, même si elle est plus faible en France qu'ailleurs, elle n'est pas dans les équations dont nous parlons, à cela s'ajoute la question de l'énergie, et puisque vous vous êtes fait le porte-parole des départements, des régions, des villes et des villages, je veux quand même rappeler que les villages de ce pays sont protégés par le bouclier tarifaire qui est le même que celui qui vaut pour les ménages. Je vais donc me concentrer sur les autres strates de collectivités, Première chose : si l'inflation pèse sur les dépenses, elle contribue parfois aux recettes, la progression des recettes de TVA des régions, c'est 9 % pour l'année en cours, la revalorisation des bases d'imposition, c'est plus un virgule 2 milliards et la revalorisation automatique, ce sera davantage l'année prochaine 2ème chose des difficultés de bouclage pour les Budgets des collectivités locales on ont connu quand tu des gouvernement que vous souteniez ont baissé de 11 milliards la DGF il y a de cela quelques années, pour la première fois depuis 13 ans. Un gouvernement, celui qui est dirigé par Élisabeth Borne propose de revaloriser le montant de la DGF de 200 puis 320 millions et c'est si vous seront présentés dans quelques jours, quatrièmement, un filet de sécurité autrement plus robustes et plus solide que celui que vous aviez contribué à construire pendant le PLFR sera inclus dans le PLF qui vous sera transmis et ça n'est que la 2ème étape de notre grande bataille qui consiste d'abord à obtenir une baisse des prix de l'énergie, c'est ce qui se joue demain et après-demain au Conseil européen et la réflexion plus que la réflexion l'établissement d'un dispositif de protection tarifaire pour les collectivités pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par le TRV à ce stade, on se bat à l'échelle européenne de on utilise. La contribution sur les rangs pour solvabiliser des dispositifs de compensations trois on ne prévoit un filet de sécurité plus plus plus pour compenser ce qui reste. Très bien monsieur le Ministre, je ne suis pas certain que le le maire déchu tiendrait les mêmes propos vous. Et je vous rassure, j'ai bien indiqué dans ma question que je parlais au niveau de pour tous les bancs, je ne parlais pas que de mes amis politiques, je parlais de tous les bancs, je crois que tous les sénateurs théâtre ici rencontre les même quand il rencontre les les vous nous parlez des villages, tant mieux, mais quand tu te rends compte, les maires des villages, ils nous disent la même chose et je vous rappelle que vos dispositif est que 45 millions de Français ne sont pas inclus dans vos mesures et donc ils vont être pénalisés aussi, donc la question, on peut toujours tourner en rond mais aujourd'hui ce qu'on propose simplement les associations d'élus, toutes les communes. Pour toutes les communes et qui n'impacte pas non plus leur capacité à investir dans l'avenir, ça on pouvait au moins la l'accepter ou pas, c'est ça la vraie question qui nous est posée, et puis il y a aussi la question des bases locatives etc vous nous parlez de mesures mais je vous rappelle, je vous rappelle que vous retirez la CVAE c'est 8 milliards de moins pour aussi pour les collectivités. La parole est à notre collègue Thierry Magnin pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président Madame la première ministre des dames et messieurs les milices, cher collègue, Monsieur le Ministre, la réponse que vous avez apporté à mon collègue : tu es mal ne nous satisfait pas, je voudrais vous rappeler que, comme vous le savez, au 31 octobre les contrats d'électricité et de gaz se termineront pour de nombreuses collectivités territoriales et les nouveaux contrats devront être signés au 1er novembre c'est-à-dire dans quelques jours, sous peine de coupure totale. Ces régions ces départements ces villes devront donc acheter l'électricité et le gaz au prix du marché dans un contexte, dans un contexte de flambée des prix de l'énergie, de nombreux élus locaux vous ont d'ailleurs alerté sur ce point, chez nous, en Seine Seine-Saint-Denis on nous annonce des prix tout à fait insupportable une multiplication par 15 des prix du gaz 32 du prix de l'électricité en Seine-Saint-Denis, comme partout en France, une commune moyenne passerait donc de 2 à 15 millions d'euros en terme de dépense d'énergie. Comme nous on avait pris l'habitude lorsqu'il s'agit des collectivités territoriales et des élus locaux, votre réponse n'est pas à la hauteur, monsieur le Ministre, le ministre des Comptes publics, il a proposé une aide 438 millions d'euros largement insuffisantes, s'il avait s'il n'avait ouvertement souhaité afficher son mépris pour les mères et il ne s'y serait pas pris autrement. Surtout, cette aide de s'appliquera qu'aux communes dont l'épargne brute s'est fortement dégradée ces dernières années, comme d'habitude, vous avez choisi de sanctionner d'abord les bons élèves, les communes qui gèrent correctement l'argent de leurs administrés. Monsieur le Ministre vous demander beaucoup d'efforts aux collectivités et aux entreprises, aux Français, vous avez demandé aux salariés de porter des cols roulés dans les bureaux, vous avez demandé aux écoliers de grelotter dans les salles de classe, les Français ont consenti beaucoup d'efforts, ils ont constitueront ils ne doivent pas être les seuls à consentir ces efforts, Monsieur le Ministre, que répondez-vous aux nombreux maires qui le savent pas aujourd'hui comment ils feront face à la flambée des prix de l'énergie doivent-ils sacrifier les services à la population pour payer leurs factures de gaz et d'électricité. Pour vous répondre, la parole est au ministre de. Ils sont écologiques et de la cohésion des territoires Monsieur Béchu. Monsieur le Président Madame la première Ministre Mesdames et messieurs les sénateurs, vous avez utilisé un mot que je n'aurais pas choisie. C'est le mot de mépris, il y a plusieurs manières de mépriser les gens, et une de celle-là, c'est d'être dans l'outrance dans la caricature et de faire en sorte de présenter les choses d'une manière qui soit totalement dévié. On peut avoir un débat. Il peut être respectueux et il veut surtout reposé sur des réalités, la réalité c'est que pour la première fois depuis 13 ans, il y a une augmentation de la DGF elle a pas été désindexer par l'actuel gouvernement, elle a été par la majorité de la du Sénat, qui se trouvait de ce côté-ci, et elle a été PC ensuite par celle-là, donc, à un moment, revenir à la réalité, c'est une nécessité sur les tarifs sur les tarifs, la a présenté ce que sont les tarifs une démultiplication par 15 ou par trente, c'est en dehors de ce qui se pratique partout et là, le conseil, c'est de ne pas signer sur des niveaux qui sont délirants d'opérateurs qui profitent de la situation dans laquelle nous trouvons. Petr si votre part en terme, je ne peux pas croire. Que vous passiez votre temps dans vos départements à relayer des fausses informations ou à alimenter une inquiétude au lieu d'insister sur les dispositifs qui peuvent exister, le rendez-vous mesdames et messieurs les sénateurs. C'est simple. les choses sont assez simples. Se faire applaudir au Sénat en disant qu'on ne donne pas assez pour les collectivités locales qui sont bien gérés par rapport à l'État qu'il est mal ça garantit le succès à tous les coups, la réalité c'est la responsabilité, la responsabilité par rapport aux finances publiques que vous ne cessez d'invoquer la responsabilité par rapport à un dispositif qui tienne la route sur le plan européen et de ce point de vue Henri gisait ce qui vous sera proposé et regarder à la fois la robustesse du filet nouveau qui a été conçu et la réalité de hausse de DGF et là on aura un débat sur le fond et pas sur des postures. La parole est à notre collègue Patrick. Dans le groupe Union centriste. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des transport, la voiture électrique est sans conteste la Star du Mondial de l'auto, et pour cause, puisque la vente des véhicules thermiques sera interdite à partir de 2035 si cet objectif se justifie sur le plan environnemental, il fait peser un risque majeur sur l'industrie automobile française en l'état actuel des choses, généraliser la voiture électrique, s'est déroulé le tapis rouge à la Chine, les grands constructeurs européens ont consenti des investissements colossaux pour améliorer les performances écologiques des moteurs thermiques avec le tout électrique, ces efforts sont passés par pertes et profits, nous sommes en train d'offrir une industrie d'excellence à l'Asie aujourd'hui la moitié de la chaîne de valeur du véhicule électrique est encore situés en Asie, la Chine contrôle 56 % de la production mondiale de batterie des batteries dont nous devons importer les principaux composants quand nous les fabriquons ici, résultat : nous ne sommes pas compétitifs, les voitures électriques chinoises de 20 à 30 % moins chères que les européennes, les constructeurs estiment qu'il leur faudra entre 5 et 7 ans pour résorber cet écart 100 des voitures électriques vendues en Europe sont d'ores et déjà fabriqués en Chine et ce ne sont pas les dispositifs d'aide à l'acquisition d'une voiture électrique qui vont les aider la location avec option d'achat ne sera pas possible avant 2024 c'est bien pour cela que vous venez d'augmenter la prime à l'achat qui va passer de 6 à 7000 euros pour les ménages les plus modestes, ce faisant, nous allons massivement subventionné les constructeurs chinois, les États-Unis viennent de réserver leurs incitations fiscales aux seuls véhicules électriques dotés de batteries produites en Amérique ne peut-on pas aussi cibler nos aides sur les constructeurs européens, je vous remercie. On vous répond : la parole est au ministre délégué en charge des transports Monsieur Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Chauvé, vous avez raison d'abord de souligner l'importance de ce Mondial de l'auto, le 1er depuis 4 ans, et de souligner ce qui est sans doute, n'auraient pas été imaginables il y a encore quelques années, comme l'a rappelé le ministre-Lescure qu'il est entièrement consacré consacré pardon aux véhicules décarbonés en particulier aux véhicules électriques, vous avez raison aussi d'alerter sur les risques sur les risques d'atteinte à notre souveraineté et de protection nécessaires notre filière automobile face à ce risque, vous avez de réponses possible, soit nous considérons que le choix de la décarbonation de la transition écologique pourrait être remise en cause, soit nous considérons dans cette hypothèse que nous ne pourrions nous pourrions faire l'économie de l'investissement dans le véhicule électrique massivement et rapidement. Je crois que renoncer à décarbonation relancer la transition écologique renoncer à l'électrification, personne ne le propose. Nous ne vous nous devons alors assumer cette transition, nous devons l'affronter et sans être naïf ni excessivement optimiste: nous avons démontré ces dernières années que affronter cette transition et ne pas la refuser pour se réfugier, si je puis dire, dans le confort du thermique ou du statu quo qui d'ailleurs a montré que la baisse de production était déjà là avant la question de l'électrification, nous avons engagé une réindustrialisation et il y a 5 ans, nous n'aurions pas penser que la France aurait pu vous avez souligné ce point produire commencer à produire des batteries retrouver progressivement et rapidement son indépendance, car le prix dans la République, a fixé ce cap est aujourd'hui crédible, nous pouvons sur les batteries atteindre l'indépendance de production d'ici 2027 la transition électrique, nous devons l'amener en réindustrialiser en investissant en soutenant l'achat de véhicules électriques et en incitant notre filière nos constructeurs et l'ensemble de l'écosystème à produire électrique en France et en Europe, on ne peut pas renoncer à cet objectif, on peut en revanche l'affronter en construisant une filière et c'est possible, votre département de la Seine Maritime le connaît avec les transformations en cours des sites de Renault en particulier, à Cléon et à Dieppe, ce qui paraissait improbable il y a quelques années est en cours relever ce défi de l'industrie ation électrique en Europe, nous pourrons le faire cela nécessitera en effet réformer nos outils de concurrence réformer nos outils de protection commerciale, aller vers la réciprocité et faire en sorte, vous l'avez dit, que les aides que nous devons aux consommateurs et aux constructeurs ne soit pas ciblées vers ceux qui, de Chine, essaie de gagner notre marché aujourd'hui. Merci monsieur le président, oui, toute la réponse était pas à la question, ceci étant, vous avez évoqué le droit européen, je crois que ça mérite de s'y pencher, parce que je voudrais simplement rappeler que, au-delà des discours, les conséquences par ricochet sur l'emploi dans cette filière automobile seront terribles, merci à vous. La parole est maintenant notre collègue. Vincent Segouin pour le groupe Les Républicains, vous avez la parole. Monsieur le Ministre, crise énergétique, difficultés d'approvisionnement et de recrutement, l'industrie et de plus en plus affecté la situation des trésoreries continue de se dégrader dans tous les secteurs et très en deçà de la moyenne de long terme conclusion du rapport de la Banque de France sur la conjoncture en octobre 2022 à ces difficultés se rajoute le remboursement du PGE des charges sociales qui n'ont pas été réclamée depuis 2021 forcément ces charges exceptionnelles sont trop lourdes pour les entreprises et les rendent vulnérables à ce sujet, ici en commission des finances, nous vous avions déjà alerté sur la durée de remboursement des PGE que l'on jugeait incompatible avec la marche des entreprises, alors vous allez me répondent que les entreprises peuvent revoir la durée de remboursement du PGE, à condition de passer par la médiation du crédit oui mais médiation est une entité adossée à la Banque de France, si la réponse est négative, l'entreprise devra rentrer dans une procédure collective, si elle est positive, l'emprunt sera apparenté à une restructuration de la dette et donc considérés comme des empreintes non performants sur le bilan, cela aura donc un impact sur la cotation d'entreprise et quel qu'en soit la taille, bilan : l'entreprise ne pourra plus souscrire aux emprunts bancaires pour innover aussi développer, vous comprenez, alors pourquoi cette option et si peu utilisé et pourquoi bon nombre de chefs d'entreprise réinjectes leur Patrimoine personnel, au risque de tout perdre l'entreprise France tu une moyenne de 6 salariés, toutes tailles confondues, y compris le CAC 40 vous avez entrepris une démarche de réindustrialisation de la France mais ne laissons pas tomber TPE et PME qui se découragent face à cette situation, pensez-vous ré-étaler le PGE sans médiation particulière et à surseoir temporairement le remboursement des cotisations sociales des années antérieures. Pour vous répondre, la parole est. Ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, monsieur Barrot. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur merci pour votre question qui est l'occasion de rappeler à quel point les prêts garantis par l'État, les PGE ont permis au début de la crise de la Covid de sauver notre tissu entrepreneurial avec 140 milliards de prêts consentis dans votre département de l'Orne, ce sont plus de 160 millions d'euros qui ont été prêtés prêtés à plus de 1700 entreprises désormais vous avez raison de le rappeler, se pose la question du remboursement, il n'y a pas de risque systémique identifiée à ce stade sur sur ces, sur ces prêts garantis par l'État puisque le le taux prévisionnel de défauts sur ces prêts est estimé aujourd'hui à 5 % mais évidemment nous sommes conscients qu'un certain nombre d'entreprises dans la conjoncture actuelle, rencontre des difficultés pour les remboursements de ces prêts et c'est la raison pour laquelle ce dispositif qui a évolué tout au long de la crise, a fait l'objet d'une de décisions pour ouvrir des facultés d'amortissement qui ont été prises en juillet 2021 et en février 2022, et en particulier pour les entreprises qui avaient pris un prêt de moins de 50000 euros, elles peuvent se tourner vers le médiateur du crédit, vous l'avez dit, placé auprès de la Banque de France pour celles qui ont souscrit un prêt de plus de 50000 euros, elles peuvent se tourner vers le conseiller départemental de sortie de crise qui va les orienter soit vers une solution de restructuration de leur dette, qu'elle soit PGE ou qu'elle soit une des Urssaf, soit vers une procédure préventive de conciliation, vous avez alerté sur la question de la notation, effectivement, certaines entreprises sont inquiets de voir leur note dégradée, il faut rappeler que pour les entreprises qui font moins de 750000 euros de chiffre d'affaires, celle-ci ne dispose pas d'une notation fille ben il y a donc pas lieu, qu'elle soit dégrader et seule la banque en question sera au courant de la restructuration pour celles qui font plus de 750000 euros, il faut rappeler que la dégradation de la note n'est pas systématique qu'elle fait l'objet d'une d'une analyse au cas par cas par la Banque de France et que la discussion est ouverte et je rappelle en conclusion que ses facultés viennent en complément des décisions qui ont été prises par la première ministre pour venir en aide de manière conjoncturelle à nos TPE et PME face à la hausse des prix de l'énergie, je vous remercie. Monsieur le Ministre, déjà, je suis surpris par rapport à vos compétences que vous répondiez à ma question, première chose la seconde vous ne venez pas vous tenez compte du taux de contentieux, sans tenir compte de la radiation des entreprises qui est de 37 % supplémentaires supérieur à celui du taux de 2019 les entreprises abandonnent aujourd'hui on vous avez prévenu sur le PGE que la durée de remboursement et serait trop courte, c'est simple, votre réponse, c'est circulez il y a rien à voir, hé bien, je suis désolé, vous étiez fier de défendre les entreprises, mais là, vous les mettez dans le décor et sans suivre navré. Merci, la parole est à notre collègue Angel. 13 villes pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, encore une condamnation pour inaction avant- hier, le Conseil d'État a condamné l'État à une astreinte de 20 millions d'euros pour non respect des seuils de pollution de l'air en dioxyde de d'azote dans les grandes agglomérations, Paris, Lyon, Marseille et sur la période du 1er juillet 2021 au 1er juillet 2022 22, l'État avait déjà été condamné il y a un an, pour les mêmes raisons, à 10 millions d'euros cela sanctionne l'insuffisance des mesures et moyens mis en oeuvre pour ramener les émissions de ce gaz sous le seuil de 40 microgrammes par m3 principal émetteur les moteurs thermiques, soit le trafic routier ce gaz le dioxyde d'azote se dissout dans l'eau pour donner de l'acide nitrique, c'est d'ailleurs un procédé de fabrication de la symétrique produit corrosif par excellence, très concrètement, si vous le respirez, mesdames et messieurs les Ministres, hé les mes chers collègues, dans votre nez dans vos poumons qui sont humides, le dioxyde d'azote, va s'dissoudre dans cette humidité et c'est de l'acide nitrique dilué, qui va se former sur les parois de votre nez et dans vos poumons, c'est pourquoi vous allez ressentir des picotements et des irritations et si vous y êtes exposé régulièrement des inflammations avec pour conséquence des quantités de pathologies crises d'asthme, maladies pulmonaires cancer du poumon, les plus vulnérables, les enfants, donc, et les plus pauvres sont les plus touchés, bilan annuel 40000 décès prématurés dans la nature, c'est le même phénomène de formation d'acide nitrique, au contact de l'eau qui provoque plus acide acidification des océans eutrophisation des eaux douces et qui constitue un facteur majeur de baisse de la biodiversité, le trafic routier par camion n'a pas baissé il s'intensifie, le fret ferroviaire n'est toujours pas revenu au niveau des années 80, soit 30 % du transport de marchandises et les mobilités douces ne sont toujours pas suffisamment encouragé, Monsieur le Ministre, pensez-vous que nous soyons sur la bonne voie. On vous réponde, la parole est au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le Président Madame la première Ministre Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice. Nous avons évidemment pris acte du maintien par le Conseil d'État de ses astreintes pour les 2 semestres depuis la condamnation d'août 2021. Je ne doute pas, compte tenu du degré de précision dans lequel vous êtes entré que vous avez lu cet avis du Conseil d'État. Qui pointent le fait qu'il y a un maintien de dépassement de seuil mais une amélioration de la situation en 2017, nous avions 13 agglomérations qui était en dépassement de seuil, ce chiffre est passé à 8 en 2020 à 5 en 2021 et il est de 3 Paris Lyon et Aix-Marseille à la minute où nous parlons, mais le sujet c'est pas le nombre. Agglo, c'est bien d'abord le nombre de décès, plus de 40000 plus de 40000 décès liés à la pollution de l'air et notre engagement, il est de faire en sorte de diminuer ces décès, la ligne du gouvernement c'est la protection des Français, cette protection, elle vaut d'abord sur les sujets environnementaux de façon extrêmement concrètes, ce que le Conseil d'État nous appelle, c'est à amplifier, a renforcé ou à rendre plus efficiente les zones à faibles émissions. Mardi prochain, je recevrai au ministère avec Clément Beaune, les présidents des intercommunalités des métropoles, les maires de toutes les villes de plus de 150000 habitants, pour faire un point sur là où nous en sommes, une dizaine d'agglomérations, ils sont déjà passés, d'autres pas certaines rencontre des difficultés d'autres. Anticipe des difficultés, on a de vrais sujets d'accessibilité sociale parce que les aider feux ne doivent pas être des moyens d'empêcher les plus fragiles d'entrer dans les villes, il y a donc la question des compensations il y a la question des moyens, il y a la question de l'information, il y a des dispositifs innovants avec Strasbourg qui testent impasse avec d'autres qui major des aides ou des primes à la conversion, tous ces sujets seront sur la table, avec un objectif : protéger les Français, améliorer la qualité de l'air, tout particulièrement dans le domaine du dioxyde d'azote et des particules fines. Merci, la parole est à notre collègue Valérie Boyer pour le groupe plairait public hein. Madame la ministre, j'associe à ma question : les amis de la justice et de la liberté, en particulier ceux du groupe France-Arménie le 13 septembre l'Azerbaïdjan a lancé une nouvelle offensive contre l'Arménie, malgré l'indifférence presque générale, c'est bien une nouvelle guerre de conquête et d'extermination qui se joue aux portes de l'Europe avec son premier lot de crimes de guerre fièrement exhiber sur la toile par les militaires azerbaïdjanais ce film dans leurs Oeuvres, de viols, de tortures, de démembrement cette logique, j'ai le sidère cette armée phobies ce racisme d'État pratiquée par l'Azerbaïdjan, avec le soutien de la Turquie n'a pas vocation à s'arrêter à ce pays, il y a, Malia d'ailleurs déclaré vouloir chasser ces chiens d'Arméniens alors Madame la Mini ce que comptez-vous faire concrètement pour éviter que cette part de l'histoire de l'humanité que ce pays souverain, la République d'Arménie ne disparaisse. Et pour la parole est à madame la ministre de l'Europe des Affaires étrangères, Madame Colonna. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Boyer je vous remercie de votre question qui me permet, qui me permet de revenir sur quelques points évoqués récemment ici même la France, vous le savez est pleinement solidaire de l'Arménie face aux violations de sa souveraineté pour stabiliser la situation pour que l'Arménie recouvre son intégrité territoriale et pour accompagner la reprise des négociations cette mobilisation porte ses fruits : outre la relance de la dynamique au Conseil de sécurité des Nations unies, sous présidence française, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont décidé lundi le lancement rapide d'une mission européenne d'observation qui se déploiera le long de la frontière arménienne cela a été rendu possible par l'accord trouvé entre les 2 pays sous l'égide du président de la République le 6 octobre ou, plus exactement, dans la nuit du 6 au 7 octobre car il y a passé un certain temps, comme le souhaitait l'Arménie, par ailleurs, nous avons aussi pu faire accepter une mission d'évaluation de l'OSCE, qui sera sur place dès vendredi et permettra de faire un constat de la situation et des besoins, notamment les besoins humanitaires et visera la relance du processus de négociation et de délimitation de la frontière, je vous avais parlé de ces 3 sujets, ils ont avancé tous trois aucune de ces avancées n'aurait été possible sans l'engagement de la France, jusqu'au plus haut niveau de l'État, madame la sénatrice, donc vous le voyez, l'Arménie, peut compter sur la France et l'oeuvre pour la paix pour la stabilité dans le Caucase, dans l'intérêt de tous, je vous remercie. Voilà moyen. Comment y croire Madame la Ministre, comment croire une Europe qui d'un côté va envoyer cette mission civile sur place mais qui de l'autre, renforce la coopération avec l'Azerbaïdjan, notamment en matière énergétique avec une Ursula von der Leyen, qui va en allié à un partenaire fiable sur lequel on peut compter, Bruxelles est prête à sacrifier la vie des Arméniens sur l'autel de ses intérêts énergétiques, qu'en est-il vraiment de la France, la vie des Arméniens Vautel vaut moins que celle des Ukrainiens cette tartufferie européenne va plus loin puisque le gaz vendu par l'Azerbaïdjan proviendrait d'une exploitation en partie détenue par une société russe l'Arménie est une part de nous-mêmes une part de notre civilisation de notre culture de nos croyances, nous avons même une journée nationale pour commémorer le génocide de 1915 les Arméniens de demande qu'une chose : le droit de vivre le droit de disposer d'eux-même, ce qui est valable pour la Russie devrait l'être pour l'autocratie azéri il y a d'ailleurs une entente entre ces 2 pays Poutine veut prendre la géographie Aliev veut annuler l'histoire le 1er conquiert le second efface dit justement Sylvain Tesson ce grand témoin, demandant des sanctions contre l'Azerbaïdjan et appliquons-les madame je long les avoirs du clan Aliev sans avoir la main qui tremble ou qui trichent opposons-nous à la diplomatie de la menace à la caviar Connection envisageant un soutien militaire pour l'Arménie des armes pour l'Arménie, ce que nous avons fait pour le Mali, pourquoi ne pas le faire pour l'Arménie et dénonçons cet accord inique sur le gaz qu'a refusé ces sanctions c'est cautionner cautionner l'épuration ethnique des Arméniens, une nouvelle phase du génocide peut être la solution finale, pour eux, malheureusement c'est clamer au monde que les valeurs dont nous nous réclamons ne sont que des supercheries alors agissons concrètement. La parole est à notre collègue Laure Darcos dans le groupe des Républicains. Merci monsieur le président, ma question s'appelle s'adresse à monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, monsieur le Ministre, la République a toujours besoin de savon, elle doit donc commencer par favoriser les pépinières scientifique : la réforme du lycée a été bâclé avec comme seul objectif, une économie de moyens, 2 ans plus tard, le bilan que nous pouvons adresser hé bien inquiétant : oui, l'heure est grave, Monsieur le Ministre, c'est toute une filière qui est en train de couler, nous ne formons plus à de scientifique, alors même que la France a fait le choix de réinvestir massivement dans la recherche publique et l'innovation en 2 ans entre 2000 19 et 2021 le nombre d'élèves scientifiques en terminale, a diminué de 24 % les élèves bénéficiant d'un enseignement renforcé en mathématiques sont de moins en moins nombreux, la part des jeunes filles dans l'ensemble des parcours scientifique est aussi en chute libre 20 ans d'efforts pour les amener à s'engager dans des formations exigeantes autrefois largement réservé aux garçons ont été balayés d'un trait de plume. Les mathématiques, la physique, la chimie, le numérique, les sciences informatiques, les sciences de l'ingénieur ont tous disparu du tronc commun et sont aujourd'hui reléguées au rang d'enseignement de spécialité ou d'enseignement optionnel en première et en terminale, les mesures annoncées à la hâte à la fin de l'année scolaire 2021 2022 ne sont qu'un écran de fumée, vous ne pouvait pas décemment former un ingénieur en lui enseignant une heure 30 de mathématiques dans le tronc commun en première et 3 heures d'option mathématiques complémentaires pour tous en terminale, c'est toute la structure du style terminal qu'il faut revoir sans délai si nous voulons répondre à l'exigence scientifique des formations du supérieur et produire les compétences dont dépend notre et notre économie, ma question est simple, monsieur le Ministre, elle dictée par l'urgence, allez-vous suspendre cette réforme et réunir toutes les parties prenantes afin de réfléchir à la mise en oeuvre de solutions efficaces et durables pour renverser ce déclin dès la rentrée 2023, à défaut, je crois que notre compatriote Hugo Duminil Copin qui a reçu en juillet dernier la médaille Fields pour ses travaux en physique statistique et qui travaille à Bures sur Yvette dans mon département, soit le dernier Français à recevoir cette prestigieuse récompense je vous remercie de votre votre avoir été ministre de l'Éducation nationale de la jeunesse, j'ai pas d'ailleurs. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Laure Darcos, je vous remercie de cette question qui m'offre l'occasion de souligner 2 points le 1er commence par un paradoxe : l'école française de mathématiques comptent parmi les meilleurs du monde, c'est un sujet de fierté pour notre pays 13 médailles Fields des prix Nobel scientifiques y compris cette année et d'un autre côté, un niveau moyen en mathématiques médiocre dans la population générale, et aussi dans la population scolaire française, on le voit aux évaluations nationales mais aussi aux classements internationaux ou la France ou la place de la France en mathématiques, du côté des populations scolaires n'est pas reluisante face à cela, nous avons d'abord de façon rapide réintroduit une heure et demie de mathématiques dans le tronc commun pour les élèves de 1ère cela obéissait à une demande insistante des sociétés de mathématiques et nous l'avons fait nous allons poursuivre cet effort l'année prochaine, mais je le reconnais, cela ne suffit pas, il faut avoir un regard global sur l'enseignement des mathématiques qui ne dépend pas du volume d'heures mathématique, car la France se situe plutôt dans le haut du panier en la matière, en revanche, quand on regarde les résultats, on voit que c'est un accord cela ne correspond pas évidemment à ce volume d'heures et donc on a bien un sujet qui est le sujet de la pédagogie de l'enseignement des mathématiques comme le rapport Torossian Villani La soulever de façon très claire,

et 2021, c'est pourquoi je vous annonce pour réfléchir et prendre des mesures fortes en la matière, je sais que la première ministre est très motivé par cette question, la tenue d'Assises nationales sur la place des femmes dans l'enseignement et dans le monde scientifique, cet Automne, avec mes collègues, Ministre de l'enseignement supérieur et de l'égalité femmes-hommes pour prendre les mesures qui s'imposent, je vous l'accorde, c'est désormais une priorité pour nous, nous devons en tenir compte dans les retouches que nous allons faire de la réforme du lycée. Merci, nous en avons terminé avec les questions d'actualité, les prochaines auront lieu mercredi 26 octobre je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 16 pour l'examen de la proposition de loi constitutionnelle visant à protéger à garantir le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse et la contraception n'a séance est suspendue.

lors du scrutin d'hier sur le le scrutin numéro 5 sur le la proposition de loi relative aux étudiants internes en médecine, je souhaitais m'abstenir et j'ai été porté comme votant pour et je voulais signaler pour le procès verbal que il en va de même de mon collègue Michel Dagbert. Dagbert. Et j'ai donné la parole à Madame Guilaine Pontaillet pour également pour une mise au point au sujet d'un vote. Merci madame la présidente, donc je vous remercie de bien vouloir noter que lors du scrutin, numéro 3 je souhaitais voter pour merci. Merci a été donné de ces mises au point, elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans l'analyse politique des scrutins, mes chers collègues par courrier en date du mardi 18 octobre monsieur le Président, Guillaume Gontard, président du groupe écologiste solidarité territoire demande que le projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et la République italienne pour une coopération bilatérale renforcée, inscrit à l'ordre du jour du jeudi 27 octobre à 10 heures 30 soit examiné selon la procédure normale et non selon la procédure simplifiée acte données de cette demande dans la discussion, je général nous pourrions attribué un temps de 45 minutes aux orateurs des groupes le délai limite pour les inscriptions de parole serait fixée au mercredi 26 octobre à 15 heures il y a pas d'opposition en est ainsi décidé, en application du 5ème alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique et de la loi ordinaire du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des finances, a émis lors de sa réunion du mardi 18 octobre 2022, un avis favorable 20 voix pour, une voix contre à la nomination de Madame Marianne Barbat Layani à la présidence de l'Autorité des marchés financiers, la parole est au président Patrick Kanner pour un rappel au règlement. Oui merci madame la présidente, très très simplement, nous allons aborder dans quelques instants, une proposition de loi extrêmement importante, très symbolique, qui est celle de la constitutionnalisation de l'IVG donc dans notre texte fondamental une un moment important, qui d'ailleurs a fait l'objet d'un avis favorable historiquement de la part du gouvernement et nous savons dans quel contexte nous allons aborder cette discussion, un contexte de remise en cause de ce droit et dans de nombreux pays et y compris des pays européens, donc il ne faut passer du temps, il ne faut passer de l'énergie et il faut surtout de la conviction en la matière et je regrette très simplement que, au même moment, nous ayons plusieurs commissions 3 commission je crois qu'sur une liste dont la commission des affaires sociales, je pense qu'il est récemment président Larché sur un autre débat, le débat concernant le les droites et femmes iraniennes et leur combat et nous sommes aujourd'hui dans la même situation, donc je souhaite vraiment, même si je sais que nous travaillons beaucoup qu'il y a beaucoup de dossiers, aujourd'hui en cours au sein de notre haute assemblée je souhaite vraiment qu'il et le ministre-Brown qui est aussi concernée par définition qui est là, donc ce sont des moments importants que beaucoup de nos collègues vont devoir se priver en se partageant entre les travaux de commission et notre séance plénière, donc je voulais faire ce rappel au règlement et je ne doute pas que nos collègues du groupe écologiste et et du groupe geste pardon seront aussi associés à cette démarche, par le biais de leur président, je vous remercie.

des textes importants avec l'IVG, l'inscription de l'IVG dans la Constitution, qui va demander du débat qui est particulièrement regardez et observez un texte sur le droit des, des sages-femmes, et c'est vrai que dans le même moment et dans cette niche de 4 heures, on a l'audition notamment du du ministre de la santé, mais pas que puisqu'on a 2 autres commission qui auditionne des ministres, donc c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on préserve ce travail parlementaire qu'on préserve aussi la question du travail dans les, dans le cadre des des niches, donc voilà moi j'en appelle à la fois aussi notamment au président et présidente et président de de commissions pour qu'il soit attentif et que on essaye pour les prochaines fois, de faire en sorte qu'on n'ait pas que nos collègues n'est pas des des choix particulièrement insensé, voire complexe affaire entre aller en commission ou suivre ce débat particulièrement important, merci. merci, ah que donner de votre rappel au règlement. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et pardon et à garantir le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, présenté par Madame Mélanie Vogel et plusieurs de ses collègues discussion générale, la parole est à Madame, Mélanie Vogel, autrice de la proposition de loi constitutionnelle et pour dix minutes chers collègues. Merci madame la présidente, monsieur, madame la ministre, madame la rapporteure chers collègues. Nous sommes réunis aujourd'hui pour répondre à une question d'une simplicité extrême est d'une importance majeure le monde, partout dans le monde, les forces réactionnaires progressent à l'heure où les droits des femmes, les droits reproductifs et sexuels sont partout attaqué à l'heure où en Europe, les femmes se préparent à la contre-offensive, à l'heure où la France peut retrouver un rôle de pionnière de modèles et d'espérance, nous devons répondre à une question préférons-nous une société où le droit à l'avortement et protégé au sommet de la hiérarchie des normes ou une société ou une simple loi peut le défaire, préférons-nous agir aujourd'hui au risque au pire que cette garantie ne se révèle jamais nécessaire ou ne rien faire, au risque de balayer le droit fondamental des générations futures, voulons-nous réponde positivement à 80 pour 100 des Françaises et des Français, toutes catégories sociales préférences politiques appartenances religieuses confondues, qui demande que le droit à l'avortement soit reconnue dans le texte qui fondent notre contrat social ou non, souhaitons-nous dire à toutes les femmes de ce pays que le Parlement et de leur côté que l'honneur de la France, c'est son idéal d'égalité c'est de considérer que la maîtrise de sa femme, de sa fécondité est une affaire de liberté mais aussi simplement une affaire de citoyenneté, d'égalité des droits et que pour cette raison, nous les régions au sommet de nos normes souhaitons nous montrer à toutes les femmes du monde à toutes celles et ceux qui se battent si nombreux et si nombreux contre le fascisme contre l'autre autoritarisme redis je celui des mollahs iraniens des évangélistes texan où des intégristes bien français à toutes celles et ceux qui, en Pologne, en Hongrie, en Italie, aux États-Unis, en Iran, au Maroc, à Malte dans tant de pays se battent pour avoir le droit d'être considérés comme des être s'humains qui disposent de leur corps et au fond de leur destin et de leur vie, que non, tout n'est pas perdu que dans cette période si sombre, il existe dans ce monde un chemin, un chemin de progrès dans lequel notre pays, a fait le choix de s'engager et dans lequel il invite les autres nations elle rejoindre le droit à l'avortement est un acquis féministes et comme tous les acquis féministes, il n'est jamais hors de danger j'mais c'est aussi un acquis profondément républicain parce qu'il répond à la promesse républicaine et universaliste d'égalité des droits, un acquis qu'il vous est simplement proposé aujourd'hui de mieux protéger où trouver l'envie en 2022 d'argumenter contre une loi qui ne ferait rien d'autre que de sanctuariser un droit que prétendument nous chérissons toutes et tous ces je vous l'assure pour tellement de personnes qui nous regardent un profond mystère je remercie évidemment madame la rapporteure pour son travail, je sais que cela n'a pas toujours été le travail le plus facile, mais je voudrais revenir sur les arguments utilisés pour refuser cette loi premièrement l'argument classique, ça ne sert à rien, d'abord parce que ce droit n'est pas menacée, donc c'est un peu comme dire je suis dans ma voiture, ça sert à rien que je mette ma ceinture parce que je ne suis pas en train d'avoir un accident, cet argument n'a évidemment aucun sens parce que par définition, on se protège d'un risque avant qu'il advienne, mais aussi parce qu'on le sait très bien le jour où il aura un risque concret en France, c'est-à-dire quoi un nombre conséquent d'élus tentés de remettre en cause ce droit, hé bien ce jour là une protection constitutionnelle sera par définition hors de portée, puisque la majorité pour changer la Constitution est supérieure à celle pour changer la loi et que c'est précisément pour ça que nous voulons l'inscrire dans la Constitution, c'est donc exactement parce qu'il existe aujourd'hui en France une écrasante majorité dans les urnes dans la rue, dans les institutions pour le droit à l'avortement que l'on peut et que l'on doit le protéger maintenant, deuxièmement, ça ne sert à rien, parce que c'est pas une protection absolue la constitution, on peut toujours la modifier, donc là c'est je mets pas ma ceinture de sécurité parce qu'on ne sait pas, il peut y avoir un tsunami alors c'est pas faux, on est jamais à l'abri d'un putsch d'une révolution d'un astéroïde qui la France donc je suis même pas tout à fait sûr de savoir, au fond, pourquoi on a une constitution des élus qui se lève le matin pour légiférer, de toute façon, il y a des gens qui viole la loi tous les jours et il y a des élus qui change la loi, en permanence, donc on a quand même d'un côté, ça sert à rien parce qu'il y a pas de risque et de l'autre, ça sert à rien parce que le risque, il est trop grand, donc c'est un peu difficile à suivre, mais c'est pas fini 3ème argument, ça ne sert à rien, parce que c'est déjà protégé par la Constitution, donc en fait je ne dois pas mettre ma ceinture parce que je l'ai déjà il faut surtout pas mettre la ceinture parce qu'il y a pas de risque, le risque est trop grand et, finalement, mesdames et messieurs, parce que heureusement, je l'ai déjà donc c'est assez épatant et là encore, le problème c'est que c'est faux, la jurisprudence du Conseil constitutionnel n'a jamais dégagé de manière positive un droit à l'interrupteur interruption volontaire de grossesse, jamais, elle s'est contentée d'affirmer que les différentes lois qui encadrent de droit à l'IVG ne violait pas la constitution et les fin juriste que vous êtes connaissent très bien la différence si demain et ça, toutes les personnes qui nous écoutent doivent le savoir : si demain une loi régressive qui viserait à réduire les délais légaux à dérembourser a ajouté des conditions pour accéder à l'avortement a imposé une ordonnance pour accéder à la pilule du lendemain, venait à être présenté devant le Conseil constitutionnel, ce dernier n'aurait rien pour statuer sur son inconstitutionnalité rien et c'est ça que nous voulons corriger argument suivant : ça ne va rien changer parce que l'important est ailleurs, comme toujours, ce n'est pas le droit, c'est l'accès au droit, alors déjà j'aimerais vous dire une chose : on n'a pas accès à un droit qui n'existe plus et puis quel est le rapport, cette loi va non seulement permettent de réclamer un meilleur accès partout, mais surtout elle ne vous empêchera pas, je vous l'assure : jamais, bien au contraire, de voter pour l'augmentation des crédits pour les associations et les centres de soins, pas du tout argument suivant la constitution ne doit pas être un catalogue et n'a pas à protéger les Français contre des changements, par exemple, faire reculer le droit à l'avortement qu'il pourrait démocratiquement vouloir demain, hé ben si parce que dans ce cas-là, à quoi ça sert d'avoir une constitution et un bloc de constitutionnalité, à quoi ça sert de protéger le caractère laïc de la République notre attachement au préambule de 46 l'interdiction de la peine de mort a rien dans ce cas-là, le dernier argument et je j'avoue, c'est un peu mon préféré, il ne faut pas importer des débats des États-Unis. Comme si il n'y avait que aux États-Unis qu'on attaqué le droit à l'IVG à côté, une proposition de loi vient d'être déposée par la droite, pas par l'extrême droite par la droite pour restreindre le droit à l'avortement, mais en France on serait nationalement immunisé, puis je trouve que nous avons d'un côté, cet hémicycle une haine très sélectif des importations de débat en particulier venant des États-Unis, parce que quand il s'agit d'importer des débats totalement construit au sujet d'un prétendu danger causé par un prétendu, concept dont personne ne se réclame en France et que personne n'est capable de définir, c'est bien, mais quand les débats prétendument moins à propos de risques bien réels peuvent générer des progrès bien réels, là c'est mal alors admettons mettez-moi de côté mais Laurence Rossignol qui le porte depuis 2012, Éliane Assassi Laurence Cohen qui, dès 2007 5 ans avant l'arrêt de la Cour de suprême avait déjà fait cette proposition daphné Ract-Madoux Xavier Iacovelli Maryse Carrère Joël Guerriau je que je remercie une fois encore, ces gens-là ne sont pas importés, hein, je suis désolé, ils sont bien ici et il pose ici au sénat français une question bien française, la France a en son coeur, des femmes qui, depuis des siècles, se battent pour conquérir leurs droits à elle et, par là même pour protéger les droits tout court, alors je vais vous dire une chose : s'il devait y avoir aujourd'hui une spécificité française, ce ne serait pas d'être prétendument le seul pays pays au monde protégé des reculs, ce serait au contraire de devenir le 1er pays au monde, a décidé d'agir en amont plutôt que de réagir quand il est trop tard, en tant que co-présidente du Parti Vert européen partageant ma vie avec une féministe allemande qui se bat depuis toujours pour qu'en Allemagne l'avortement soit du droit du code pénal, je peux vous dire une chose, vous mesurez très mal, très mal l'importance pour l'Europe entière du vote d'aujourd'hui la force que cela donnerait à des millions de défense des 2 défenseurs des droits humains, elles ne peuvent être méprisés par le pays qui se veut celui des droits universels, j'ai passé ces dernières semaines des jours et des nuits à chercher quels arguments marche le mieux pour convaincre la droite sénatoriale de voter ce texte au nom de ce que je crois être le sens profond de notre mandat, et puis je me suis dit qu'en fait c'était à vous de convaincre de convainc les Françaises et les Français que le droit à l'avortement et pour vous, vraiment un droit fondamental, vous avez la majorité c'est vrai une victoire aujourd'hui serait la vôtre est un échec aussi. Je voudrais finir en m'adressant à toutes les personnes mobilisées qui nous écoutent et qui attendent de nous que nous les protégions je veux vous dire je ne sais pas si on va y arriver aujourd'hui, mais je sais qu'on y arrivera un jour et je sais que ce jour tous ceux qui s'opposent aujourd'hui à ce progrès l'applaudiront très fort en seront très tandis qu'ils seront encore très occupé ahan freiner d'autres alors ne lâchez rien, jamais, c'est vous, par votre mobilisation qui depuis toujours, écrivez l'Histoire et en particulier l'histoire des combats, des droits des femmes, je vous remercie. Merci, la parole est à Madame Agnès Canayer, rapporteur de la commission des lois pour dix minutes. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, Madame la Ministre, Monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, le droit à l'interruption volontaire de grossesse et la contraception font partie intégrante de notre Patrimoine juridique fondamental ses acquis ont été obtenus grâce au courage et à l'engagement de Simone Veil et de Lucien Neuwirth qui se sont battus avec détermination pour les faire inscrire dans la loi aujourd'hui ces droits sont pleinement protégés par le droit positif, le Sénat s'est toujours montré fortement attaché à ses libertés de la femme, depuis la loi du 17 janvier 1975 la liberté d'interrompre sa grossesse n'a cessé d'être conforté par cette fois, le législateur a renforcé avocat encore récemment l'allongement du délai à 14 semaines quant à la contraception, consacré par la loi du 28 décembre 1967 son accès n'a cessé d'être étendu au fil des années la contraception est délivrée gratuitement pour les mineurs, depuis cette année, elle est pour toutes les femmes de moins de 26 ans, et à partir de 2023 la Debs exception d'urgence sera gratuite pour toutes les femmes aujourd'hui à ma connaissance personne dans cette assemblée ne veut revenir sur ces avancées, la proposition de loi constitutionnelle dont nous avons à débattre aujourd'hui et partez et porté par notre collègue Mélanie Vogel et co-signé par 118 sénateurs, elle a été introduite en réaction à l'actualité américaine marquées par le revirement de la jurisprudence de la Cour suprême du 24 juin dernier d'Obs versus Jackson, cette proposition de loi constitutionnelle tend à inscrire au titre 8 de la Constitution un article 66 de qui affirme : nul ne peut porter atteinte au droit à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, la loi garantit à toute personne qui en fait la demande, là c'est l'accès libre et effectif à ces droits selon les auteurs, cette inscription vise à garantir un accès effectif libre et inconditionnel à l'IVG, ainsi qu'à la contraception et à prévenir de toute régression si l'on peut comprendre l'émotion suscitée outre-Atlantique par la jurisprudence de la Cour suprême, la révision constitutionnelle ne peut être en France, une réponse pertinente, tout d'abord, il n'y a pas lieu d'importer en France un débat lié à la culture américaine et à la nature fédérale des États-Unis, ce débat n'est pas le nôtre, la situation institutionnelle en France n'est en rien comparable à celle des États-Unis, contrairement à ces derniers, la République française et une et interdit autrement dit les lois Veil et Neuwirth ce qui ce ne sont pas remises en cause aujourd'hui en France s'applique de manière identique sur tout le territoire, la question centrale en France reste l'effectivité de ses droits, seules des mesures concrètes, comme la lutte contre les déserts médicaux, notamment en milieu rural, la valorisation des actes médicaux des personnels soignants pratiquant l'IVG, l'augmentation des moyens, des plannings familiaux permettront le plein accès à ces droits, mais ces mesures relèvent du domaine réglementaire, l'inscription dans la Constitution n'est donc pas la réponse adaptée pour renforcer la garantie de ses droits inscrits dans notre Patrimoine juridique, l'IVG, le droit à la contraception, font déjà l'objet d'une protection constitutionnelle solide et durable, solide, car l'IVG est inscrite dans notre droit, depuis 1975 le Conseil constitutionnel, la toujours jugées conformes à Caen de la Constitution et par 4 fois, s'est prononcé en faveur de ce droit en 1975 en 2001 en 2014 en 2016, l'IVG est aujourd'hui une composante de la liberté de la femme découlant de l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui se concilie avec le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, comme contre toute forme de dégradation plus que solide, cette protection est durable, comme le témoigne la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel qui a toujours considéré que bien que le législateur dispose de larges marges de manoeuvre pour définir les conditions d'exercice d'un droit ou d'une liberté, il ne peut en remettre en cause son effectivité, c'est le fameux effet artichauts que nous devons doyen Favoreux on ne peut toucher au coeur des droits et des libertés reconnues d'ailleurs en 2018 Agnès Buzyn et Nicole Belloubet alors ministre, avait affirmé devant le Parlement l'inutilité d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution en l'ex-en les raisons de l'extrême solidité de sa protection constitutionnelle 4 années plus tard, la proposition de loi constitutionnelle dont nous débattons ce jour comporte toujours des risques, largement supérieur à la seule portée symbolique, recherché par les auteurs, l'inscription dans la constitution du droit à l'IVG à la contraception, tente à dénaturer l'esprit de la Constitution et à ouvrir une boîte de Pandore en effet la constitution voulue par le général de Gaulle est avant tout un texte qui régit le fonctionnement de nos institutions, en faire un catalogue de droits, risque de porter atteinte au rôle protecteur de la norme suprême et à minorer la portée de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, gardien de nos droits et de nos libertés en 2008, Simone Veil, présidente du comité de réflexion sur le préambule de la Constitution recommandé elles-mêmes de ne pas modifier le préambule ni d'intégrer dans la constitution des droits et des libertés, liés à la bioéthique qui intégré d'IVG, elle préconise clairement le refus d'inscrire des dispositions de purement de portée purement symbolique : seuls 4 raisons justifient une modification de la Constitution pour introduire un droit nouveau pour déroger à un principe que la Constitution impose ce fut le cas en 1999 et en 2008 pour autoriser la parité pour ratifier un engagement international, l'inscription dans la peine de de dans la constitution de la peine de mort en 2007 était nécessaire pour entériner le Pacte international des droits civils et politiques pour revenir quatrième raison sur une interprétation jurisprudentielle du Conseil constitutionnel, comme en 1993 pour le droit d'asile, l'objet de la proposition de loi soumise à notre examen ne se peut se rattacher à aucune de ces raisons de plus, force est de constater qu'il n'existe aujourd'hui aucun consensus sur la manière de constitutionnaliser l'IVG et le droit à la contraception, 6 propositions de long de loi constitutionnelle ont été introduites à l'Assemblée nationale et au Sénat, en réaction à l'actualité américaine chaque fois qu'une propose une version différente l'inscription par défaut dans le titre 8 de la Constitution prévue par plusieurs propositions de loi constitutionnelle dont celle de la sénatrice Vogel n'est pas satisfaisante, l'intégration du droit à l'envers à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception au sein du titre consacré à l'autorité judiciaire, juste après l'abolition de la peine de mort, a de quoi surprendre et pourrait créer une possible interférence du juge dans le droit des femmes à avorter, ce qui n'a pas lieu d'être des propositions de rattachement à l'article 1er ou l'article 34 de la Constitution relatif aux compétence du législateur ne font pas plus consensus auprès des constitutionnalistes, de plus, la formulation soumise à notre examen s'ouvrent, lève des difficultés importantes, elles, laisse entendre que l'accès à ces droits seraient inconditionnel, or le législateur doit pouvoir en fixer les conditions comme pour toutes les libertés publiques, enfin, une procédure de révision constitutionnelle, à l'initiative des parlementaires impose le recours au référendum conformément à l'article 89 de la Constitution, or il existe un risque réel que cette initiative se retourne contre les droits qu'elle est censée protéger comme nous, ont alerté toutes les personnes auditionnées, y compris des auteurs recourir au référendum mettrait au coeur d'une actualité bouillonnante un sujet pour lequel il n'y a pas de remise en cause et pourrait réveiller un réveil et pourrait n'oublions pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions pour toutes ces raisons, la commission des lois vous propose ne pas adopter. Cette proposition de loi constitutionnelle. Merci, la parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la justice.

Madame la présidente, madame le Ministre. Chère Isabelle. Monsieur le président de la commission des lois. Madame la rapporteure. Madame la sénatrice Mélanie Vogel, mesdames et messieurs les sénateurs. L'histoire, je le crois profondément fourmille. L'exemple de liberté de droits fondamentaux conquis au prix du sang. Des larmes. Que tous croyaient définitivement acquis. Et qui, dans la stupeur. Ou l'indifférence ont été balayés comme des fétus de paille. C'est d'ailleurs l'histoire de la femme qui nous offre. Les plus cruels exemple car oui. Les premiers droits qui disparaissent sont souvent ceux des femmes. Et c'est ce que nous rappelle la décision de la Cour suprême des États-Unis. Le droite à l'avortement qu'on croyait acquis depuis 50 ans. En réalité, ne l'était pas. Désormais. Dans cette grande démocratie, l'interruption volontaire de grossesse n'est plus un droit garanti par la Constitution fédérale et les États fédérés sont libres de l'interdire ou de la légaliser. Cet exemple rend plus que jamais, criant de vérité, les célèbres mots de Simone de Beauvoir, rapportée par Claudine Monteil n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique, religieuse, pour que les droits des femmes soit remise en question, ces droits ne sont jamais acquis ou de rester vigilant, votre vie durant. Parce que nous avons en effet désormais la preuve que plus aucune démocratie. Même la plus grande d'entre toutes. N'est à l'abri. Parce qu'il nous faudra toujours rester vigilant, les auteurs de la présente proposition de loi, la sénatrice Mélanie Vogel en tête, propose d'inscrire notamment le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans notre Constitution, je veux ici les remercier chaleureusement pour leur initiative le 13 juillet dernier. En accord avec la première ministre. J'avais solennellement déclaré devant cette assemblée qu'en tant que garde des sous. Je soutiendrai avec force pour les voir aboutir. Toutes les initiatives parlementaires qui viserait à constitutionnaliser le droit à l'IVG, voici donc au rendez-vous accompagner. De ma collègue. Isabelle Rome. Alors j'entends déjà s'élever et j'ai entendu s'élever. Des voix pour dire que le droit à l'IVG est déjà suffisamment protégé en France et que l'exemple américain n'est pas transposable dans notre pays. Qui aurait pu songer que le wokisme serait transposée dans notre pays. On pourrait multiplier les exemples, la liste est évidemment très longue. Oui, mesdames et messieurs les sénateurs, nul ne peut nier que nos institutions fonctionnent différemment. Oui, c'est vrai, le conseil constitutionnel français n'est pas la Cour suprême américaine oui, bien sûr, les juges constitutionnels français passés et actuels ont une conscience accrue de leur rôle et juge régulièrement qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur, c'est là l'usage républicain et l'esprit de nos institutions, oui, il est vrai, encore que le droit à l'IVG a été confortée au fil des ans depuis qu'il a été consacrée pour la première fois dans notre droit par la loi Veil du 17 janvier 1975 je pense ici à la dernière loi en date du 2 mars 2022 qui a allongé le délai légal pour recourir à l'IVG et le porte désormais de 12 à 14 semaines, je pense aussi aux lois qui ont précédé, comme par exemple la loi du 4 août 2014. Pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, loi qui a supprimé le critère de la situation de détresse. Pour autant. Je persiste et je signe : accompagner les initiatives parlementaires pour graver dans le marbre de notre Constitution le droit fondamental à l'IVG, me paraît aujourd'hui pertinent en ces temps troublés où des projets politiques n'ont certes pas cours dans cet hémicycle, ou si peu. Projet qui grandissent et rendent possible des recul drastique pour le droit des femmes d'abord, disons-le, cette inscription aurait la force du symbole. Force du symbole qui n'est pas anodine lorsque l'on parle de la loi suprême de notre pays, car oui, la Constitution et les textes fondateurs de notre État de droit, le socle commun des valeurs de notre République et des libertés fondamentales de notre société. Dès lors, quel beau symbole pour la France, pays des droits de l'homme que celui d'élever au plus haut rang de la hiérarchie de ces normes, le droit de la femme à disposer, monsieur le sénateur, de son propre corps. En ces temps de division. De perte de repères, quel plus beau message envoyé à plus de la moitié de la population française pour lui dire que la Constitution lui garantit lui garantit le droit à disposer de son corps et donc le droit à l'émancipation car oui, au-delà du symbole, il y aurait des conséquences concrètes, alors que le Conseil constitutionnel a rattaché l'IVG ah je cite la liberté de la femme qui découle de l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, inscrire l'IVG dans la Constitution permettrait de le consacrer enfin comme un droit fondamental et non simplement comme une liberté autonomie comme disent les juristes constitutionnelle mais il y a une autre raison. Plus pragmatique sur laquelle je veux insister un instant en tant que garde des Sceaux, cette raison elle est évidente : changer la Constitution est beaucoup plus difficile le changer la loi aujourd'hui consacré par la loi, si le droit à l'IVG était demain protéger au niveau constitutionnel, il ne pourrait être remis en cause que par le pouvoir constituant. Car cela nécessiterait à tout le moins, que les 2 chambres et vous connaissez bien sûr la règle soit d'accord pour y consentir premières difficultés et pas des moindres, puis dans un second temps, que le Parlement réuni en Congrès ou que nos concitoyens par référendum valide ce qui serait une régression terrible pour la condition des femmes, je veux m'appesantir un instant. Pour vous dire le fond de ma pensée. Du fond de mes tripes et pardonnez-moi cette familiarité. Je veux montrer comment la course, des choses comme disait Alain justifie que nous soutenions l'inscription de l'IVG dans notre Constitution. Alors que Simone Veil s'exprimait le 26 novembre 1974 devant l'Assemblée nationale pour porter cette grande loi elle inscrivait son projet sous le signe de l'espérance, permettez-moi humblement de reprendre ici ces mots alors qu'elle concluait son discours pour convaincre les députés encore hésitants. Mesdames, messieurs les députés, je ne suis pas de ceux. Et de celles-ci redoutent l'avenir c'est simple. Simone Veil croyez profondément que la loi qu'elle portait alors permettrait à la société française de progresser et l'avenir lui a bien heureusement donné raison mais. Mais, mesdames et messieurs les sénateurs, j'aimerais tant vous dire à cette tribune, hein, 19 octobre 2022 presque 50 ans après la légalisation de l'avortement que non, moi non plus je ne redoute pas l'avenir, j'aimerais tant aujourd'hui ne pas être de ceux qui tremblent face à l'avenir et aux incertitudes qu'ils charrient parfois j'aimerais tant être de ceux qui tranquille et d'un pas assuré avance insouciants sur le chemin de la vie. Croyant, ce qui est acquis. Et que ce qui est acquis est acquis. Et que ce qui est là, le sera pour toujours, j'aimerais tente enfin. être de ceux qui, d'un revers de main balayant les exemples étrangers et en particulier l'exemple américain, où le droit recule et avec lui souvent la condition des femmes qui peut aujourd'hui dire. Ce qui s'est produit aux États-Unis. Ne pourrait pas se produire en France, soyons clairs, qu'est ce qui a amené la décision de la Cour suprême américaine l'élection d'un président populiste. Légitimement élu certes disposant d'une majorité au Sénat américain, qui a pu nommer au cours de son mandat, 4 juges de la Cour suprême. Pardon. Je ne pense pas que les membres du Conseil constitutionnel soit nommé exclusivement par un président de la République futile populistes, pardon, il y aurait là de quoi déstabiliser une véritable institution, je ne pense pas que nos textes le permettent, le constat il est simple, il est simple, politiquement et juridiquement un président ou une présidente. Disposant presque naturellement d'une majorité pourrait, je dis bien pourrait. Revêtir en latin actuel du droit sur cette avancée historique et démocratique que représente le droit à l'interruption volontaire de grossesse, c'est d'ailleurs le cas chez certains de nos voisins européens, c'est donc pour des raisons totalement opposées à celles. De l'illustrent : Simone Veil. Parce que précisément je redoute l'avenir que je suis aujourd'hui favorable à ce qu'on élève sa grande loi, celle de 1975 tels qu'aujourd'hui modifier sa grande conquête : celle de toutes les Françaises au sommet de la hiérarchie des normes oui mesdames et messieurs les sénateurs, je veux mettre le droit à l'IVG dans notre constitution, là précisément où il ne sera pas possible de l'en retirer sans l'accord du Sénat. Car je sais que là encore. Il sera comme toujours le garant de nos droits les plus fondamentaux, je le dis sans aucune flagornerie inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, c'est aussi s'assurer que le Sénat dans sa grande sagesse, soient assurés d'avoir le dernier mot, si d'aventure. Un président. Une présidente. Et sa majorité l'abroger je crois avec force au rôle presque informel mais pourtant bien réelle et durable du Sénat en tant que garant de notre bien commun de notre conscience collective. On dit souvent que le président Mitterrand a été particulièrement courageux d'abolir en 1981 la peine de mort, alors que le compatriote y était majoritairement opposés mais ce que l'on ne dit jamais, c'est que le Sénat a lui aussi tout aussi courageusement adopté conforme 12 jours à peine après l'Assemblée nationale, la loi que portait alors, Robert Badinter, mesdames et messieurs les sénateurs, ne vous trompez pas inscrire aujourd'hui le droit à l'IVG dans notre Constitution n'est pas une mesure gadget. Un artifice de communication ou un mouvement de panique face à un exemple étranger lointain inscrire le droit à l'IVG, cette liberté fondamentale et inaliénable de la femme, c'est une sécurité pour toutes les femmes de ce pays. Mesdames et messieurs les sénateurs, faites en sorte que personne ne puisse abolir demain ce droit sans que vous soyez consultez. Les temps troublés et les remous ne sont jamais loin dans le frêle et ce qui fait de la démocratie qui mérite toute notre attention en tant qu'ancien avocat mais aussi en tant que citoyen, j'ai toujours essayé de faire en sorte. Que jamais l'on oublie que notre démocratie, notre état de droit, les libertés fondamentales qu'ils consacrent. Ce sont des biens précieux nos joyau commun pour lesquels il est indispensable de se battre sans relâche en tant que garde des Sceaux, il est désormais de mon devoir de les préserver, c'est pourquoi je dis aux sénatrices et sénateurs, que vous êtes, ne prenons pas de risques et protégeons autant que notre droit le permet cette liberté fondamentale des femmes qui est le droit à l'IVG, que les choses soient claires : ne s'agit pas d'une entreprise aisée, je le dis avec gravité : on ne doit toucher à la Constitution, selon la formule consacrée, que d'une main tremblante, c'est pourquoi il nous faut avoir à l'esprit que le détail de la rédaction qui serait in fine et retenu sera déterminant, tout comme le périmètre exact de la réforme, une rédaction inadapté, pourrait en effet conduire à consacrer un accès sans condition à l'IVG. Je pense par exemple à des IVG, bien au-delà de la limite légale en vigueur, ce qui n'est pas souhaitable, nous en convenons une écriture mal soupeser pourrait également s'avérer trop rigide et empêcher une adaptation possible possible du dispositif actuel, si celle-ci s'avérait nécessaire, comme cela a d'ailleurs été le cas en mars dernier, il nous faudra au cours des débats ici et à l'Assemblée, rester très vigilant sur les possibles effets il nous faudra également rester vigilants sur le choix de la place à laquelle inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution afin de donner tout son sens à cette reconnaissance toute sa cohérence au regard naturellement des autres dispositions constitutionnelles, mais ma crainte première. Et elle semble fondée. C'est qu'il n'y ait justement pas ce débat. Car j'ai pris acte du rejet du texte par votre commission des lois. Mais chez moi vous dire. Avec la liberté qui est la mienne. Que je le regrette. Pas tant pour le détail de l'écriture de la proposition de loi de la sénatrice Vogel sur laquelle je rejoins d'ailleurs un certain nombre de crainte de la rapporteure Agnès Canayer, je le regrette car cette décision souveraine de votre commission acte au fond un refus de principe de constitutionnaliser le droit à l'IVG. Il n'est même pas question pour la commission de travailler sur une meilleure rédaction possible, non, il s'agit d'un refus pur et simple qui condamne par anticipation toute initiative d'où qu'elle Vienne, or vous le savez sans doute, sans l'aval du Sénat le verrou crée de notre constitution ne peut être levé. Il faut pourtant que le débat vive j'espère donc que l'hémicycle dira non, nous ne fermons pas la porte d'emblée essayons d'avancer ensemble sur cette proposition ou celle de la présidente berger ou essayons d'entendre les pour, mais aussi bien sûr les contres, essayons d'entendre les craintes pour les apaiser et surtout travaillons ensemble pour trouver la meilleure rédaction possible et de ne pas manquer cette occasion alors que les planètes s'alignent aujourd'hui pour permettre enfin cette constitutionnalisation. Je le dis et je le regrette, si le Sénat est prête à avancer avec prudence et sans idéologie sur cette question, le gouvernement répondra présent, de fait, il répond déjà présents aujourd'hui devant vous, car oui, le gouvernement vous l'avez compris, est favorable à la constitutionnalisation du droit à l'IVG, je le dis également le gouvernement répondra présent pour soutenir chacune des initiatives parlementaires qui sont nombreuses en la matière. Les rédactions proposées sont diverses et je suis persuadé que ces initiatives, je pense à celle de la présidente Aurore Bergé à sa collègue Marie-Pierre Rixain qui portent toutes les deux avec force et Constance ce combat nous permettront d'atteindre, je le crois, la meilleure rédaction possible avant de conclure mon propos, je veux dire ici à ceux qui nous regardent, il ne s'agit pas de livrer telle ou telle parlementaire à la vindicte des réseaux sociaux comme cela a pu être fait. Je pense. Ah, la présidente, bilan. Lors de la présentation de sa proposition de loi, j'ai éprouvé personnellement depuis 2 ans. Et sur de très nombreux textes. Votre engagement sans faille, madame la sénatrice Canayer pour la défense de notre état de droit et des droits de nos concitoyens, le débat politique, il les fait bien sûr de désaccord. Et tout le monde a dans cet hémicycle le droit d'exprimer librement ses opinions sans crainte d'être inquiété le débat politique, il est aussi fait d'accord et de convergence patiemment construit sur le chemin du compromis avançons ensemble sur ce chemin du compromis, mesdames et messieurs les sénateurs, comme nous l'avons fait. Tant de fois. Sans démagogie, sans idéologie pour renforcer à nouveau les droits de l'homme, qui sont cet après-midi, ceux de la femme. La parole est à Madame Isabelle Rome ministre. Le déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes de la diversité et de l'égalité des chances. Madame la présidente. Monsieur le garde cher Éric mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, merci monsieur le garde des Sceaux pour votre discours puissant, merci pour vos mots. C'est la première proposition de loi qu'il me revient de soutenir aujourd'hui devant vous, comme ministre délégué auprès de la Première ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, je suis fier qu'il s'agisse de celle consistant à inscrire le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans notre constitution d'entourer ce droit conquis de haute lutte après des années de combats féministes et grâce à l'opiniâtreté et la force de Simone Veil, de l'entourée d'un rempart car il faut le préserver le protéger. Contre les menaces de vent mauvais où les courants réactionnaires ce rempart doit être à la hauteur de ce qui fonde notre République une libre égal fraternel. C'est pourquoi il est nécessaire d'inscrire le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution du 4 octobre 1958 vous l'avez rappelé monsieur le garde des Sceaux, il est beaucoup plus difficile de changer une Constitution que de changer la loi, qu'une autre loi, une autre majorité peut défaire en quelques mois parce que non, madame la rapporteure, malgré le respect que je peux avoir pour vos travaux, nous ne sommes à l'abri de rien quel américaine aurait imaginé il y a 2 ou 3 ans encore voir s'effondrer la protection de ce droit soumis désormais aux aléas politiques des différents États membres des États-Unis. Aurait-on penser il y a moins de 2 ans au sein même de l'Union européenne que des États reviennent sur le droit à l'IVG en autorisant les femmes à avorter seulement en cas de viol ou de grave danger ou en les contraignant à écouter le coeur du foetus avant de prendre leur décision, depuis 2017, le gouvernement et la majorité non, au contraire, c'est de renforcer la législation en matière de droits sexuels et reproductifs en donnant un accès gratuit à la contraception pour toutes les femmes jusqu'à 25 ans en allongeant les délais d'accès à l'IVG de 12 à 14 semaines de grossesse en prévoyant le tiers payant intégral de l'IVG, afin notamment d'en assurer la confidentialité et en soutenant résolument le planning familial dont les financements seront augmentés pour pour le lancement de leur Chat visant à lutter contre la désinformation. Ce combat avec François Braun, ministre de la Santé nous le poursuivons en rendant dès l'an prochain, la pilule du lendemain gratuite sans ordonnance pour toutes les femmes, ce combat avec Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, nous le menons cet après-midi avec la représentation nationale et je remercie madame la sénatrice Bella 10 Vogel de nous en donner l'occasion à travers cette proposition de loi constitutionnelle une proposition que porte également la majorité parlementaire, emmenée par Aurore Bergé. Je remercie par ailleurs, l'ensemble des parlementaires engagés et particulièrement les membres de la des délégations à l'égalité femmes-hommes du Sénat conduite par Annick Billon avec laquelle j'ai change de manière très régulière et très. Ce combat, la France le mène également hors de ses frontières, c'est dans ceci on que le président de la République, a affirmé le 19 janvier dernier devant les eurodéputés, vouloir inscrire le droit à l'IVG dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et c'est dans ce sillon que s'inscrit notre diplomatie féministe dans le Forum génération égalité organisé à Paris en juillet 2021 a constitué le point culminant, la contribution de la France pour les droits sexuels et reproductifs à l'échelle internationale se hisse à hauteur de 400 millions d'euros sur 5 ans. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, les droits sexuels et reproductifs conditionne tous les autres droits des femmes détricoter écorné ou n'ayez chez droits constituent assurément une forme de violence fondée sur le genre. Parce que les droits des femmes sont des droits humains, ils ne sont ni chez Cable ni hiérarchie ce ne sont pas des droits à moitié mais des droits fondamentaux, inaliénables qu'il convient de protéger et de consolider. Aucune femme aucune de nos filles ne doit vivre en France, dans la peur d'être un jour dénoncer. Arrêtée, jugée pour avoir avorté, comme ce fut le cas de Marie-Claire en 1973 jugé au tribunal de Bobigny est remarquablement défendue par Gisèle Halimi, cette garantie notre République doit leur apporter, c'est pour toutes ces raisons que comme l'a déjà exprimé la première ministre, le gouvernement est favorable à la constitutionnalisation de l'IVG. Et n'en déplaise à l'extrême droite qui malgré le vernis qu'elle tente de nous montrer n'a jamais été et ne sera jamais l'allié des droits des femmes, nous devons être collectivement lucide. La menace d'un retour en arrière n'est pas une chimère. L'exemple américain, le pays d'Elizabeth qui distingue tonnes est un avertissement. S'attaquer à l'avortement, c'est s'attaquer à toutes les femmes et c'est s'attaquer à la liberté. Le gouvernement sera toujours du côté des femmes et de la liberté, je vous remercie. Merci quand nous. Dans la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable. Stéphane Ravier a déposé une motion distribuée sous le numéro 1 tendant à opposer la question préalable au texte en discussion, la parole est donc à monsieur Stéphane Ravier pour la motion et pour trois minutes. Madame la présidente, monsieur le Ministre, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'immigration jusqu'au remplacement l'islamisme se jusque dans nos écoles, l'insécurité, jusqu'à la barbarie, la fiscalité jusqu'au raquette la précarité jusqu'à la pauvreté de masse, les sujets graves j'ai sujets graves ne manquent pas en France mais nous voilà en train de perdre un temps précieux en discutant d'une problématique importée des États-Unis, sans aucun rapport avec la réalité de notre pays et c'est pourtant ce dont les auteurs de ce texte se réclame dans l'exposé des motifs, vous êtes hors sujet, je dirais même qu'il n'y a pas de sujet, c'est pourquoi je vous propose mes chers collègues d'enterrer ce texte avant même son examen un texte. Dangereux, inutile, qui permet à ses auteurs, de faire de l'agit-prop comme l'a lui-même analysé et dénoncé dans Le Figaro du jour, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, Jean Éric Chatel, vous avez voté le prolongement de l'avortement jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée dans un texte de loi du mois de mars, ces attaques envers la vie ne vous suffisent-t-elle pas, c'est complètement anachronique de dire que l'avortement est menacée dans notre pays quand il existe un délit d'entrave de 2 ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende pour quiconque tenterait d'y opposer un avis contraire, ce sont encore 223000 avortements qui ont été réalisés, aggravant l'hiver démographique français, cela ne vous suffit toujours pas, il y a des impératifs de santé dans notre pays, dans ce texte nous détourne l'avortement invoqué dans le cas pour les cas d'urgence dans la loi Veil est devenu un avortement encourager en 2022 pourtant, il faut le rappeler, ce n'est pas un acte anodin, moi je suis plutôt inquiet tournure que prennent les propositions actuelles, je vous rappelle cet amendement sur l'avortement à neuf mois 9 mois en invoquant une détresse psychosociale vous considérez que cet infanticide légalisée est un progrès, je considère que c'est une ignominie qui vous déshonore souvent les femmes avortent sous la contrainte psychologique ou économique accompagnant les soutenons-les, elle est là la mission du politique, il est là notre devoir de plus sur le plan juridique, ce texte vient encombrer la constitution dans un, dans son article 8 pourtant consacré au pouvoir judiciaire, la Constitution régit l'organisation des pouvoirs publics, elle n'est pas une charte de droits, j'ai entendu que les auteurs de la loi souhaitée constitutionnaliser un droit pour empêcher les lois régressives je trouve pourtant que l'objectif régressif et tout à fait celui qui correspond aux infâmes lois bioéthiques que nous avons voté que vous, vous avez voté ces dernières années et quelque chose me dit que le pire est encore devant nous, cette proposition de loi cosignée par 5 présidents de groupes écologistes, socialistes, communistes, Renaissance et radicaux nous donne à voir un front commun, c'est une clarification de position pour une plus grande clarification. Merci, cher collègue, je vous propose la parole est à Madame, Mélanie Vogel contre la motion, merci, je crois que vous pouvez le dire toujours, ça dépend, je suis toujours. C'est pas grave. Madame Vogel, vous avez la parole Je vais vous dire une chose Monsieur Ravier, j'aurais presque envie de vous remercier, évidemment je ne vais pas le faire, mais vous êtes exactement en train de démontrer pourquoi nous sommes en train de faire ce que nous faisons, comme l'a dit. Comme le dit si souvent et si souvent si bien Laurence Rossignol, il n'y a pas d'exception française, eut égard à l'extrême droite, l'extrême droite française, elle est comme l'extrême droite partout, elle s'oppose aux droits des femmes, elles s'opposent aux droits sexuels et reproductifs elle déteste tous les acquis de la République tous les progrès que les féministes sont acquis de haute lutte, elle déteste l'égalité des droits à la liberté et n'ayez aucun doute cher collègue, sa détermination à les détruire si par le pire des malheurs de l'histoire et l'arrivée au pouvoir en France et Total évidente et parfaitement transparente, on nous raconte que le droit à l'IVG n'est pas menacée en France, qu'aucun parti politique en France ne peut revenir sur le droit à l'avortement, hé bien voilà la force politique qui a fait 42 % des voix au second tour d'élection présidentielle vient de vous prouver le contraire, alors oui c'est vrai il y a une clarification, il y a ce dans cet hémicycle, celles et ceux qui sont en faveur des droits et des libertés fondamentales, y compris les droits et libertés fondamentales des femmes et celles et ceux qui ne le sont pas, alors, chers collègues, la question, de quel côté êtes-vous, je vous le demande, encore une fois surtout à celles et ceux qui, dans cet hémicycle tient encore à tenir l'extrême droite et son projet à distance, prenez la mesure du moment historique que nous vivons les fascismes progresse et avec eux les attaques de nos droits les plus fondamentaux, personne ne sait qui gouvernera la France en 2027, quelle sera la prochaine majorité à l'Assemblée nationale, personne, nous sommes ici une majorité je crois dans cette assemblée, a rappelé notre attachement au droit à l'IVG, hé bien, prouvant le. Merci, quel est l'avis de la commission, même le rapport. Merci madame la présidente, alors la commission des lois n'a pas pu se réunir, mais j'émets un avis évidemment défavorable à cette question préalable, il est nécessaire, même si nous avons des oppositions justement que le débat démocratique se fasse ici au Sénat, de manière calme et serein et c'est ici la force du Sénat de pouvoir débattre en respectant les convictions des uns et des autres. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs. Nous pensions avoir exposé tous les arguments qui n'qui nous était venu en tête, nous avons partagé d'ailleurs un certain nombre de de ses arguments, évidemment, et puis voilà que, Monsieur le Sénateur Ravier nous chamboule. Voyez. Au fond, monsieur le sénateur, l'imaginaire, voyez-vous, et souvent le dernier refuge de la liberté. Et alors, vous nous donnez une formidable raison. De voter ce texte.

moi je pense que l'avortement est sérieusement menacée dans ce pays, vous voyez. Ah oui. Bon, et puis je vais vous dire une chose là quand on parle de droits de l'homme et surtout le droit de la femme, on n'est jamais hors sujet, monsieur le sénateur, voilà

un peu plus à droite encore mauvais, il était, il a été élu sous l'étiquette de Marine Le Pen, il est parti plus à droite encore, bon, nous verrons tout ça, ça c'est de la petite politique politicienne. Mais merci, merci de nous avoir apporté ce témoignage moi, monsieur le sénateur, les mots que vous avez utilisé à la tribune, je n'aurais jamais osé les prononcer, merci d'être là, vraiment, merci. monsieur le garde des Sceaux. Je vais passer aux explications. De de vote, je voudrais vous rappeler que, s'agissant d'une proposition de loi constitutionnelle il y aura un scrutin public et je passe la parole à Monsieur Iacobelli.

aux atteintes aux droits des femmes qui traverse les différents pays et d'ailleurs pas seulement outre-Atlantique je pense sur le continent européen, je pense à l'Italie qui dernièrement avec Mélo ni souhaite développer des alternatives d'ailleurs vos amis et Monsieur Ravier. Vos amis qui sont aux responsabilités,

c'est. Ce qui équivaut à une interdiction de l'interruption volontaire de grossesse en Hongrie, un autre ami à vous Monsieur Ravier le mois dernier a durci la réglementation et que tout le monde le sache aujourd'hui, vous savez ce qu'est-ce qu'ils ont demandé, ils ont demandé aux femmes qui souhaitent avorter d'écouter le le coeur de leur fait, pour éviter d'avorter, voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui de votre famille politique à travers leurs propres et c'est ça la réalité des attaques contre le l'interruption volontaire de grossesse, alors moi, chers collègues, j'ai

cette grande loi de progrès, est ce que nous soutenons le droit des femmes à disposer de leur corps est ce que nous soutenons, en tant que Français, nous sommes attachés à ce que la France qui reste ce phare des droits dans un océan de pays qui attaquent effectivement les droits des femmes à travers le monde et est ce que nous souhaitons, et là je je pose la question aussi au gouvernement et ce que nous souhaitons que par cette constitutionnalisation, nous puissions pousser le gouvernement à faire en sorte que ce droit soit effectif dans l'ensemble des territoires et notamment dans la ruralité

Monsieur Kessler bah, mes chers collègues, sommes-nous sénat de la République. Encore capable aujourd'hui de discuter sereinement d'un sujet essentiel pour la vie de notre société. Sommes-nous capables de laisser un instant de côté les patients. Et de faire un travail utile pour notre pays, je le souhaite, je le garde des Sceaux. Vous avez invoqué Simone Veil. Bien que j'ai été l'un de ses plus proches collaborateurs, et que ce lui soit resté fidèle jusqu'au bout. Je ne parlerai pas en son nom, nul n'a le droit de le faire. Mais le vrai combat, c'est elle qui l'a mené le vrai courage, c'est elle qui l'a eu. Et il importe aujourd'hui encore de lui en rendre hommage car les équilibres qu'elle a su trouver sont ceux sur lesquels nous vivons 50 ans, un peu moins après et c'est très important de le dire ne déplaçons pas ces équilibres alors monsieur le garde des Sceaux. Je ne comprends pas exactement votre position, vous avez parlé de symbole de beau symbole d'accord pour les beaux symbole mais ici nous légiférons et quand tu nous légiférons sur la constitution, nous ne cherchons pas des symboles, nous cherchons à être utile à notre pays, or, à la fin de votre propos, vous n'avez pas manqué et vous ne pouviez pas faire autrement. De prendre des distances à l'égard du texte qui nous est proposé et de montrer que celui-ci devrait être améliorée sur bien des points parce qu'ne vous paraît pas

Merci madame la présidence, Madame la Ministre, Monsieur le garde des sceaux, chers collègues, le groupe de l'Union centriste ne votera pas cette motion tendant à opposer la question préalable parce que le débat a eu lieu sereinement commission. Madame Vogel a été invité à présenter sa proposition de loi. ça a été un vote de la commission des lois, qui l'a permis, mon cher collègue, la rapporteure, a fait un travail qui est un travail équilibré et le le débat a pu avoir lieu, le principe d'une discussion générale, c'est de permettre à tout un chacun d'exposer son son opinion et je trouve qu'à l'instant où on se parle le débat dérape donc j'aurais, pour le coup, compte de l'du groupe de l'Union centriste, l'occasion de rappeler la position majoritaire dans le respect de ceux qui voteront différemment, et donc je souhaite, au nom de mon groupe que ce débat puisse avoir lieu et que le calme revienne. Merci, cher collègue, alors je vais consulter le Sénat. Sur la motion tendant à opposer la question préalable, je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du texte en discussion en application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire et de droit, le scrutin sera ouvert dans quelques instants, le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter Le scrutin clos. Voici le résultat du scrutin numéro 7 sur la motion numéro compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs aux groupes politiques et notifié à la présidence, nombre de votants 345 Nombre de suffrages exprimés 345 pour l'adoption, hein, contre 344 le Sénat n'a pas s'adopté dans la suite de la discussion générale, je vais donner la parole à monsieur Stéphane Artano pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour quatre minutes chers collègues. Madame la présidente, mesdames, messieurs les Ministres Monsieur Président, la commission des lois, madame le rapporteur, mes chers collègues, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour les droits des femmes soient remis en question ces droits ne sont jamais acquis, vous devrez rester vigilant, votre vie durant oui vigilant, nous devons l'être, mes chers collègues, cet avertissement de Simone de Beauvoir est tristement prémonitoire et et d'actualité, on est fait, 50 ans après l'adoption de la loi Veil, force est de constater que le droit à l'avortement est loin d'être acquis entre interdiction totale et restrictions il faut savoir que les avortements clandestins provoquent en moyenne, la mort d'une femme toutes les 9 minutes dans le monde sont me livrer à un commentaire de la jurisprudence de la Cour suprême américaine je retiendrai que le droit à l'avortement et l'une des premières cibles des conservateurs excessif, alors j'entends, et d'une certaine façon, je comprends les arguments mis en avant par notre rapporteur, il n'y a rien de faux à dire que ce procédé n'empêcherait pas d'une part la possibilité d'une nouvelle révision constitutionnelle afin de faire céder la disposition protectrice notre part son inscription pourrait anticiper participer pardon à une inflation des droits constitutionnels assimilable à une heure, l'inflation législative, les reproches faits à la loi bavarde se reporteraient sur la Constitution et plus largement sur le bloc de constitutionnalité dont dont à à devenir trop large et perdant en efficacité à cela vous ajoutez que le Conseil constitutionnel des fonds déjà l'accès à l'IVG comme composante de la liberté de la femme à laquelle découle de l'article de la déclaration des droits de l'homme et du Citoyen de 1789 d'un point de vue du droit, tout cela se tient d'autant qu'en France, fort heureusement, de ceux qui voudraient remettre en cause l'IVG et la contraception sont extrêmement minoritaires, nous sommes donc face à un texte qui d'un point de vue juridique on peut justifier qu'il ne soit pas nécessaire d'un point de vue social non plus, pour autant, j'en suis signataire de cette proposition, portée par notre collègue Mélanie Vogel et je la voterai bien évidemment en 1er lieu parce qu'il faut y voir un moyen de défense des droits des femmes dans notre pays, en second lieu parce que c'est une façon de dire aussi que la France ne cédera pas à l'obscurantisme et au populisme montrons l'exemple d'autres cède au recul des idées pour la liberté et l'émancipation continuons affirmé que les droits à l'IVG à la contraception ne saurait être malmené à l'avenir, ils ne sont pas tributaires d'interprétation, il est trop précaire de se résoudre sur un tel sujet à la seule interprétation depuis 2002 par les juges d'un article datant de plus de 2 siècles par ailleurs à un revirement de jurisprudence et d'interprétation serait trop simple justifier, j'entends déjà ceux qui nous expliquerez qu'au sens strict ou historique, l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne se réfère ni à l'IVG, ni à la contraception, autrement dit ce qui est arrivé aux États-Unis pourrir arriver chez nous également, il faut donc aller au-delà, comme le propose cette proposition de loi la constitutionnalisation d'un droit est un processus efficace, vous l'avez rappelé monsieur le garde des Sceaux, afin de sanctuariser le dans le texte suprême un droit autonome et le protégé de toute volonté politique que ce soit celle du législateur ou des juges, bien sûr, dit qu'il y a un droit constitutionnel fondamental ne sera pas suffisant à faire qu'il le soit, nous devons poursuivre nos efforts mais ça été rappelé pour qu'il soit effectif, qu'il s'inscrive dans les moeurs, l'éducation des jeunes générations est essentiel de ce point de vue, il faut aussi empêcher toute restriction de personnel et de suppression de 100 pratiquant l'avortement lors de restructurations hospitalières et nous en sommes évidemment bien d'accord, vous l'aurez compris dans sa grande majorité, le groupe RDSE votera en faveur de cette proposition de loi. La parole est à Madame Muriel Jourda pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes chers collègues. Madame le président monsieur garde des sceaux, Madame le Ministre, Monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, mes chers collègues, à l'instar de la quasi-totalité des sénateurs du groupe, les républicains je ne voterais pas à ce texte, je ne voterai pas et j'ai peu de temps pour vous expliquer pourquoi je ne voterai pas et je risque d'être un peu brutal, je ne voterai tout simplement pas parce que c'est de la mauvaise législation. C'est la mode de gestion et nous sommes essentiellement des législateurs ici nous ne sommes pas des militants quand nous rentrons dans cet hémicycle, nous ne descendons pas des brevets de morale, nous ne faisons pas de la politique fiction, nous faisons la loi et ce serait à l'évidence de la mauvaise loi, ce serait la mauvaise loi, d'abord parce que c'est un texte de réactions réactions effectivement à une décision qui a été prise par la Cour suprême des États-Unis et qui vise à renvoyer aux États fédérés le soin de légiférer sur l'IVG. Le fait que pas moins de 6 propositions de loi, été déposée démontre bien que c'était en réaction à cet événement que ce texte nous est proposé aujourd'hui visant à constitutionnaliser la liberté des femmes de recourir à l'IVG, la réaction précède toujours la réflexion et elle nous fait envisager une situation par la fenêtre étroite et déformante de l'émotion plutôt que de l'envisager dans toute sa complexité, le 2ème défaut de cette législation et que vraisemblablement, sans vouloir, elle met à mal notre ordonnancement juridique, alors je ne suis pas une fétichiste du droit et je pense que le droit n'est qu'un outil, mais avons France nous avons une boîte à outils assez garni et si nous voulons qu'elle reste opérationnelle et il y a, il faut qu'elle soit toujours ranger, or la Constitution contient l'organisation des pouvoirs publics et aussi, affirme un certain nombre de droits fondamentaux, le Conseil constitutionnel nous indique quant à lui dans une jurisprudence constante que le droit des femmes, la liberté des femmes d'avoir recours à l'IVG et la déclinaison d'un de ses droits fondamentaux, mais si nous inscrivons dans la Constitution la déclinaison de tous les droits fondamentaux, au mieux, nous en serons espèce de code général au pire nous la rendrons lisible et nous en détruirons tous les effets, cela est à peu près intangible, mes chers collègues, et enfin, et je reprends là les mots de monsieur le garde des Sceaux, ce texte est fait pour être un symbole. La loi n'est pas un symbole, la Constitution elle n'est pas un symbole : nous sommes tous touchés ici par le cas des femmes américaines qui, suivant les États dans laquelle ils vivront ne pourront plus profiter de cette liberté d'avoir recours à l'IVG et nous l'entendons parfaitement, même si la France est le phare où a été le phare des libertés individuelles et de l'universalisme, nous ne pouvons pas nous servir de notre constitution, comme d'un message à envoyer aux femmes du monde entier. Un texte de loi est faite pour produire de l'effet pas pour être symbolique, alors il ne m'échappe pas que l'effet escompté de ce texte et de protéger sa liberté des femmes de recourir à l'IVG. Mais là encore, mes chers collègues, la Constitution n'est pas un coffre-fort ou alors le législateur, on a le code depuis fort longtemps, puisque depuis 1958 nous n'avons pas modifier la Constitution, moins de 24 fois et ça été fait, n'est guère protecteur, mais d'autres ont le temps de le développer après moi et puis, surtout, les protégés de quoi. Quel danger menace aujourd'hui la liberté des femmes. Quel danger menace : nous avons eu récemment des élections nationales, quel parti politique a développé dans son programme l'abrogation de l'interruption volontaire de grossesse, aucun, aucun, car cela n'est pas à l'ordre du jour, personne en France n'est opposé à l'IVG, ça ne veut pas dire que personne ne le soit à titre personnel mais chacun garde sa dans son for intérieur, aujourd'hui, et c'est précisément tout le danger de ce texte car vous savez que pour aboutir cette procédure doit nous conduire au référendum, proposé par le président de la République, chacun sait que les résultats des référendums éclaire moins sur l'état de l'opinion sur la question posée que sur la popularité de celui qui pose la question, tout cela est très hasardeux, me semble-t-il et surtout lorsque nous avons référendum, nous avons un débat et lors de ce débat, ce qui gardaient leur opposition à l'interruption volontaire de grossesse dans leur for intérieur, hé bien nous serons amenés tout à fait légitimement à le déposer sur la place publique et nous, on est arrivé à Aix ce avec ce texte nous allons arriver à la situation dans laquelle, pour protéger la liberté des femmes d'une menace qui était inexistante en France et nous légiférons pour le sol français et pour le droit français, nous allons remettre en débat une liberté qui semblait pour les femmes qui, depuis des décennies, alors mes chers collègues, si véritablement vous voulez protéger les femmes ne votaient pas ce texte. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues avant janvier 75 c'était hier. L'avortement était un délit pénal sanctionné jusqu'à 5 ans de prison les médecins pouvaient être condamné à une interdiction, interdiction d'exercer. Et les femmes concernées, elles étaient contraintes d'aller à l'étranger ou de recourir à des avortements clandestins. La reconnaissance de l'interruption volontaire de grossesse a été le fruit d'un long combat, on se souvient du Manifeste des 343. On se souvient de l'acquittement de la jeune Marie-Claire, on se souvient, moins de la première tentative très encadré de légalisation qui a échoué en 1973 et porté par Michel Poniatowski, à l'époque, ce sujet a profondément divisé la société les débats au Parlement, se sont déroulées dans une rare violence, Simone Veil, soutenu par Jacques Chirac, par une partie de la majorité et par l'opposition, défendra son texte avec acharnement, malgré les attaques personnelles, son combat, c'était celui de toutes les femmes. Lors de son discours devant l'Assemblée nationale, elle déclara aucune femme ne recourt de gaieté de coeur à l'avortement, cette phrase. C'est évidemment toujours une réalité car même s'il s'agit d'une décision réfléchie. Peser et assumer un avortement demeure et demeurera toujours un événement marquant un drame dans la vie d'une femme. Suppression de la notion de détresse, allongement des délais d'avortement remboursement à 100 % par la Sécu, depuis la loi s'est adapté a été amélioré. Nous pouvons ici tous ensemble en convenir, la France n'est pas aujourd'hui, je vais le je veux dire à l'heure à laquelle on parle menacés de connaître un retour en arrière sur ce sujet. D'ailleurs, aucune parole crédible ou comme telles, ou en tout cas qu'il y a une certaine audience ne le réclament, ou ne le revendique. Bien qu'attachés à la protection fondamentale de l'interruption volontaire de grossesse, certains des collègues de mon groupe ne voit pas la justification juridique de cette démarche. Il considère qu'il s'agit d'un texte déclaratif qui n'aura pas d'issue positive un symbole qui ne fera pas avancer concrètement l'accès à l'IVG à l'avortement et quand enfin toucher à la constitution sur des questions sociétales revient à ouvrir une boîte de Pandore, c'est la raison pour laquelle certains élus de notre groupe, ça s'abstiendront ou voteront contre cette proposition. Sur le sujet, d'IVG nous sommes forcé de constater que toutes les autres démocraties n'avancent pas au même rythme que la France au sein même de l'Union européenne en Pologne : une loi vient de restreindre l'avortement qui n'est plus autorisé qu'en cas de viol ou d'inceste, de l'autre côté de l'Atlantique, la Cour suprême a remis en cause l'avortement, chaque État est désormais libre d'interdire l'avortement une dizaine d'ailleurs ont déjà commencé à faire marche arrière à nos frontières en Italie Madame Meloni, qui vient de remporter les élections assume de favoriser le droit à ne pas recourir à l'IVG, preuve que le combat de la liberté d'avorter n'est pas acquise, là on ne vend ont pensé qu'il était intouchable, madame la sénatrice. Il y a certaines des convictions, vous portez que je ne partage pas votre conception de la société n'est pas vraiment la mienne le propos que vous avez tenus tout à l'heure, est un peu agressif et un peu culpabilisant et je ne suis pas certain que ce soit la meilleure manière de défendre la cause que vous portez néanmoins comme d'autres collègues du groupe, je voterai en faveur de propositions car ce qu'une loi fait, une autre peut la défaire ce sera beaucoup plus difficile quand elle sera inscrite et gravé dans le marbre de la Constitution. Pour en terminer, je fais remarquer que ça demande pas de saveur de voir celles et ceux qui remettent en cause nos institutions qui parle souvent de la VIe République, finalement, s'appuyer sur la Constitution voulue par le général de Gaulle pour protéger un droit fondamental, essentiel des femmes de ce pays, je voulais souligner cette avancée ainsi comme je l'ai exprimé dans mon propos, fidèle à l'ADN du groupe, les indépendants, chacun votera selon ses convictions, merci. Merci, cher collègue, la parole est au président Guillaume. Tant pour le groupe écologiste solidarité et territoires pour 4 minutes. Merci madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre madame la rapporteure, mes chers collègues. Qu'est-ce qu'une constitution. Les étudiants en première année de droit et de sciences politiques dès leur 1er cours de droit constitutionnel, sont soumis à cette épineuse question et la réponse tient en 3 points. Premièrement, un traité d'organisation des pouvoirs publics garantissant leur séparation. Deuxièmement, un système de subordination des normes et troisièmement, un corpus de droits et de valeurs, la constitution et notre norme suprême chacun sait ici la force juridique comme symbolique du texte constitutionnel comme des principes à valeur constitutionnelle, quand j'entends sur nos bancs qu'inscrire le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution ne servirait pas ou peu. Je suis saisi par la surprise encore plus après les propos abjects du sénateur Ravier alors non la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne protège pas positivement le droit à l'IVG, hé oui, son inscription dans le marbre constitutionnel beaucoup plus dur à tailler que le calcaire de la loi est une protection considérable accordée aux femmes. Dont rêvent beaucoup à travers le monde et que l'on pleure de l'autre côté de l'Atlantique, c'est un truisme, qu'il faut étrangement répété et vous avez raison, Monsieur le Ministre, de le faire, il est bien plus complexe, de modifier le texte constitutionnel que la loi, a fortiori dans notre 5ème République rationaliser où l'exécutif tient le Parlement dans sa main de l'autre côté des Alpes, malgré sa victoire d'une ampleur inédite, la coalition des fascistes de la droite n'est pas en mesure de changer la Constitution et c'est un soulagement. Comme l'a rappelé le monsieur le garde des Sceaux, ne prenons pas de risques le funeste destin politique de nos voisins transalpins nous rappelle d'ailleurs que si l'IVG n'est pas aujourd'hui menacée dans notre pays, il faut profiter de ce moment pour le protéger, avant qu'il ne soit trop tard, pareille occasion ne se représentera pas de sitôt, alors comment inscrire le droit à l'IVG dans le corpus de droits et de valeurs qui est notre constitution, ce débat est légitime et il est vrai que dans la tradition constitutionnelle française, ses droits et valeurs sont plutôt énumérés dans les textes historiques qui font la grandeur de notre pays, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le magnifique préambule de la Constitution de 1946 textes rattaché au préambule de la Constitution de 1958 mais ce n'est pas une exclusive et on retrouve tout au long de ces articles de la Constitution, nombre de valeurs cardinales et de droits fondamentaux de notre République, parmi lesquels l'égalité, la laïcité, la souveraineté nationale, l'abolition de la peine de mort. Alors que faire écrire une nouvelle charte des droits des femmes, pour compléter la trop masculine : déclaration des droits de l'homme et du citoyen, renforcer l'article 1 qui assure déjà la parité politique créé un article 66 de pour interdire l'entrave à l'IVG, ce débat est fécond et légitime, mais ce n'est pas le débat du jour, nous ne souhaitons pas aujourd'hui sur la base de ce texte engagé un processus de révision constitutionnelle d'origine parlementaire qui déboucherait sur un référent référendum nous souhaitons aujourd'hui envoyer un message politique au gouvernement pour le rassurer, pour lui signifier qu'il trouvera ici au Sénat une majorité pour faire adopter un projet de loi inscrivant le droit fondamental à l'IVG dans notre Constitution, libre à lui, libre à vous, monsieur le garde des Sceaux de choisir la la la rédaction qui vous conviendra le mieux de convoquer une commission spéciale d'éminents juristes ou même une Convention citoyenne pour écrire une charte du droit des femmes,

Pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants pour quatre. 3 minutes et merci de respecter votre temps, je le rappelle. Madame la présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues. Dans ce mandat il y a des prises de parole qui sont plus importantes que d'autres, il y a des textes que l'on aborde avec le sentiment que nos mots compte davantage cette proposition de loi constitutionnelle en fait partie, si le groupe RDPI dans sa majorité, co-signe ont co-signé ce texte et s'il est unanimement attachée au droit des femmes à l'IVG et à son plein accès, c'est en tant que co-signataire je ferais une petite fenêtre avant pour vous dire que je viens d'un territoire où le taux d'avortements est 3 fois supérieure en moyenne à la France, et si le taux le plus élevé de France et où l'on ose à peine imaginer ce qu'un recul de ce droit pourrait provoquer, je vous laisse imaginer la proposition de loi constitutionnelle que nous examinons cet après-midi, vise à protéger à garantir ce droit fondamental en l'inscrivant dans la Constitution nous l'abordons allô cas que l'issue de nos débats ne fait guère de doute, ben je je souhaite me tromper. Mais puisqu'il s'agit de prendre rendez vous, j'aimerais revenir sur les arguments qui ont été avancés par la commission des lois pour justifier le rejet du texte, le premier argument d'ordre politique consiste à dire que le droit à l'IVG n'est pas menacée en France, il ne l'est pas, en effet, si l'on considère les professions de foi des principaux partis politiques ou même l'attachement des Françaises et des Français à ses doigts et cela, mes chers collègues, nous vous rejoignons la vraie question, cependant, c'est de savoir si le droit à l'IVG sera menacé demain cette menace existe aujourd'hui, on l'a vu aux États-Unis et plus près de nous, en Pologne, en Hongrie, et même en Italie, cette menace, nous la retrouvons dans les propos actuels actuels ou passés, des responsables politiques qui s'ils ne s'opposent pas frontalement à l'IVG ou à la contraception cherche insidieusement insidieusement c'est ce constat que nous sommes nombreux à partager sur ces bancs et dans notre pays, qui nous amène à contester le 2ème argument soulevé par la commission la semaine dernière, elle a estimé qu'une modification de la Constitution ne s'imposait pas, qu'il s'agissait d'une mesure purement pour pas m'asseoir et symbolique qu'il ne prenait pas, je cite, d'apporter une réponse aux difficultés d'accès à l'IVG soit mais l'enjeu n'est pas ici de renforcer un doigt ou même de le rendre plus effectif, il s'agit d'empêcher un retour en arrière : en cas de changement de majorité politique, il s'agit peut-être de politique-fiction mais l'actualité nous montre chaque jour que la fiction peut devenir soudainement réalité il s'agit ici de rehausser le niveau de protection de droit qui fait désormais pleinement partie de notre contrat social qui est justement consacré par la Constitution et de rendre plus difficile une régression que la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne saurait interdire aucune loi fondamentale le protège aujourd'hui dans le monde, le droit des femmes à avorter à constitutionnaliser le droit à l'IVG, notre pays feraient également de pionnier et fidèle Afar vocation universaliste, il enverrait un message fort aux pays ou le droit à l'avortement n'existe pas et un message clair aux pays où se doit aujourd'hui est bafoué, je terminerai en rappelant que la constitutionnalisation du droit à l'IVG ne serait pas exclusive de son inscription dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que, au côté du président de la République, nous, nous appelons de nos voeux. C'est dans la perspective de ces combats que nous serons nombreux au groupe RDPI à voter ce texte là. Merci, cher collègue, la parole est à madame la présidente, Laurence Rossignol pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour six minutes chers collègues. Madame la présidente, madame la rapporteure, mes chers collègues, je vais d'abord Madame la rapporteure m'attacher à votre rapport, selon vous, l'IVG ne fait l'objet d'aucune remise en cause aujourd'hui en France, hé bien je ne partage pas votre sérénité les courants hostiles à l'IVG n'ont jamais désarmé depuis 1975 il dispose de moyens financiers considérables, a traîné un international s'appuie sur des institutions puissantes, comme la Fondation Lejeune, ils sont hyper actif sur le net est capable d'organiser comme il y a 15 jours, des manifestations de 600 personnes à Lyon, ce que je prends très au sérieux, aujourd'hui, c'est vrai, ils n'ont pas ou peu de relais affichée dans le monde politique, mais d'autres collègues l'ont dit avant moi qui gouvernera la France dans 5 ans, j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que le risque d'une coalition autour de l'extrême droite n'est pas exclu et j'observe que partout où des conservateurs, des réactionnaires, des populistes, d'extrême droite sont au pouvoir, partout le droit à l'IVG leurs cibles et leur hostilité aux droits des femmes et leur étendard, je ne crois pas Mélanie Vogel a eu la gentillesse de me citer tout à l'heure en effet à une quelconque exception française de l'extrême droite en la matière et pour tout vous dire, ce n'est pas l'intervention de notre collègue représentant d'extrême droite dans le Sénat qui m'a rassuré sur ce point. Vous dites que notre PPL un porte des débats, des États-Unis, mais enfin il n'y a pas besoin d'aller si loin, d'autres l'ont dit avant moi dans l'Union européenne, Malte, la Pologne, la Hongrie et maintenant l'Italie sont dirigés par des formations politiques hostiles à l'IVG, élu sur ces programmes là sur leur hostilité à l'IVG, quant à la Suède déjà la nouvelle coalition a indiqué vouloir mettre un terme à la diplomatie féministe, nous les surveillons avec beaucoup de vigilance, vous affirmez que le Sénat est attaché aux lois Veil et Neuwirth. Permettez-moi madame la rapporteure de souligner que votre attachement est quand même assez minimaliste depuis 75 à loi Veil a été modifié, cette fois, vous l'avez d'ailleurs rappelé comme un acquis collectifs, vous et vos prédécesseurs, vous y êtes systématiquement opposée encore il y a 18 mois lorsqu'il s'agit de voter la loi Gaillot, si on vous avez écouté. L'IVG ne seraient. Si on vous avez écouté l'IVG ne serait toujours pas remboursé en 1982 la loi Roudy a été rejeté par le Sénat, les femmes devraient toujours prouver qu'elles sont réellement détresse les mineurs devrait toujours obtenir l'autorisation de leurs parents et je ne suis même pas sûr que la pilule du lendemain seraient en vente libre, vous êtes terriblement prévisible. Quelle que soit la question dès lors qu'il s'agit d'améliorer l'accès à l'IVG, la réponse est non. Enfin, quelques mots sur la phrase maintes fois entendue qu'il ne faudrait modifier la Constitution que d'une main tremblante depuis 2011, le groupe LR au Sénat a déposé 10 propositions de loi constitutionnelle votre main ne tremble pas toujours et sous les présidences Chirac et Sarkozy, il y a eu pas moins de 5 réforme constitutionnelle. Le vote que nous allons émettre tout à l'heure n'est pas destiné à enrichir les chroniques de droit constitutionnel, c'est un vote politique que la PPL soit adopté ou rejeté le Sénat enverra un signal et ce ne sera pas le même si nous adoptons d'abord nous sécurisons davantage à venir et nous enverrons un message aux femmes. Hé ho progressistes qui revendique affronter l'adversaire de leur liberté, si le Sénat rejette ces PPL personne ne retiendra vos subtilité juridique tous les adversaires des libertés des femmes, tous ceux qui préfèrent les avortements clandestins au droit de choisir ceux-là se sentiront plus fort parce que moins seul et appuyés par une puissante institution la nôtre ils reviendront, car l'IVG le totem des réactionnaires, des conservateurs, des niveaux néofascistes de tout ce qui s'oppose à l'émancipation des femmes. Il y a 8 jours. Nous étions là au même endroit. Ensemble, pour témoigner de notre solidarité avec les femmes iraniennes et nous étions unanimes. Et j'ai dit ce jour là que nous devions combattre avec la même détermination tous les intégrismes et les totalitarismes religieux, tous ceux qui prétendent que des lois de Dieu sont supérieures à celles des hommes, et il n'y a pas de différence entre obliger les femmes à dissimuler leur. Encore et leur interdire de choisir quand et avec qui elles seront. Qui sont les activistes anti-IVG. Qui sont-ils, ces militants qui veulent empêcher les femmes d'avorter qui veulent nous renvoyer aux avortements clandestins Civitas les CD, vive les survivants et d'autres, ce sont tous des militants intégristes et traditionalistes chrétiens, catholiques ou évangéliques qui clament leur hostilité à la liberté des femmes car il n'y a pas plus de liberté pour les femmes dans les idéologies religieuses qui leur impose le port du foulard islamique que dans celles qui leur refusent le droit à l'avortement ou à la contraception, voilà ce que nous voulons faire avec cette PPL, protéger les droits des femmes et dire clairement à ceux qui refusent des valeurs de la République que dans la confrontation avec les intégristes de tout poil, à la fin, grâce à nous, c'est toujours la République qui gagne. Enfin, monsieur le garde des sceaux, madame la ministre. Je n'aurai qu'un mot. Bien sûr, vos 2 interventions nous ont conforté. Mais prenez la main puisque les rédactions ne sont pas bonnes probablement déposer sans une mais vous auriez pu aussi amendé madame la rapporteure parce qu'il n'est pas rare que vous mendier des PPL de l'opposition. Mais, déposer un projet de loi, épargnez-nous ces allers et retours, c'est votre à l'aléatoire, dites que le gouvernement ne soutient pas simplement le parlement mais qu'il ne veut que le droit à l'IVG soit constitutionnalisé. La parole est à Madame Laurence Cohen pour le groupe communiste, républicain, citoyen. Et écologistes Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier le groupe geste d'avoir inscrit dans leur niche cette PPL co-signée par plus de 100 sénatrices et sénateurs, dont les membres de mon groupe, le groupe CRCE cette volonté de constitutionnaliser le droit à l'IVG n'est pas nouvelle : cela fait 10 ans, c'est-à-dire depuis 2012, que le parti communiste porte cette idée notre groupe avait déposé une PPL en ce sens dès 2017 donc avant même la Cour suprême des États-Unis et faute d'avoir pu l'inscrire dans notre espace réservé, nous l'avions proposé et nous avions tenu un débat ici-même dans l'hémicycle, avions-nous tort de vouloir protéger davantage ce droit nos craintes face à la montée des mouvements conservateurs et réactionnaires étaient-elle infondée exagéré, malheureusement non, je ne vais pas faire la liste des pays qui depuis ont pris ou prennent un chemin inquiétant, ça a été fait mais personne ne peut affirmer ici que le monde actuel, ça pèse et va vers un renforcement des droits des femmes, alors avec cette PPL importe ton comme cela a été reproché en commission des lois, un débat lié notamment à l'organisation constitutionnelle propre aux États-Unis, mes chers collègues, en France, pays des lumières, des droits de l'homme, il me semble que des signes concrets et inquiétant existent et nous en avons encore une preuve de la Manif pour tous au groupe ProChoix aux mensonges déversés sur Internet pour culpabiliser et détourner les jeunes femmes de leur projet d'avortement en passant par l'élection récente de 80 9 députés de la droite extrême, la remise en cause du droit à l'IVG constante s'inscrivant dans un tout cohérent d'atteinte aux libertés individuelles, d'autant qu'on ne peut ignorer la fermeture de 58 s'est IVG en 2018, qui s'ajoute à celle de 130 d'entre eux, de 2000 à 2010 à cette casse organisée, s'ajoute ici en France, mes chers collègues, le manque de gynécologues, renforçant les difficultés d'accès et je pourrai agir ajouter l'existence de la double clause de conscience, ou encore la non-parution des décrets pour autoriser les sages-femmes à pratiquer des IVG instrumentales ainsi en France, le droit à l'IVG sans cesse menacée malgré quelques récentes dispositions législatives favorables obtenus, mes chers collègues, contre l'avis de la majorité sénatoriale, et je pense particulièrement à la loi Gaillot maîtriser le corps des femmes vieille lune du patriarcat est un enjeu de pouvoir, sinon comment comprendre qu'il est remis en cause partout, toutes ces attaques sont révélatrices du fait que les femmes sont toujours considérés comme des être mineur qu'il faut encadrer, contrôler car elles ne peuvent décider seul, alors que ce droit soit inscrit dans le code de la santé publique, la question qui nous est donc posée aujourd'hui est la suivante est-ce que ce droit chèrement conquis par la lutte des féministes, des progressistes, progressistes, a besoin d'être protégés au regard des quelques éléments que je viens de citer, cela ne fait aucun doute, et la question de l'emplacement dans la constitution est en réalité secondaire et ne peut servir de prétexte pour ne pas soutenir cette loi, de quoi avez-vous peur, mes chers collègues de dénaturer notre constitution, je remarque que celles et ceux qui s'opposent à la constitutionnalisation du droit à l'IVG et à la contraception, sous le prétexte juridique que cela ne serait pas nécessaire sont les mêmes qui s'opposent systématiquement au renforcement de ce droit et d'une manière générale, qui s'oppose à la conquête de nouveaux droits pour les femmes depuis des années, aujourd'hui encore, que cela vous plaise ou non, les femmes veulent maîtriser leur fécondité et choisir au nom de mener à bien une grossesse notre corps nos choix, nos droits, mes chers collègues, l'heure est à regarder objectivement ce qui se passe en France, à l'aune de ce qui se passe également en Europe où dans le monde ne nous croyons pas dans un état de droit, qui serait meilleur et plus solide qu'ailleurs, le garde des sceaux l'a souligné utilisons au contraire tous les outils de notre disposition pour renforcer notre législation actuelle face à un droit de toute part menacé

Madame la présidente, madame la Ministre, monsieur le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure madame l'auteur de la proposition de loi constitutionnelle, mes chers collègues, la volonté d'inscrire l'interruption volontaire de grossesse et la contraception dans le marbre constitutionnel n'est pas nouvelle et ce n'est pas moins de 6 propositions de lois qui ont été déposées entre fin juin et début septembre 2022 sur les bureaux des 2 assemblées, c'est c'est bien évidemment l'actualité américaine qui fait que nous siégeons cet après-midi, c'est même l'actualité d'une juridiction, la Cour suprême des États-Unis ou un revirement de jurisprudence, l'arrêt d'Obs vers ce Jackson cette année est venu modifier l'arrêt Roe versus Wade du 22 janvier 1973 qui avait accordé une protection fédéral à l'avortement sur le fondement du 14ème amendement de la Constitution des États-Unis, lequel dispose notamment qu'aucun État ne privera quiconque de la vie de la liberté ou la propriété sans procédure légale régulière désormais aux États-Unis d'Amérique, la question de l'avortement est redevenue une compétence des États fédérés. Chers collègues, Mélanie Vogel, vous avez commencé votre votre intervention en disant que la Constitution fondrait le contrat, le c'est donc confié à notre texte fondamental, une fonction qui ne peut évidemment pas être la sienne, je m'explique : si votre proposition de loi a été adoptée dans les mêmes termes au Sénat puis à l'Assemblée nationale, et enfin par une ratification populaire par référendum, c'est le Conseil constitutionnel qui deviendrait l'instance en charge de veiller à la portée du texte lui-même, c'est risquer de déposséder la représentation nationale, de la capacité à modifier les règles qui encadrent l'IVG et la contraception, depuis 2008 le Conseil constitutionnel peut être saisi de QPC qui permettrait de contraire à la Constitution des dispositions législatives plus ancienne encore si donc à des membres nommés par le président de la République, celui du Sénat ou de l'Assemblée nationale qu'il reviendrait d'en décider, qu'ils soient davantage conservateur ou davantage progressiste avec par principe, l'absence de tout contrôle démocratique de cette institution, notre pays, conformément à l'article 1er de notre constitution d'une République indivisible, c'est-à-dire que le législateur dispose d'une plénitude de compétences et les lois appliquées de la même manière, à chacun de nos concitoyens sur l'ensemble du territoire national, à cet égard, aucune comparaison avec les États-Unis n'est possible, je voudrais revenir sur 2 lois qui, aujourd'hui, définit l'accès à l'IVG et à la contraception, d'une part, la loi du 17 janvier 1975 portée par Simone Veil et personne ne peut remettre en cause évidemment les Liens qui unissent le groupe Union centriste et Madame Veil madame Veil est alors ministre de la Santé, elle a porté la loi sur l'IVG qui est venu encadrer la dépénalisation de l'avortement dans notre pays depuis les conditions n'ont jamais cessé d'évoluer avec notamment son remboursement le possible accès d'une femme mineure sans le consentement d'un adulte, la suppression des notions de situations de détresse et de délai obligatoire de réflexion, d'autre part, la loi du 28 décembre 1967 porté par Lucien Neuwirth relative à la régulation des naissances depuis l'accès à la contraception, a lui aussi évolué considérablement au fil des années il semble important de rappeler qu'aucun parti politique n'a jamais appelé à remettre en cause l'IVG dans son principe et encore moins la contraception, nous sortons tout juste des élections électorales majeures, entendu aucun candidat à la présidentielle, y compris aux extrêmes de l'échiquier politique, remettre en cause les acquis de la loi Veil et la loi Neuwirth, aucun candidat à la présidentielle, autrement dit le risque politique que vous invoquez en France en 2022 n'existe pas et c'est tant mieux, notre collègue Mélanie Vogel a insisté en commission sur le fait que justement c'est parce que ce droit n'est pas encore menacé qu'il faudrait modifier notre norme fondamentale qu'après il serait trop tard, cet argument ne m'a évidemment pas convaincue. Par ailleurs, mes chers collègues, n'oublions pas le vrai sujet. Dans un concert dans un contexte de désertification médicale, c'est le membre de la commission délégation droits des femmes qui le dit, l'accès à l'IVG et parfois rendues très difficiles, notamment afin d'obtenir les rendez-vous médicaux obligatoires les plus touchés, ce sont les femmes originaires des territoires ruraux, si le droit existe, il n'est pas appliquée de manière pleine et entière sur le territoire de notre pays, alors avant de s'interroger sur la nécessité avant tout symbolique de l'inscription dans la constitution, nous devons le gouvernement doit se préoccuper de l'effectivité de l'application de la loi, il est vain d'inscrire ce droit dans la Constitution, si au quotidien dans l'ensemble de nos territoires, certaines de nos compatriotes ne peuvent pas, ils ne concrète au sont prévaloir notre commission des affaires sociales et la délégation aux droits des femmes du Sénat se sont intéressés à ses complexités, elles estiment que si sujets repose avant tout sur l'organisation du système de soins et sur des mesures concrètes du pouvoir réglementaire dépassant alors largement le débat que nous avons cet après-midi sur la révision constitutionnelle. En respectant. Les collègues de mon groupe qui ont cosigné cette proposition de loi constitutionnelle ou ceux qui s'apprêtent à voter pour cette proposition de loi constitutionnelle, le groupe de l'Union centriste dans sa majorité suivra les conclusions de Madame la rapporteure Agnès Canayer et ne soutiendra pas l'adoption de ce texte. Merci, cher collègue, de donner la parole à Madame Estelle. Benbassa pour 3 minutes chers collègues. Madame la présidente, madame la rapporteure, monsieur le Ministre, Madame la Ministre, chers collègues, la lutte pour la légalisation de l'IVG a été d'abord incarné par Gisèle Halimi, signataire du Manifeste des 343 salopes ces française courageuse ont alors publiquement assumé leur avortement malgré les poursuites pénales encourues sans suivi le procès de Bobigny en 1972 qui bouleversa l'opinion et ouvrit la voie, 3 ans plus tard, à la fameuse loi Veil, dont je salue l'oeuvre et la mémoire, nous ne voulons pas de retour en arrière, nous sommes probablement quelques-unes dans cette assemblée à avoir avorté. Même aujourd'hui, nous n'osons pas le dire ouvertement, en raison des convenances qui régissent encore notre milieu. J'en fait partie. En revanche, nos tour est de protéger nos filles, nos soeurs et nos concitoyens en leur garantissant formellement le droit de choisir leur maternité sans souffrance sans honte ni culpabilité, nous voulons librement disposer de notre corps aux hommes la société accorde bien le privilège de choisir leur paternité, y compris le droit de reconnaître ou non leur enfant pourquoi la sexualité féminine devrait-elle toujours être contrôlés. Le contexte social est particulièrement difficile, où l'extrême-droite ne cesse de gagner du terrain, la menace d'un Donald Trump français à l'Élysée, dans quelques années, n'est pas illusoire, il nous faut donc légiférer sans plus attendre pour empêcher qu'un jour la majorité au pouvoir puisse décider de revenir sur ce droit fondamental, sans qu'il y face à elle une véritable armure constitutionnelle, je tiens à saluer l'initiative parlementaire de ma collègue Mélanie Vogel et de des cons, signataires de ce texte de ce texte qui permet ce débat et porte le droit à l'avortement et à la contraception jusqu'au sommet de notre ordre juridique en même temps, nous connaissons tous ici la difficulté d'un référendum, si une telle PPL était adopté dans les mêmes termes par deux chambres, particulièrement en cette période politique instable, j'appelle donc l'exécutif va se saisir de ce texte et à le faire sien par un projet de loi je profite également de cette intervention pour demander au président de la République de faire transférer la dépouille de Gisèle Halimi au Panthéon, son combat a contribué à changer la vie de millions de Françaises, sa place est auprès de Simone Veil. Si beaucoup cher collègue, la parole est à Madame Marie Mercier pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Madame le président, monsieur le garde des sceaux, Madame la Ministre, Monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, mes chers collègues, faut-il inscrire le droit à diviser dans la Constitution, cela est-il nécessaire et utile pour garantir son accès aux femmes, à part quelques groupuscules, personne ne remet en cause cette liberté des femmes de notre pays, ni la loi Veil 220000 IVG en France pour 700000 naissances l'inscription de ce droit dans la Constitution, c'est une fausse bonne idée pour ne pas dire une fausse protection c'est un principe général qui serait inscrit dans la constitution de points, les femmes ont le droit d'avorter mais les modalités resteraient défini par une loi qui pourrait en restreindre les concours, même en ce moment, restreindre ses concours par rapport à ceux qui sont en vigueur aujourd'hui, par ailleurs, si les plus compliqué de modifier la Constitution, qu'une loi, c'est pour autant possible et nous l'avons vu j'ajouterai, en tant que médecin élu local parlementaires défenseurs convaincus et déterminé des droits des femmes et de l'IVG que tant de droits humains nécessite d'être protégée tant de nobles causes et de grands principes, mérite d'être sans je suis arrivé, comment imaginer possible de tous les faire entrer dans la Constitution et qui peut déterminer entre une priorité et je pense à l'inceste utile mais non encore moins, peut-être même dangereux s'il devait y avoir référendum campagne et les répercussions pourraient être malheureuse inattendu imprévisible et pour les femmes, à l'heure où notre démocratie est fatigué ou le socle de notre vie commune et malmené inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, c'est peut-être d'ailleurs avoir chipie, confiance en l'avenir de notre démocratie, vous avez si peur de 2027, la seule vraie garantie que nous veillons à ce que ce droit demeure consiste à protéger à animer notre vie démocratique à éduquer nos enfants à la démocratie au vote au respect de l'autre à la protéine sont des plus fragiles, le le populisme l'ultraconservatisme les dérives autoritaires, les gouvernements rétrograde amène une régression démocratique et menace le droit à l'avortement, notre vrai combat et là d'ailleurs à l'observation du monde, en quoi la constitution, ça aurait été un obstacle aux ennemis de la démocratie et du droit des femmes, il y a là une naïveté à le penser, peut être une fausse des politiques à prétendent le contraire, or il faut se parler vrai, se parler juste sanctuariser le droit à l'IVG passe par la préservation de nos institutions, très différente des États-Unis par exemple, et à la préservation, je le redis de notre démocratie, alors y a-t-il quelque chose à faire : ben oui, oui, une loi doit être assortie d'une obligation de moyens, il faut soutenir les plannings familiaux, promouvoir les médecins et les infirmiers scolaires, lutter contre la sous-densification médicale et les inégalités territoriales une maternité qui ferme, c'est potentiellement aussi un centre IVG qui disparaît dans une scène du film Simone on voit Simone Veil, ministre de la Santé, refusé de rentrer dans une chambre vide, elle refuse de faire semblant en adoptant des postures purement symbolique, quelle leçon les femmes méritent en effet mieux qu'à faire semblant qu'une inscription dans la Constitution, au cas où qu'un faux-semblant, en réalité, alors oui il faut prévenir et protéger, il faut prévenir en informant par une éducation sexuelle sérieuse nos jeunes garçons et filles, il faut protéger les femmes, c'est-à-dire permettre un égal accès à l'IVG pour toutes dans des conditions médicales correctes par des professionnels formés et à leur écoute, c'est-à-dire aussi les accompagner ensuite dans l'après, avec une prise en charge adaptée, voilà ce qui servirait réellement la cause des femmes voilà j'étais nous sommes en droit d'exiger, voilà ce que nous sommes en droit d'obtenir. Merci, cher collègue. La discussion générale est Close, la commission n'ayant pas et là. De textes, nous passons à la discussion de l'article unique de la proposition de loi constitutionnelle initial et j'ai une demande de prise de parole de monsieur le questeur Philippe Bas. Merci madame la présidente, Madame Rossignol, je la cite veut envoyer un message, le garde des Sceaux, je le cite, nous dit quel beau symbole ce serait. Mais nous devons écrire le droit. Nous devons écrire la législation et de ce point de vue, je veux dire ma conviction que ce texte n'est pas seulement inutile : il serait également inefficace du point de vue des objectifs que s'assigne ses auteurs et j'attends en juriste qu'on vient de me démontrer le contraire, tout d'abord, il était inutile : pourquoi est-il inutile parce que le Conseil constitutionnel dès 1975 a validé la loi sur l'IVG, en soulignant que son article 1er qui énonce le respect de tout être humain dès le commencement de la vie doit pouvoir connaître des limites et ces limites en cas de nécessité, c'est justement l'IVG et en 2001, le Conseil constitutionnel est allé beaucoup plus loin puisqu'il a dit que ça résultait de la liberté de la femme enceinte qui trouve son fondement dans les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est donc inutile, c'est aussi inefficace, toutes les avancées, selon ce qui se sont exprimés dans ce sens, qui ont été mises en place depuis la loi Veil, le délai passé à 12 et 14 semaines le remboursement, la suppression de la condition de détresse le raccourcissement du délai de réflexion, l'accès des mineurs à l'IVG, hé bien, aucune de ces avancées entre guillemets ne serait susceptible d'être protégé par la rédaction, qui a été proposé, c'est très simple, à partir du moment où on programme le libre accès à l'IVG mais qu'on reconnaît qu'il ne peut pas être illimité, le législateur garderait pleinement compétence pour apporter des restrictions à l'exercice du droit à l'IVG, c'est donc à la fois inutile. Et merci Jean Moloui efficace merci, la parole est à monsieur Éric. Merci merci madame la présidente, il y a pas que les civilisations qui sont mortels, il y a également les édifices juridique la conquête en général se fait par le droit, mais le recul et les remises en cause peuvent également se faire par le droit et croire que le droit et le droit notamment dégagé par le conseiller le conseil constitutionnel suffit à nous sauver, est une grave erreur, parce que c'est comme croire l'histoire du loup et des 3 petits cochons et penser que justement le LOU parce que le loup est présent, on a eu un petit louveteaux qui s'est exprimé tout à l'heure. Hé bien, le loup est toujours là et il peut souffler le vent et détruire les édifices juridique dans la décision Roe versus Wade ou plus exactement dans la dans la façon dont elle a été remis en en cause. Les arguments sont très simple, c'était de dire que cette décision n'était qu'une décision juridique que elle constituait une décision erronée et qu'elle constituait un abus d'autorité judiciaire et dans les décisions préparatoires qui ont été menées, il y avait des considérations qui n'étaient pas des considérations juridiques, comme je cite le fait que, un être humain qui n'est pas encore né, tuer un être humain qui n'est pas encore né, pose des problèmes de morale, ça ce n'est pas du droit, c'est de l'idéologie et quand on dit un petit peu plus loin que la question de la vie des américaine n'a pas été vraiment transformé pas par la décision Roe versus Wade s'est encore de de l'idéologie, alors en effet, ce texte aurait pu ah mais être améliorée, vous auriez pu l'améliorer mais vous n'avez choisi de ne pas le faire je finirai par un point le grand puisque Philippe Bas est sensible au droit : le grand constitutionnaliste anglais William autre disait au XIXe siècle, qui avait deux partie dans la constitution, il y avait une partie efficace et il y avait une partie qui suscite le respect, hé bien j'aurais voulu que cet après-midi en francs, ensemble nous auriez nous aurions pu construire justement un texte qui pour toutes et pour tous, suscite le respect. Mais la parole est à Madame Michèle Meunier. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, Madame la Ministre, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous réunit, ce soir, vise à inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution avec celles et ceux qui ont déposé ses propositions de loi, nous voulons affirmer encore avec plus de détermination, ce droit des femmes à disposer de leur corps dans notre pays, je ne reviens pas sur les arguments juridiques échangés ici est promu par la droite de ces bancs pour repousser cette inscription de la dans la Constitution, notre combat est politique et symbolique, Laurence Rossignol, la race, elle a rappelé à la tribune, il vise à soutenir encore et toujours les femmes qui souhaitent une IVG, nous assistons impuissante à un recul du droit d'accès à l'avortement dans le monde, mais aussi en France où ce droit est de plus en plus attaqué par des franges minoritaires et réactionnaire, qui se base sur des fondements religieux personnel pour les imposer au plus grand nombre, nous ne pouvons pas laisser passer cela dernièrement à Nantes lors d'un rassemblement au soutien aux femmes dans le monde, privés du droit à l'avortement des banderoles haineuses ont été brandies par des anti-des inscriptions, on salue on salit nos trottoirs, assimilant l'IVG à un génocide, cela n'est pas tolérable, j'attendais de l'ensemble de nos groupes politiques au Sénat une forme d'unanimité de consensus dans ce soutien à la constitution constitutionnaliser elle n'est pas au rendez-vous et je le regrette, combien de temps encore notre majorité va-t-elle entretenir le flou avec cet arc réactionnaire, ne pensez-vous pas que ne votre famille politique risque de se déshonorer par un tel silence Madame de La Gontrie. Merci madame la présidente, évidemment, notre groupe votera ce texte et nous remercions Mélanie Vogel d'avoir pris l'initiative pour son groupe de le situer dans un temps de débat parlementaire qui peut lui être consacré, nous avons été coauteur avec elle. Mais j'ai entendu des propos à la droite de cet hémicycle qui me surprennent parce que je les avais connu dans d'autres circonstances plus courageux, plus sincère car les arguties juridiques avancés par Philippe Bas ne sont pas opérants. Et ce qui est très intéressant, c'est de devoir finalement avoir recours à ces arguties quand on n'a pas le courage de dire simplement : je suis hostile à l'IVG. Pourquoi ne sont-ils pas opérants par. Président bah président bah. Vos arguments ne sont pas opérants parce que vous vous référez à une jurisprudence,

se référer à la jurisprudence, vous le savez bien président bah, c'est une faiblesse, pourquoi, parce que cette jurisprudence peut évoluer, on a suffisamment parlé de l'exemple américain, mais c'est une bonne illustration, vous le savez très bien la jurisprudence du Conseil constitutionnel n'est qu'une jurisprudence, ce que nous voulons c'est que désormais ce soit inscrit dans la loi vous dites ici que nous sommes des législateurs, oui nous sommes des législateurs, nous sommes aussi des responsables politiques et nous avons aussi à référer aux électeurs et aux Français, et donc je le dis au président bah, ayez le courage d'assumer votre position, vous tous, à droite, qui vous a prêté à refuser ce texte. alors je vais mettre. Trop voix l'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi constitutionnelle le vote sur l'article vaudra vote sur l'ensemble de la proposition de loi, il y a-t-il des demandes d'explications de vote, hein, monsieur le questeur bah. Madame la présidente, tout d'abord, je me suis senti insulté par les propos de Madame de La Gontrie. Je n'y reviens Je n'y reviens pas, mais je tenais à le dire, je voudrais dire ici que nous sommes tous ouverts au débat et nous avons voulu que ce débat ait lieu, nous aurions pu l'empêcher. Mais. Encore faut-il que l'objet du débat soit au coeur des échanges à aucun moment, nous disons : nous n'avons discuté de la réalité du texte qui nous était soumis la réalité de ce texte, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un texte inefficace et inutile si les auteurs de ce texte avait voulu consacrée dans la Constitution, l'article 1er de la loi Veil qui en fonde les principes fondamentaux, alors peut-être, aurions-nous accepter d'en discuter ensemble, puisque nous vivons depuis maintenant près de 50 ans sur ces principes qui sont des principes essentiels, validée par le Conseil constitutionnel qui empêcherait aujourd'hui la suppression de l'IVG, en revanche il n'empêcherait pas malgré l'adoption de votre texte des retours en arrière sur le périmètre de l'IVG, c'est une réalité juridique, et ça n'est pas la peine d'agiter des idées générales qui sont parfois aussi des idées creuses, je regrette de le dire, nous avons à discuter d'un texte, nous ne l'avons même pas fait ici, nous aurions dû le faire, c'est un mauvais texte revenait avec un bon texte, nous en reparlerons. Merci monsieur radié. Quel est l'argument des porteurs de cette proposition de constitutionnalisation de l'IVG, quel est l'argument juridique qui reposent sur des déclarations qui reposerait sur des déclarations sur des prises de position. Peut-être que, un jour, s'il y a une catastrophe économique, militaire environnemental ou je ne sais trop quoi, peut-être qu'il y aurait un pouvoir qui seraient amenés à vouloir changer peut-être la loi. Vous reposez votre démarche repose sur du fantasme, vous êtes dans une volonté de créer une sorte de phobie, vous êtes en réalité dans une volonté de diviser, de faire de l'agitation de faire de la provocation jusqu'à, comme l'a si bien dit notre collègue Philippe Bas jusqu'à insulter jusqu'à insulter les sénateurs qui n'abonde pas dans votre sens, jusqu'à la dernière jusqu'à la dernière lettre de votre texte, parce que même quand on on ne met pas en cause et personne ici ne remet en cause le droit à l'IVG, même quand on ne remet pas en cause l'IVG vous pousser le bouchon toujours plus loin, vous êtes constamment dans la provocation pour exister pour exister politiquement, c'est un coup politique que vous essayez de mettre en place aujourd'hui, cela a été très bien dit par l'ancien secrétaire général, encore une fois du Conseil constitutionnel, vous êtes dans l'agit-prop qui n'est vraiment pas propres, pour le coup, vous êtes dans la propagande toujours du wokisme que vous voulez toujours porté ça ne prend pas ça ne prend pas sur moi, vous pourrez toujours compter sur moi pour dénoncer vos méthodes qui nous rappelle les méthodes de Fouquier-Tinville, sauf qu'aujourd'hui, hé bien Monsieur Fouquier-Tinville est sur les talons. Merci, merci, cher collègue, même la présidente Rossignol. D'abord, un autre collègue Ravier, je ne crois pas un mot de ce qu'il nous dit. Je ne crois pas un mot de ses dénégations. Luis le courant politique auquel il a pas appartient les courants politique auquel il appartient, les les sauteurs auquel il se réfère parle continuellement d'avortement de confort et d'avortement de con de convenance, je sais depuis des années que les mots avortement de confort et avortement de convenance non qu'une finalité : réduire le droit des femmes à l'avortement, en soumettant leur accès un jugement extérieurs sur les raisons qui les amène à avorter. Donc voilà pourquoi vous êtes un représentant d'un courant politique dangereux pour l'IVG quant à mes collègues de droite, j'écoute avec intérêt leurs explications juridiques mais je l'ai dit tout à l'heure, je vais le redire : j'ai un peu d'expérience avec vous ces 12 ans que je suis là, bientôt 12 ans que je défends les droits des femmes à disposer de leur corps, 12 ans que je défends des textes en faveur de l'égalité d'accès à l'IVG en faveur la l'allongement des délais, en faveur de la suppression de la condition de détresse 12 ans que j'ai défendu un texte ici en tant que ministre pour sanctionner les sites internet qui trompe les femmes en les attirant sous prétexte de les informer pour les dissuader de recourir à l'IVG, pas une fois, pas une fois vous n'avez trouvé que ce que nous nous disions valait la peine d'être votée, comme dit l'adage, au bout d'un moment des pointillés, ça fait une ligne et quand, jamais, jamais, jamais, le droit ne vous convient, c'est que c'est plus le droit de sujet c'est le fond du dossier dont nous discutons alors voter une fois une fois un texte en faveur de d'IVG et après je vous croirai. Merci madame la présidente, s'il vous plaît, madame la présidente, monsieur Brisson a seule la parole, merci, s'il vous plaît. Merci madame la présidente, je n'avais pas l'intention d'intervenir j'intervient après les propos de Madame un country et de Madame Rossignol et je veux dire à Philippe Bas toute notre solidarité, notre amitié. Je ne suis pas juriste comme Philippe veut pas mais je sais que 3 choses : d'abord ce que la France n'est pas l'Amérique, que le code textes constitutionnels et juridiques ne sont absolument pas les mêmes que la France, la France n'est pas un état fédéral qu'elle n'a pas tranché entre l'État fédéral et les États fédérés et que son rapport à la Constitution, historiquement, n'est absolument pas le même que les États-Unis d'Amérique. veux dire, deuxièmement et avec force. Comme que je suis favorable à l'ensemble des lois qui autorise le trois à l'interruption volontaire de grossesse et que je me battrai. Pour les défendre, si elles étaient menacés. C'est ma conviction. Mais j'ai aussi ma conviction, c'est que notre constitution ne pourrait pas être soumises au débat et aux émotions qui viennent d'outre-Atlantique, j'ajouterais concernant la défense des droits des femmes, dont Madame Rossignol veut dans cette assemblée, faire son monopole, j'ajouterai que notre majorité sénatoriale avec les travaux de la délégation aux droits des femmes en particulier a fait dans le dernier rapport auquel vous avez participé Madame Rossignol, mais aussi avec Alexandra Borchio Fontimp de grandes avancées et que c'est ici que ça s'est passé et que c'est la majorité sénatoriale qui a porté ce débat. Merci, cher collègue Madame Cohen. Mes chers collègues, moi je trouve que dramatiser le débat comme vous le faites sur les bancs de droite, ça n'est pas digne, je vous ai écouté, je vous ai écouté, ça n'est pas digne du Sénat, pourquoi je dis ça parce que, quel que soit ce que l'on peut porter jusqu'à présent, on a un respect mutuel, les uns envers les autres, je ne parle, je ne parle pas, pas de la droite extrême à laquelle je ne réponds pas seul, ce serait le lui donner trop tôt, trop d'honneur et je ne confonds pas mais mes chers collègues, à droite, vous devez prendre quand même vos responsabilités les lois qui ont été jusqu'à présent voter y compris loi Veil, une très grande dame extrêmement courageuse, pourquoi cette loi arrive au Parlement, d'abord par la mobilisation des femmes, des féministes, parce que rien ne s'obtient sans qu'il y a un rapport de force dans la rue, ça c'est la première chose et la 2ème chose, elle n'aurait jamais été voter s'il y avait pas eu la mobilisation totale de la gauche, donc ça c'est aussi quelque chose d'important, ça ne vous plaît pas, mais ce sont les faits c'est factuel, alors au lieu d'essayer de prendre des prétextes jusqu'à présent, moi j'ai l'habitude depuis 2011 d'avoir des c'est un Sénat responsable quand il y a une loi qui est pas tout à fait bien ficelé, il y a des propositions pour la la pour faire en sorte qu'on puisse la voter ensemble si vous étiez vraiment d'accord pour protéger le droit à l'interruption volontaire de grossesse, vous l'auriez fait le fond du problème, c'est que vous allez envoyer un message qui dit que vous n'êtes pas d'accord et c'est ce que l'on vit, à chaque fois que l'on défend le droit des femmes à disposer de leur corps, c'est la réalité des faits que ça ne vous plaisent pas changer vos vote. Monsieur le Président, buffet. 1er point, vous ne pouvez pas dire ma chère collègue madame de La Gontrie à Philippe Bas, qu'il est contre l'IVG, il a été, il a rappelé tout à l'heure, oui mais la vérité et le respect des gens est aussi une des règles de notre haute assemblée, il a été le plus proche collaborateur de Madame Simone Veil, il a lui-même rédigé une partie du texte et il a soutenu. Est-ce que vous le contestez est-ce que vous consiste contester est-ce que vous contestez se fait la polémique, hé bien sûr hé ben voyons, votre réponse suffit à qualifier votre attitude, je n'en dirai pas plus. J'ai entendu avec intérêt les propos de Monsieur Gontard tout à l'heure à la tribune, reconnaissant à demi-mot la difficulté du texte, les problématiques posées tout en disant que, il faudrait trouver le moyen de progresser, il y a plusieurs initiatives, le ministre nous l'a dit tout à l'heure parlementaire Mélanie Vogel au sein de notre assemblée, mais également d'autres collègues à l'Assemblée nationale, il y a donc une mobilisation réelle sur cette thématique, moi je crois que. Je crois que ce qui serait intéressant, c'est que le gouvernement parce qu'il est le gouvernement. Puisse mettre un peu d'ordre dans tout cela et ça nous permettrait peut-être d'avancer dans un débat serein sérieux avec effectivement des propositions qui pourrait peut-être venir de différents bancs de cette assemblée, mais qui en tous les cas ne sortirait de l'impasse de ces discussions qui ma foi parfois dérape de façon tout à fait inutile, alors que nous sommes tous d'accord, sans exception, pour protéger les droits des femmes, naturellement, alors de grâce, si on pouvait terminer ce débat sans invectives et on était à peu près sérieux parce que le débat que nous vous me donner les images que nous venons de donner, c'est potentiellement celle qui pourrait se passer en cas de référendum en France, je pense qu'on n'a pas besoin de cela sur une initiative du gouvernement, nous aurions à ce moment-là d'autre porte de sortie juridique beaucoup plus sérieux, je vous remercie. je, je suis désolé de de rompre peut être cette proposition, mais je voudrais répondre à aux collègues Brisson Jean Jean j'entends bien que vous nous donniez des leçons et que vous essayer aujourd'hui de défendre une loi, une loi qui, je vous rappelle, vous n'avez pas voté une loi qui vous avez même voté la motion préalable en première lecture et en 2ème lecture alors venir nous donner maintenant des leçons de morale sur la défense de l'IVG et la défense du droit des femmes, c'est un peu fort de café. Merci madame Gréaume. Chers collègues, je vais pas faire le procès d'intention de personne, je vais simplement rappeler la loi française, la loi française, elle garantit le respect de l'autonomie personnelle sur les droits procréation et l'accès aux soins et services de santé toute personne a le droit à une contraception adaptée gratuite ainsi que le recours librement à l'IVG, le fait de passer cette loi dans la Constitution devient un droit fondamental et assure la pérennité à travers la stabilité de la constitution du respect de l'autonomie personnelle. On n'oblige personne, c'est simplement la personne qui le désirent, pour pouvoir pouvoir y accéder, je rappelle que c'est sur l'autonomie personnelle merci. mettre aux voix l'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, en application de l'article 59 du règlement, le scrutin public et de droit, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin sera ouvert dans quelques instants, le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter, le scrutin est clos. Alors voici le résultat du scrutin numéro 8 sur l'ensemble du texte, et compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs aux groupes politiques et notifié à la présidence, nombre de votants 336 Nombre de suffrages exprimés 311 pour l'adoption 139 contre 172 le Sénat n'a pas adopté. Alors je vais suspendre la séance pour quelques instants afin de permettre à chacun de s'installer pour le prochain point à l'ordre du jour, la séance est suspendue.

La séance est reprise, l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale visant à faire évoluer la formation de sages-femmes dans la discussion générale, la parole est à Madame Agnès. Hein Le Bodo, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. La Ministre c'est à vous.

votre assemblée se prononce cet après-midi sur une proposition de loi inscrite à l'ordre du jour du Sénat à l'initiative du groupe écologiste solidarité et territoires le gouvernement accueille favorablement la mise à l'ordre du jour de cette proposition de loi le le fruit, vous le savez, d'une initiative parlementaire à l'Assemblée nationale, sous la précédente législature, le groupe Agir ensemble à l'Assemblée nationale, qui était le mien avait défendu cette proposition visant à mieux reconnaître les spécificités de la profession des sages-femmes, alors qu'elle joue un rôle essentiel dans l'accès à l'offre de 1er recours je tiens d'ailleurs à souligner l'implication de l'Ordre des sages-femmes, aux côtés de l'ensemble des ordres réunis dans le cadre du Clio santé de la signature, la signature, le mercredi 12 octobre dernier d'un accord proposant des solutions concrètes en matière d'accès à la santé pour nos concitoyens face à la situation d'urgence que nous connaissons cet accord apporte des solutions inédites en vue de libérer du temps médical et répondre aux besoins des Français dans tous les territoires, grâce au développement de l'interprofessionnalité le fruit de ce travail collectif constitue une avancée majeure, elle s'inscrit pleinement dans la démarche de la refondation engagée par François Braun et moi-même, dans le cadre du CNR santé lancé au Mans le 3 octobre dernier. Parmi les propositions désordres figurent l'amélioration de l'attractivité des professions de santé, il s'agit de mieux valoriser les compétences des professionnels de santé au travers de leur formation initiale et continue, il s'agit aussi de garantir une démographie des professionnels de santé, cohérente avec les besoins de la population, c'est en effet une nécessité et cette proposition de loi constitue une partie de la réponse, elle constitue en effet un nouveau pas vers l'intégration universitaire de la formation initiale des sages-femmes l'inclusion des formations paramédicales et de maïeutique dans l'université permettra le développement de la recherche, par exemple en sciences, infirmière en réadaptation et en maïeutique l'objectif, c'est que tous les étudiants en santé apprennent à coopérer dès les bancs de l'université et bénéficient des mêmes droits et des mêmes services que les étudiants inscrits dans un cursus LMD, nous avons avancé sur ce sujet, même s'il reste encore du chemin à parcourir, depuis la loi du 21 juillet 2000. La transformation en particulier de plusieurs facultés de médecine en faculté de santé à accélérer les rapprochements avec les écoles de maïeutique la loi d'organisation et de transformation du système de santé du 24 juillet 2019 a ouvert la voie à des expérimentations en la matière et relancer le processus d'intégration universitaire des écoles de maïeutique, la création d'une section du Conseil national des universités en 2019 constitue une étape supplémentaire dans le renforcement du caractère universitaire de la formation, une mission relative à l'université Ariza Sion des formations en santé, en lien avec les services du ministère de la Santé et de l'enseignement supérieur sera prochainement confiée au professeur Christine Amirati et l'inspection générale de l'enseignement supérieur et de la recherche sera également mandaté sur ce sujet. La création d'un statut de maître de stage universitaires en maïeutique prévue par l'article 1 bis se constitue une réponse aux besoins d'encadrement des étudiantes et des étudiants, il était essentiel cependant que ce statut fasse l'objet d'un travail plus large à des fins d'harmonisation avec les autres professions en ce sens, un groupe de travail relatif à la maîtrise de stage universitaire associant les acteurs de la formation et les représentants des étudiants et employeurs sera lancée cet Automne par la DGOS. La rédaction du 3ème alinéa de cet article sur la formation du maître de stage universitaire a pu susciter des interrogations au sein de la communauté universitaire, nous travaillons sur ce sujet, en lien étroit avec la Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche je tiens ici à dissiper les éventuelles inquiétudes, les conditions de l'agrément des sages-femmes sont renvoyées à un décret en Conseil d'État, et même si la rédaction actuelle, précise une formation obligatoire auprès de l'université ou de tout autre organisme habilité, il ne s'agit pas, en réalité, d'élargir au-delà des centres de formation actuelle votre commission l'avait d'ailleurs utilement souligné lors de vos débats en commission la rédaction prévue par l'article 1er, reprend les dispositions de l'article L 41 31 6 du code de la santé publique qui concerne la filière de médecine en cohérence dans le cadre de l'élargissement de la maîtrise de stage universitaire à la filière de maïeutique, il est plus adapté de maintenir ce dispositif, le code de la santé publique a été modifié par la loi au TSS, du 24 juillet 2019 pour permettre au delà des organismes habilités par l'Agence nationale du développement professionnel continu aux universités de former des praticiens agréés maître de stage, des universités au final, ce sont bien les universités qui donneront les agréments au maître de stage, universitaire. Je reviens à la création d'une 3ème cycle d'études de maïeutique prévues par cette proposition de loi, vous le savez, l'émission des sages-femmes ont été progressivement élargi depuis 2009, elle couvre désormais de suivi de prévention et de contraception des femmes tout au long de leur vie, tant en ville qu'à l'hôpital, le suivi de la santé de la femme, le suivi des femmes avant et après leur accouchement s'est par ailleurs ouvert sur une prise en charge en ville cette nouvelle mission justifie une adaptation de la formation initiale, le gouvernement soutiendra la proposition de loi dans sa version issue des travaux de votre commission par amendement de Madame la rapporteure, la commission des affaires sociales a choisi de reporter l'entrée en vigueur de la réforme à la rentrée universitaire 2024, c'est-à-dire aux étudiants entrant en année de pas là à la rentrée universitaire 2023 le gouvernement partage pleinement cette analyse, le maintien du dispositif actuel aurait conduit à embarquer dans la réforme, les actuellement les étudiants actuellement en 2ème année et troisième année de 1er cycle il était judicieux de décaler son entrée en vigueur, pour gérer dans de bonnes conditions, l'harmonisation des différents cycles de formation entre la préparation des terrains de stage supplémentaires et l'impact de l'année blanche en 2028. Le gouvernement soutiendra cette proposition de loi d'ailleurs saluée par les représentants de la profession, à l'issue de son examen à l'Assemblée nationale, elle avait fait l'objet d'un soutien unanime des députés, je formule le voeu qu'il en soit de même au Sénat, je vous remercie.

Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues la proposition de loi que nous examinons, a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, en novembre dernier, comme en commission des affaires sociales au Sénat le 5 octobre. Merci pour les femmes, cette phrase lancée par des sages-femmes, lors de la dernière audition signe l'attente forte de la profession quant à l'adoption de ce texte visant à faire évoluer la profession de sage-femme et cette phrase : nous leur adressons au retour, merci aux sages-femmes les sages-femmes se sont à près de 97 % des femmes mobilisés pour la santé des femmes lors des auditions à de nombreuses reprises, une question a été posée par des sages-femmes, mais pourquoi si peu de considération et la question se prolongeait est parce que nous sommes des femmes qui prenons en soin les femmes le Champ de compétences des sages-femmes et le plus important d'Europe et n'a cessé de s'étendent ces dernières années la France reconnaît depuis plus de 2 siècles caractère médical de la maïeutique et confie aux sages-femmes des responsabilités plus importantes qu'ailleurs en opérant un accompagnement global des femmes et des familles, les sages-femmes pratiquent un métier du Caire du prendre soin, connus pour leur présence en salle de naissance, elles effectuent aussi la surveillance gynécologique le suivi prénatal post-natal, celui du nouveau-né, et ce dans la maîtrise de la frontière entre physiologique et pathologique, malgré ces avancées majeures contribuant asseoir son rôle, la profession vit actuellement un profond mal-être, elle a la conviction depuis trop longtemps de ne pas être reconnu et l'a exprimé ces derniers mois à plusieurs reprises les conditions de travail des sages-femmes à l'hôpital se dégrade le taux d'encadrement, il est toujours fixé par des décrets de périnatalité de 1998 qu'il serait temps de réviser leur formation ne s'est pas adapté suffisamment et demeure établi sur un modèle hospitalier régional correspondant à celui des professions paramédicales. Leurs conditions de rémunération et leur statut ne correspondent pas, de l'avis de toutes les organisations représentatives de la profession aux responsabilités aujourd'hui exercer, il faudrait que la courbe de rémunération reflète celle de l'élargissement des compétences, l'attractivité de la formation en maïeutique et à travers elle de la profession semble d'ailleurs se dégrader à la rentrée 2022 20 % environ des places offertes en deuxième année de maïeutique sont restées vacantes les étudiantes font état d'une formation incomplète dont l'intensité seraient pourtant bien supérieure à celle d'autres formations médicales 70 % dans 13 déclarent souffrir de symptômes dépressifs, or la profession de sage-femme à l'hôpital comme en ville, est essentiel à la santé des femmes et à la santé publique partout sur le territoire, à cet égard le récent rapport sur la santé périnatale de santé publique France fait état d'une situation préoccupante de la santé périnatale de façon globale en France et rappelle que l'état de santé de la petite enfance et de l'enfance conditionne la santé à l'âge adulte, la présente proposition de loi ne résoudra pas l'ensemble des difficultés auxquelles la profession est confrontée, elle pose des jalons d'une meilleure reconnaissance de la profession, ainsi la proposition de loi entend en 1er lieu renforcer le caractère universitaire de la formation en maïeutique, l'article 1er vise à achever l'intégration universitaire des formation de sages-femmes initiée par le législateur, il y a plus de 13 ans, ce processus est aujourd'hui à l'arrêt, d'après le ministère, seulement 14 écoles des 35, école de sage-femme sont intégrés à l'université, la majorité des écoles de bord donc adossé un centre hospitalier, ce modèle qui correspond à celui des formations paramédicales n'est pas adapté à la profession de sage-femme il ne favorise pas notamment le développement de la recherche en maïeutique, c'est pourquoi le texte que nous examinons substitut à la faculté d'intégration, une obligation assortie d'un délai l'intégration des écoles de sages-femmes à l'université devra être achevé au 1er septembre 2027 ce délai nous semble nécessaire en regard des nombreux obstacles, y compris en terme de rémunération qui, localement, ont souvent entravé le processus d'intégration, la loi fixe également les modalités de cette intégration, les écoles de sages-femmes seront intégrés préférentiellement c'est important aux unités de formation et de recherche en santé mixte réunissant donc plusieurs professions médicales et seulement quand cela n'est pas possible, elles seront intégrées aux UFR de médecine ces dispositions, soutenu par l'ensemble des organisations de sages-femmes auditionné permettent de préserver l'autonomie pédagogique et de gouvernance des écoles de sages-femmes tout en favorisant la nécessaire collaboration entre professions médicales interdépendantes la maïeutique n'est-ce pas l'art de faire accoucher les esprits afin d'encourager le recrutement d'enseignants chercheurs dans la discipline, l'article 3 vise par ailleurs à faciliter la conciliation des activités d'enseignement et de recherche avec le maintien d'une activité clinique qu'elle soit ambulatoire ou à l'hôpital, contrairement aux autres professions médicales, les sages-femmes ne bénéficient pas aujourd'hui d'un statut leur permettant de cumuler ses activités. Malgré l'ouverture en 2019 d'une section maïeutique par le Conseil national des universités, le recrutement de sage-femme enseignants-chercheurs reste marginal au milieu de cette année, notre pays comptait une professeur des universités, on dit quelquefois, une une 2ème est en cours et quelques dizaines de maîtres de conférence, la recherche en maïeutique est peu développé alors même que la France compte parmi les pays où la formation est la plus longue et où la profession exerce plus de responsabilités, la proposition de loi vise en 2ème lieu à renouveler profondément le contenu de la formation des sages-femmes pour l'adapter aux mutations de la profession, elle crie, cela a été dit à statut de sage-femme agréée mère maître de stage, des universités, inspiré de celui existant pour les médecins généralistes, ce statut permettra de mieux encadrer les stages en ambulatoire et d'accompagner leur développement en cohérence avec les nouvelles conditions d'exercice de la profession, le gouvernement doit cependant réfléchir à la manière de mieux encadrer et qui a, également, les stages à l'hôpital, les personnes auditionnées ont fréquemment décrit comme un terrain de stage difficile et ont regretté le manque de valorisation dans la loi de la fonction de référent à l'hôpital, surtout l'article 2 de la proposition de loi réforme en profondeur le contenu de la formation, il crée un 3ème cycle d'études de maïeutique lors d'une audition, une sage-femme soulignait enfin un 3ème si, comme pour les autres professions médicales parallèlement une révision de l'ensemble des référentiels de formation est également prévue est nécessaire, les étudiants obtiendront désormais à l'issue de leurs études et après soutenance d'une thèse d'exercice, un diplôme d'état de Docteur en maïeutique cette mesure soutenue par l'ensemble des organisations de sages-femmes que nous avons auditionnés réduira l'intensité d'études jugées trop dense enrichira leur contenu pour mieux tenir compte des nouvelles compétences confiées à la profession comme de la diversification des modes d'exercice, elle favorisera nettement le développement de la recherche, enfin, cette proposition de loi vise à conforter la reconnaissance des sages-femmes comme profession médicale, le 4ème Arctique invite à modifier la classification des sages-femmes dans de nomenclature de l'Insee, la statistique est elle aussi traversée par le Jean, bien plus qu'un miroir, elle participe à créer des catégories nombre de sages-femmes auditionné s'en réjouissent, car, selon les mots d'une d'une d'entre elles, c'est un peu notre histoire, c'est un peu l'histoire de notre vie, de ne pas être dans la bonne case si la commission a approuvé ces dispositions, elle a toutefois modifié leurs modalités d'application, le texte imposait la réforme aux étudiants, actuellement deuxième et troisième années d'études qui sont, qui se sont engagés dans cette filière, sans savoir que celle-ci serait allongée seul cet échéancier ne permettait pas d'assurer la cohérence du cursus pour tenir compte des inquiétudes des étudiants comme des enseignants, la commission a adopté 2 amendements visant à à remporté la réforme à la rentrée universitaire 2000 vingt-quatre et elle ne l'appliquer qu'aux étudiants qui entreront à compter de cette date, en deuxième année ce report facilitera la gestion de l'année blanche sont sortis de sages-femmes diplômés que la réforme générera nécessairement ce soit qui permettent également d'établir les nouveaux référentiels de formation en concertation large avec l'ensemble des parties prenantes, en conclusion, ce texte est à la fois nécessaire et urgent à cet égard, j'aurais souhaité vous proposer mes chers collègues, son adoption en termes identiques à ceux de l'Assemblée nationale, afin qu'il puisse entrer en vigueur le plus rapidement possible, mais si les inquiétudes partagées relatives au calendrier, nous ont conduit m'conduit à proposer à la commission des années, des affaires sociales de le modifier ce souhaite toutefois que ce texte soit rapidement mis à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Else Joseph ah pour le groupe Les Républicains et pour cinq minutes. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues est-ce que ça oui, ce que vous savez pourquoi on dit sage-femme non pas parce que la femme est sage, mais parce que c'est une personne qui connaît les femmes, donc ça chez donc messieurs que l'on peut être homme et sage-femme le texte qui nous est proposé qu'une bonne nouvelle pour les sages-femmes, c'est non seulement la reprise des propositions de l'IGAS sur leur formation, mais c'est d'abord et avant tout la prise en compte d'une revendication légitime formulées depuis des années par celles et ceux qui exercent un des plus beau métier du monde et surtout une profession dont les missions ont évolué et qui vont désormais de la déclaration de grossesse au suivi post-natal et hors du Champ de la grossesse avec un pouvoir de diagnostic et un droit de prescription élargit les sages-femmes assurent des responsabilités médicales dans un cadre limité à leur métier alors, compétences, ils peuvent répondre à tous les actes lorsque la mer est en bonne santé. Une profession, plus que jamais incontournable, le législateur a enfin tenu parole par rapport à un combat mené sur tous les bancs du Parlement. Loin de l'image d'Epinal, la profession de sage-femme et profondément exigeante, elle suppose une formation longue, qui sera intégré à l'université après nos débats, elle concerne la naissance mais aussi l'avant et l'après, comme certaines professions liées à la santé, la profession de sage-femme mérite d'être honoré d'un parcours universitaire cela illogique logique par rapport à nos politiques de santé publique et à notre soucis d'un enseignement universitaire cohérent pour cette raison, je me réjouis de cette université Ariza Sion, que ce soit dans les UFR de santé ou même dans une composante de formation en médecine parce que c'est une formation longue, j'approuve la mise en place d'un doctorat qui pourra couronner ce parcours universitaire. Dans cette même logique, j'approuve la création d'un 3ème cycle d'études pour les étudiants en maïeutique s'est en effet rapproché le parcours d'une sage-femme des autres matières enseignées qui font toutes l'objet d'un 3ème cycle cela est également logique à une époque où la spécialisation et dont tous les parcours d'études. Enfin, cette proposition de loi tient compte des impératifs propres à ceux qui enseignent, ils pourront exercer conjointement des activités de soin de recherche, d'enseignement, c'est aussi un aspect important que l'on retrouve notamment en médecine car il est difficile de dissocier la théorie de la pratique surtout dans les domaines de la naissance. En raison de cette proximité, il est aussi pertinent qu'un statut de maître de stage universitaires en maïeutique soit défini, cela participe d'un accompagnement optimal des étudiants pendant leurs stages, mais cette reconnaissance d'un statut universitaire n'est pas la seule avancée de cette proposition de loi tant attendu, le texte modifie la place des sages-femmes dans la nomenclature de l'Insee, je me réjouis de les voir classé dans le groupe activités des médecins et des dentistes et non plus dans autres activités pour la santé humaine et donc dans cet entre-deux qui fragilise leur positionnement. Vous l'aurez compris, nous sommes dans une situation qui n'est pas éloigné de la médecine, faire de la sage-femme, un acteur de référence pour la prévention, la santé gynécologique des femmes doit être une priorité et c'est urgent, c'est une juste reconnaissance. Tous ces dispositifs doivent rendre la profession plus attractive, donner plus de visibilité en repensant les carrières encourageant les vocations et si nécessaire, comme en témoigne la pénurie dans les hôpitaux. Ce métier connaît une crise profonde qui s'est traduite par de fortes mobilisations début 2021 sont beaucoup d'écho car les sages-femmes sont peu nombreuses. Mais cette amélioration que je salue et que je vous invite à approuver doit être accompagné d'autres progressions en particulier en termes de statut et de rémunérations, pourquoi ne pas aller non plus vers un statut de praticien hospitalier. Certes, les conditions d'études seront améliorées mais il ne faut pas oublier les conditions d'exercice tout court de cette profession, c'est une profession jeune et il faut investir dans cette filière où les résultats sont bons. Comme pour d'autres professions, nous avons besoin d'être plus attractif pour les sages-femmes dans les zones rurales dans le périurbain, une femme doit pouvoir accoucher au plus près de son lieu de vie et en sécurité. Elles sont pour le gouvernement un exemple alors Madame la Ministre, qu'on vous mettez en place les IPA et que nous connaissons les résistances qu'il peut y avoir les sages-femmes par leur pratique et leur histoire éclaire le chemin au lieu d'ignorer les demandes des sages-femmes, ces dernières années, c'est l'inverse qu'il fallait faire les écouter et en faire un exemple. Leurs compétences dans le domaine de la santé gynécologique de l'IVG médicamenteuse de l'IVG instrumentale et expérimentale, actuellement, les sages-femmes permettent au quotidien, l'accès à des soins essentiels en augmentant leur Champ de compétence, on trouve ainsi une réponse à un sujet démographique médicale préoccupant, les sages-femmes attendent de ceci depuis longtemps des nouvelles perspectives ont ainsi s'offrir en termes de recherche et d'exercice du métier, les sages-femmes sont indispensables à la santé des femmes, on a besoin de leur expertise et c'est le cas en particulier en terme de détection des violences sexuelles de maltraitance dans la famille et de détection des personnes vulnérables, n'oublions pas ce rôle social que je voulais, sage-femme,

Suis désolé hein, je suis le maître du temps si on finit pas 20 heures 40 le texte, il sera revu, à une date ultérieure, alors on va faire attention en allemand, on est bien, c'est bon, mais je me permets de rappeler cela à chacun d'entre vous, la parole est à Madame Colette Mélot pour le groupe, les indépendants et pour 4 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission madame la rapporteure, mes chers collègues, nous sages-femmes jouent un rôle majeur dans notre société, celui de permettre de donner la vie, un rôle essentiel au moment de la grossesse de l'accouchement et du suivi post-natal, n'oublions pas qu'elle réalise 80 % des accouchements dits normaux en France malgré le fait que chacun s'accorde sur leur importance pour les familles, ainsi que dans le secteur de la santé, la profession est plutôt mal reconnu, ce qui est paradoxal, alors que leur Champ de compétence ne cesse de s'accroître, et tout naturellement leurs revendications le métier évolue continuellement importante toujours plus de sécurité pour les parturientes et leur bébé, je tiens à saluer les auteurs de cette PPL qui a déjà été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale signe s'il en fallait du sujet crucial que nous examinons, je remercie le groupe écologiste solidarité territoire pour son inscription au sein de sa niche parlementaire la PPL a également été voté à l'unanimité par les membres de la commission des affaires sociales et je remercie notre rapporteur pour le travail effectué afin de permettre une application très prochaine de ces nouveaux dispositifs: les 5 articles que contient cette PPL constitue une véritable réforme il vise purement et simplement supprimé le flou autour de la profession sur son appartenance au secteur médical ou au secteur paramédical avec la création du diplôme d'État de Docteur en maïeutique proposée par la PPL ce flou n'a plus lieu d'être, les sages-femmes sont insérées au sein du statut médical cette formation fera désormais partie des formations médicales et universitaires, cela répond à la revendication principale des sages-femmes et je me réjouis de cette avancée, c'est essentiel pour la formation, bien sûr, mais également pour l'attractivité de la profession, la rémunération, mais aussi l'offre et la qualité des soins prodigués, je tiens à encourager le développement de cette formation sur tous nos territoires, nous sommes nombreux dans cet hémicycle, à savoir combien il est important d'avoir des offres de formation implantée sur l'ensemble de l'Hexagone, les étudiantes et étudiants restent généralement dans les villes où ils ont étudié il renforçant l'offre de soins, à l'heure où l'on évoque de manière récurrente, les déserts médicaux cette pratique pourrait contribuer à des avancées significatives dans ce domaine, c'est pourquoi je me félicite également de la création du statut de sage-femme agréée maître de stage des universités l'an, l'accompagnement des étudiantes et étudiants et gage d'une formation complète et de professionnels compétents, bien sûr, tout essentiel : quelle est cette PPL ne sera pas suffisante et la porte cependant une solution adéquate à la situation actuelle, clarifier le statut de sage-femme doit être appréhendée comme la première étape d'une réforme plus profonde. Je pense d'ailleurs que cette réforme doit être plus globale et concerner l'ensemble notre système de santé, il a déjà bien évolué, mais les dernières années nous ont montré que des changements doivent être déployés pour cela nous devons poursuivre nos réflexions et ajouter aux avancées déjà réalisées, des nouveaux progrès le groupe, les indépendants, conscient de l'importance de cette PPL et des améliorations qu'elle engendrera votera en faveur de ce texte, merci. Merci, cher collègue, la parole est à Madame Monique de Marco, pour le groupe écologiste solidarité et territoires pour 4 minutes. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi a été adoptée il y a près d'un an à l'Assemblée nationale, le groupe écologiste sur la vérité, territoire a souhaité l'inscrire à l'ordre du jour pour aider une profession souffrance et de céder les études en 2018 déjà, l'association nationale des étudiants sages-femmes relevé que 70 % des sages-femmes en formation présenté des symptômes dépressifs et que 27 % songé à quitter la profession malgré ces signaux d'alerte, peu de choses avaient été faites pour répondre à cette détresse en juillet 2021, un rapport de l'IGAS relancer la question de l'intégration du cursus de sage-femme à l'université, une circulaire de 2012 fixé le même objectif : elle n'a jamais été appliqué nous avons conscience du contexte dégradé d'exercice pour les sages femmes placée désormais sous l'autorité de médecins obstétriciens et dans un contexte budgétaire hospitaliers contraint dans le même temps, le rapport de notre société, ananas qualité a évolué avec la baisse du taux de fécondité et les exigences des patients, enfin l'ensemble du corps médical se sont accrues. La détérioration des conditions d'exercice des personnes accompagnant les maires dans leur grossesse et l'accouchement n'a pas été pris à bras le corps. Nous cherchons aujourd'hui à apporter une première Pierre à l'édifice dans la rue, Valérie. Sont de cette profession essentielle à la vie, nous voulons leur dire ici toute notre confiance. La santé des femmes et celle des sages femmes vont de Pair, l'histoire nous montre d'ailleurs que la valorisation de cette fonction autrefois confiée à des matrones sans formation à toujours améliorer la prise en charge des patientes et des nouveau-nés. La professionnalisation et de renforcement du matériel pédagogique, sous l'impulsion de personnalités ingénieuse comme Angélique de Coudray au XVIIIe siècle, ont contribué à faire chuter la mortalité des nouveau-nés et des mères, elle avait créé un petit mannequin pour expliquer les manoeuvres obstétrical cette proposition de loi répondent donc sans ambiguïté. Au besoin de revalorisation du métier de sage-femme, par exemple avec l'intégration universitaire de l'ensemble des écoles de sages-femmes d'ici 2027. également, avec la création du titre de Docteur en maïeutique. En facilitant, ensuite c'est la possibilité pour les sages femmes de pouvoir enseigner, faire de la recherche tout en même tenant une activité clinique. Et enfin par la reconnaissance de la nomenclature Insee de la profession de sage-femme comme médicales et non paramédical. Au même titre que les médecins et les dentistes, il s'agit d'une demande de longue date de la profession. Le texte ne répond pas à toutes les attentes et notamment aux espérances en matière de rémunération. Madame la Ministre notre geste parlementaire de revalorisation universitaire devra se doubler d'un geste du gouvernement pour une heure revalidation budgétaire. Pour un exercice apaisée de la profession d'autres changements doivent intervenir, je pense notamment au statut de sage-femme référente porté par le groupe écologiste solidarité territoires en 2021 lors de l'examen de la loi. Visant à l'amélioration de la santé, pas la confiance et nous attendons toujours la publication du décret pour que cette nouvelle disposition puisse rentrer en vigueur grâce à l'initiative d'Enis ça peut donc je salue la présence en tribune et au travail de Raymond. Pensez Monge dans son rôle de rapporteur, nous espérons que cette proposition de loi puisse rapidement entrer en vigueur et dans les meilleures conditions, je souhaite que notre chambre puisse faire preuve de sagesse transpartisane en lui apportant un soutien unanime comme à l'Assemblée nationale et en commission des affaires sociales, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à messieurs Xavier Iacovelli. Pour le groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants et pour quatre minutes chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, chers collègues, la profession de sage-femme a progressivement évolué, elle a évolué du point de vue de la reconnaissance nécessaire et celle-ci a toujours fait l'objet de combats de cri d'alerte de mobilisation de ces femmes et ces hommes qui tiennent souvent nos enfants avant nous. Elle a évolué, surtout du point de vue de leurs compétences, de leurs missions qui se sont largement renforcé au fil du temps, notamment dans le domaine de l'obstétrique et de la périnatalité, elles se sont par ailleurs élargies en matière de gynécologie, depuis les années 2000, leurs missions sont essentiels puisque les sages-femmes suivent en toute autonomie une patiente de la déclaration de la grossesse jusqu'à la réalisation des soins post-nataux du nouveau-né et de la mer, ainsi que la réalisation de certaines vaccinations, elles peuvent également conduire l'entretien prénatal précoce qui est fondamental pour préparer l'arrivée d'un nouveau né et des bien sûr les parents et les futurs parents à le devenir et dissiper les doutes et questionnements qui peuvent peser sur sur eux dans cette période particulière la loi du 21 juillet 2009 a par ailleurs élargi leur Champ de compétence, sous réserve de suite : formation, elles peuvent désormais réaliser des échographies gynécologique des actes d'ostéopathie prescrire des contraceptifs hormonaux ou encore posé des dispositifs contraceptifs sous-cutané conduire des consultations de contraception et de suivi gynécologique dans une logique de prévention auprès des femmes, enfin en 2021, elles peuvent, depuis 2021 bon, elles peuvent prescrire certains médicaments et des arrêts de travail, sans limitation de durée, pourtant ces évolutions majeures ne sont pas accompagnés d'une reconnaissance croissante de leur métier et c'est bien là dont il s'agit, car le nombre d'étudiants sages-femmes n'a jamais cessé d'être de de baisser, il est jamais été aussi bas avec 20 % de places vacantes pour cette année universitaire malgré l'action du gouvernement qui avait acté une augmentation du nombre de places de un virgule 5 pour 100 par rapport à 2020, le constat est alarmant, chers collègues, sur 1000 sages-femmes 100 quittent la profession dans les 2 ans qui suivent l'obtention de leur diplôme, face à cette pénurie due au décalage criant entre les niveaux de responsabilité et la reconnaissance dont elle bénéficie, le gouvernement à apporter des réponses concrètes afin de renforcer l'attractivité du métier, je pense bien sûr à la revalorisation financière de 500 euros Net par mois en moyenne pour les sages-femmes hospitalières, je pense également à la prolongation du doublement du taux de promu Promovac bleu dans la fonction publique hospitalière sur la période 2022 2024, il s'agit là d'un engagement inédit du gouvernement puisque l'ensemble de ces mesures de revalorisation représente 100 millions d'euros en 2022 par ailleurs la création d'un entretien post-natal précoce obligatoire et les campagnes d'information visant à promouvoir les compétences des sages-femmes confier à la CNAM dans le cadre du dernier Plfss traduisent la reconnaissance de l'État envers celles et ceux qui oeuvrent aux côtés des parents et des nouveau-nés à cet égard la proposition de loi que nous examinons visant à faire évoluer la formation des sages-femmes comporte des dispositions intéressantes que nous saluons, puisqu'elles vont dans le sens d'une meilleure reconnaissance du métier, elle permettra de renforcer la qualité de la formation en créant un site, un diplôme d'état du Docteur en maïeutique et pour rendre systématiquement l'organisation de la formation initiale des sages-femmes au sein des universités, elle crée également un statut de maître de stage universitaires pour mieux accompagner les étudiants et créer un 3ème cycle d'études pour les étudiants en maïeutique conformément à l'engagement du gouvernement afin de leur permettre de découvrir les différents modes d'exercice sur le territoire, leur place dans la démocrature statistiques permettra de reconnaître davantage le caractère médical de la pro de la promotion, ce que bien sûr nous saluons cette proposition de loi comporte d'autres dispositions intéressantes puisque grâce à ce texte, les sages-femmes, enseignante chercheuse pourront désormais exercer une activité de soins en parallèle de leur fonction d'enseignement et de recherche pour toutes ces raisons et je viens d'en évoquer plusieurs notre groupe votera favorablement pour cette proposition. merci beaucoup, la parole est à Madame Émilienne rôle pour le groupe socialiste, écologiste et républicain et pour six minutes chers collègue. Comme la présidente, madame la Ministre Madame la rapporteure, madame la présidente de la commission, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier le groupe écologiste solidarité territoires et la rapporteure, Madame Raymonde Poncet mange d'avoir mis ce débat à l'ordre du jour ne souhaite rassembler aujourd'hui ce texte très attendu par les sages-femmes sera je l'espère, l'occasion de faire entendre leur voix et de porter la reconnaissance et la valorisation que la profession de sage-femme mérite au fil du temps avec la médicalisation et la technicisation croissante des accouchements, les sages-femmes ont vu leur rôle évoluer leurs compétences élargir mais leur statut lui est resté inchangé en effet alors que le code de la santé publique reconnaît le métier de sage-femme comme une profession médicale leurs actes ne sont que partiellement reconnu dans les nomenclatures, cette situation est paradoxale car face au manque de gynécologues sont aujourd'hui devenus les relier les piliers indispensables du parcours de santé de la femme ainsi depuis plusieurs ardennaise exerce de nouvelles activités en dehors du centre-traditionnel de la grossesse, telles que le suivi gynécologique, la prescription de contraceptifs, la pratique de l'IVG, la préparation à l'assistance médicale à procréation ainsi que la prévention et l'éducation à la sexualité, cet enrichissement des compétences des sages-femmes a nécessairement conduit à augmenter la densité de leur formation initiale, qui a par re-aujourd'hui comme trop dense, hé bien supérieure à celle des autres professions médicales, comme un volume supérieur de 1246 heures par rapport à d'autres formations médicales qui dure au minimum six ans c'était une densité des études nuit au bien-être étudiant et à l'attractivité des études en maïeutique et selon la en 2018, plus des 2 tiers des étudiants de la maïeutique souffrait de symptômes dépressifs face à ces constats, il était indispensable de réformer la formation du des sages-femmes et à cet égard la présente proposition de loi consacrent dizaines penser que nous saluons, dans un article 1er le texte établit la nécessité de parachever l'intégration universitaire des sages-femmes afin de lutter contre les inégalités entre les différentes écoles puisqu'aujourd'hui, sur 35 écoles 24 fonctionnent encore selon une régulation financement régional, tandis que 11 ans d'opter pour le financement, universitaire, ce qui crée une disparité préjudiciable à titre d'exemple, dans certaines écoles, les financements régionaux n'ont pas évolué et la réforme du numerus apertus effectué l'année dernière n'a pas pu être mis en oeuvre, donc le nombre de places en formation pour les sages-femmes n'a pas augmenté au contraire en donnant aux universités la compétence d'agréer de financer des écoles cet article 1er renforce ainsi le statut médical des sages-femmes, la création de statut de sage femme agréée maître de stage, des universités ou au même titre que pour les médecins généralistes par l'article 1 représente une avancée importante de l'encadrement des étudiants et dans la valorisation de la fonction de d'encadrement, sages-femmes, l'article 2 en consacrant la mise en place d'un 3ème cycle universitaire, répond à une demande forte de la profession et le groupe certes ils soutiennent depuis longtemps cette mesure se félicite de sa mise en oeuvre dès la rentrée 2024 et nous avons expliqué pourquoi nous regrettons néanmoins que, renforcement de la formation continue des sages-femmes en passant de 2 et demi à 15 jours par an, comme le demandent les syndicats et lourde ne sont pas prévu dans ce texte, autres mesures pour renforcer l'attractivité de la profession, c'est l'article 3 qui prévoit la possibilité donc aux doctorants, de la filière maïeutique d'exercer simultanément leur activité professionnelle et des activités d'enseignement et de recherche, enfin dans un article IV la présente proposition de loi reconnaît l'activité de sage-femme comme une activité de pratique médicale au sein de la nomenclature, ce qui était importante des activités françaises de l'Insee, cette mesure répond à une demande récurrente de la profession et mis fin à une situation injustifiée eu égard ou à leur activité, mes chers collègues, donc ces 2 propositions de loi adoptée, cela a été dit à l'unanimité par l'Assemblée nationale présente de réelles avancées pour la reconnaissance de la profession de sage-femme et le groupe socialiste, écologiste et républicain la soutiendra, néanmoins, la réforme de la formation ne représente qu'une partie de la réponse à apporter au sentiment de déclassement des sages-femmes et au besoin d'attractivité de la profession depuis de nombreux mois, les sages-femmes alerter les pouvoirs publics sur leurs conditions de travail et face au silence des pouvoirs publics, elles ont manifesté, elles ont fait grève ainsi les questions de rémunération qui sont encore en deçà des autres professions médicales, les questions des conditions de travail loin du modèle, une sage-femme, telle que mise en place certaines de nos voisins européens, un enfant du manque de personnel, la révision des décrets de péril la vitalité devront faire l'objet de prochains textes aujourd'hui une sage-femme est amené à prendre en charge jusqu'à 3 patientes par garde de 12 heures en salle de naissance et 25 patiente ensuite de couches dans certains contextes, il paraît difficile pour les sages-femmes d'avoir assez de temps pour accompagner correctement tous les couples qu'elles doivent suivre les conditions de travail dégradées ont des conséquences sur la santé mentale des sages-femmes et près de 40 % d'entre elles ont un burn-out en milieu hospitalier, le métier de sage-femme et tellement perte d'actrice d'attractivité qu'on a enregistré en France, près de 20 pour 100 de postes vacants, je me permets donc de vous interpeller madame la ministre sur la nécessité d'un texte plus large sur la périnatalité et sur l'accompagnement de la santé des femmes et des nouveau-nés dans la lignée se dirait du rapport sur les 1000 premiers jours un texte d'autant plus nécessaire que l'Agence nationale de santé publique dans ce rapport du 20 septembre sur la santé périnatale note de grandes inégalités territoriales avec une situation qui s'est aggravée

Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je remercie à mon tour, le groupe écologiste et ça rapporte Raymonde Poncet Monge d'avoir repris un texte adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale visant à faire évoluer la formation des sages-femmes sont 23400 et prennent en charge chaque année plus de 750000 femmes qui accouchent et autant de nouveaux-nés elles assure la surveillance, le suivi médical de la grossesse prépare à la naissance à la parentalité, cette proposition de loi vise donc à moderniser la formation des sages-femmes, en parachevant l'intégration universitaire de leur formation, d'une part en créant un 3ème cycle d'études en facilitant la recherche en maïeutique et d'autre part on réaffirmant le statut médical du métier de sage-femme depuis de nombreuses années les étudiantes en maïeutique ainsi que la communauté des sages-femmes milite pour l'intégration universitaire des études de sage-femme parmi les professions médicales, celle des sages-femmes, et la seule dont la formation n'est pas intégralement assuré par les universités cette situation entraîne de fortes disparités sur le territoire, selon une enquête de l'association nationale des étudiants sages-femmes, réalisé en 2019 seuls 16 % des écoles aurait mis en place des référents la création d'un stage de maître de stage, univers d'un statut, pardon de maître de stage universitaires prévues par le texte répond donc à une attente forte des étudiantes, les études en maïeutique comporte aujourd'hui un volume horaire nettement supérieur aux autres formations médicales qui explique pour une part que cette étudiante sur 10 présentent des symptômes dépressifs, la création d'un 3ème cycle d'études en maïeutique vise donc à alléger le volume horaire des enseignements et à mettre en cohérence, la formation des sages-femmes avec leurs compétences, qui n'ont cessé de s'étendent ces dernières années, tant en matière obstétrique gynécologique pédiatrique qu'en matière de prévention, les sages-femmes constitue une profession de santé aux conditions de travail dégradées à qui l'on demande toujours plus sur le plan médical sans que la reconnaissance sur le plan statutaire et salariale suive, on se souvient toutes et tous, ici, de leur longue mobilisation pour se faire entendre, gouvernements successifs ont ajouté des compétences étendues les attributions des sages-femmes sans compensation salariale ni amélioration de leurs conditions de travail et revalorisation de leur qualification, comment expliquer que cette profession médicale soit si mal reconnu, Madame la Ministre, si ce n'est peut-être parce qu'elle est exercée quasi exclusivement par des femmes dans la fonction publique hospitalière, les sages-femmes n'appartiennent pas à la catégorie des personnels médicaux, alors qu'elles sont titulaires d'un diplôme de niveau bac plus cinq incluant une première année de médecine, elle commence entre 1600 et 1800 euros Net par mois et sont exclus du bénéfice de diverses il faudra donc continuer à légiférer pour reconnaître le métier de sage-femme améliorer leurs conditions de travail revaloriser leur rémunération, contrairement au gouvernement qui ajoute une dixième année de médecine dans le PLFSS 2023 sans sans discussion avec les internes, ils réflexions sur leurs études, cette proposition de loi ajoute une année d'études en prenant en compte le rythme de la de la formation, le contenu pédagogique et les nouvelles compétences des sages-femmes depuis de plus, elle autorise les enseignante chercheuse en maïeutique à pouvoir cumuler la recherche et leur activité clinique, sans possibilité de refus, autant d'avancées, je note bien sûr que l'association nationale des étudiants sages-femmes aurait voulu que le texte aille plus loin en accordant un statut spécifique permettant la bi-appartenance hospitalière et universitaires, cette proposition de loi ne répond pas l'ensemble des revendications de la profession, mais elle constitue une première étape et c'est important, et je pense à mon ami et camarade, le Docteur Paul Cesbron, qui l'aurait salué lui le militant infatigable de la reconnaissance de cette profession comme hautement médical en attendant donc, hé bien, les sénateurs et sénatrices du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste voteront en faveur de cette proposition de loi, je vous remercie et madame la présidente, je vous cède 8 second. C'est parfait, merci beaucoup, la parole est à monsieur. Que son mari vend le Reneberg pour le groupe Union centriste et pour six minutes. madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure et chers collègues qu'il est loin le temps des accoucheuse voilà 2 ans, de siècle pardon que le législateur donne de plus en plus de responsabilités aux sages-femmes justement qui nous offrent le 1er souffle de vie quitter le domicile pour la maternité, fut une évolution dans la prise en charge médicalisée de l'accouchement mais l'exigence accrue de sécurité, entraînant la fermeture en 25 ans de 40 % de ces maternité trop petite ou sans obstétricien et au passage la marginalisation des sages-femmes de leur rôle, le discrédit est aujourd'hui telle que, selon la sur l'association nationale des étudiantes à peine plus de la moitié d'entre elles penseraient à exercer uniquement à l'hôpital, pire, la vacance de 20 pour 100 des places ouvertes cette année en formation, souligne ce désamour la souffrance au seul stade de la formation, mais aussi dans les fonctions professionnelles nous interpelle les mouvements sociaux de l'année passée, nous l'ont très justement rappelé en effet la barque des sages-femmes s'est vu chargé au fil du temps, de nouvelles responsabilités médicales mais qu'en est-il de la reconnaissance, le sentiment exprimé par la profession et celui d'un entre-deux d'une zone grise qui ne reconnaît pas leur travail à sa juste valeur, au fond, je crois qu'on ne saurait dissocier la question du statut des sages-femmes de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais nous ne pouvons plus les laisser dans un statut qui ne correspond pas à leur rôle dans notre système de santé donc défendre les sages-femmes, c'est aussi défendre les femmes, le gouvernement a apporter une première réponse et je la salue sur les salaires, le parlement se charge aujourd'hui de la question de la formation, je me félicite que cette proposition de loi madame la rapporteure puisse nous appuyer une démarche sur une démarche aussi consensuel en en ce sens, l'article 1er vice-donc à valoriser la formation initiale des sages-femmes en posant les bases de son intégration universitaire, un chantier, vieux d'une décennie en décloisonnant les formations en santé, nous pourrons tendre vers une plus grande égalité entre les étudiants et je l'espère rendre cette filière plus lisible et plus attractive, c'est aussi l'occasion de faire de la pluridisciplinarité, une richesse pour notre système de santé pour ne plus enfermer les acteurs dans une spécialité où il sera difficile d'évoluer même de sortir, ceci fait écho à l'accord que vous avez rappelé : Madame la Ministre, dont je me réjouis, qui vient de se conclure entre les 3 ordres, l'Ordre des médecins, des kinés, des infirmiers dans la continuité, l'article de vient quant à lui, créer un 3ème cycle d'études réaffirmer les connaissances physiologiques des sages-femmes et nécessaire renforcer leur discernement sur les situations pathologiques, en y associant, bien sûr, l'apport des nouvelles technologies l'est aussi, ce passage à bac plus six est une avancée dans le chantier de l'attractivité de ce métier, la rémunération résonnait déjà de sa faiblesse à bac plus cinq, alors il faudra y être encore un peu plus attentif, pardon, de formation, l'article 3 permettra de rompre avec l'inégalité, une de plus entre les sages-femmes et les médecins, pharmaciens ou chirurgien dentiste en autorisant les doctorants, de la filière maïeutique à exercer simultanément leur activité professionnelle avec la recherche, l'enseignement, ce sont les sages-femmes de demain qui gagneront l'article 4 enfin vient reconnaître l'activité de chasse de sage-femme comme pratique médicale, alors que le code de la santé publique, considérer les sages-femmes comme une profession médicale, la nomenclature enfin des activités françaises là cantonné au domaine paramédical, cette évolution est donc bienvenue sur ces bases, l'Union centriste votera donc favorablement ce texte mais restera aussi attentif que vous, chers collègues, à ce que le 1er pas en faveur de la formation en la d'autres plus franc sur les conditions de travail, merci beaucoup de votre attention. Si cher collègue, la parole est à monsieur Stéphane Ravier pour 3 minutes.

Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, où sont les sages-femmes vraiment le commandant tous les deux oui les sages femmes vont mal, nous en convenons tous les maux de la profession sont connus des salaires trop faibles commençant en 1700 euros Net par mois après cinq et peut être bientôt 6 années d'études sélectives, un manque d'attractivité, alors qu'à la rentrée 2022 20 pour 100 des places en deuxième année d'études sont restées vacantes des études très intense, alors que 70 % des étudiants présentent des symptômes dépressifs des sous- effectifs chroniques qui font que 44 % des sages-femmes ont déjà fait un burn-out, une sage-femme a toujours plusieurs femmes, plusieurs maires à gérer en même temps, alors qu'elle ne devrait en avoir qu'une seule, pour un suivi de qualité car oui n'en déplaise au planning familial et aux idéologue d'extrême gauche, ce sont bien les femmes qui tombe enceinte et qui accouche et que l'on appelle maman est pas parents ou parents de mais au-delà de ces chiffres alarmants, il y a une réalité qui n'est pas quantifiable toutes les sages-femmes que j'ai rencontrés m'ont dit une chose, elle manque de reconnaissance qui a fait le gouvernement macronien depuis 5 ans au mieux les ignorer, au pire, les mépriser au début de la crise sanitaire, elles ont été tout bonnement oublié dans la distribution des masques destinés à protéger les professionnels de santé, les syndicats de sages-femmes ont également été oubliés dans les négociations du Ségur de la santé de 2020, aujourd'hui encore, leur profession n'est toujours pas reconnu comme essentiel puisque sur une grande partie du territoire, elle ne fait pas partie des métiers prioritaires pour accéder aux stations essence ces vexations répétées ne sont peut-être rien pour vous, mais elles en disent beaucoup de la considération dans laquelle cette majorité les tiens et surtout, surtout, café le gouvernement contre le manque d'effectifs qui transforment leur journée de travail en enfer comme les autres professions médicales, il a été décidé de suspendre les sages-femmes non vaccinés contre le Covid 19 parce qu'elle souhaitait disposer librement de leur corps, ces personnes ont été brutalement humilié à l'heure où toutes les études démontrent que ces vaccins n'empêche pas la transmission du virus, il n'est pas trop tard pour pour faire amende honorable et revenir sur cette décision odieuse pallier le manque d'effectifs est une urgence avant de prétendre former de nouvelles sages-femmes, ce qui prendra six ans il faudrait commencer par réintégrer celles qui le sont déjà, en ce mois d'octobre rose où nous alertons sur les dangers des cancers du sein, rappelons que les sages-femmes sont des interlocutrices de choix pour effectuer des dépistages à ce titre aussi, nous devons les choyer cette proposition de loi n'est certes pas dépourvue d'intérêt, il reprend certaines demandes de la profession, chez moi à Marseille et l'ensemble de la formation est déjà intégré à l'université et cela fonctionne, mais plus que des mesurettes ces de reconnaissance, j'insiste, de reconnaissance dans les sages-femmes ont besoin afin qu'elles retrouvent la dignité liée à une profession essentielle car une société qui ne sait plus accueillir la vie est une société qui. C'est magnifique, merci beaucoup la, elle est à Madame Kilène Pantel pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour quatre minutes chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure chers collègues. Bon nombres d'éléments pertinents ont été évoquées par les orateurs précédents et je ne m'y attarderai pas je souhaiterais simplement souligné dans mes propos introductifs l'importance du texte que nous examinons aujourd'hui au Sénat, après son adoption à l'Assemblée nationale le 25 septembre 2021 en effet au cours du premier confinement au printemps 2020 la notion de travailleurs essentiels a fait irruption dans le débat public avec certes quelques controverses sur le périmètre que cela pouvait recouvrir mais avec un large consensus autour de leur nécessaire revalorisation, le secteur de la santé et entités nettement ces dernières décennies, les professionnels comme les sages-femmes ont fait partie de ces personnes exerçant à l'hôpital ou un libéral identifié par nos concitoyens comme n'étant pas suffisamment reconnus à leur juste mesure. à la suite d'un recueil de plusieurs témoignages et notamment celui d'une sage-femme, un établissement de santé privés d'intérêt collectif, ce déficit de reconnaissance s'ajouter selon elle à des stéréotypes sur la profession consistant à les imaginer comme des 12 subalterne dans le rôle ne sur Syrte à la participation aux accouchements, or la moindre prise de recul, nous enseigne que c'est bien loin d'être leur seule mission fondamentale et que d'autres responsabilités tacite viennent se greffer dans leur quotidien, c'est en grande partie, ce qui a motivé les auteurs de cette proposition de loi par l'étouffement de la formation de sages-femmes et son rapprochement avec les études de médecine. L'intégration universitaire de la formation de sages-femmes est une mesure positive pour une meilleure appréhension des relations avec la myriade d'acteurs que les étudiants seront terminées à côtoyer, idem pour la création du 3ème cycle qui leur conférera de solides compétences et un statut pérenne de Docteur à magnétique. La possibilité de combiner leur activité professionnelle avec des activités d'enseignement et de recherche est une belle ambition, mais qui ne doit pas se traduire par des pertes de revenus, nous connaissons la grande précarité subie par les doctorants en France. Par ailleurs, ces avancées notables ne doivent pas nous faire oublier les alertes liées aux difficultés de recrutement, en effet, cela a été dit à maintes reprises la profession vient une véritable pénurie de main-d'oeuvre général, les explications sont plurielles et on identifie notamment celle du syndrome d'épuisement professionnel qui trouve son origine à la surcharge de travail. Anne, outre les sages-femmes constate une extension de leurs attributions, tandis que les autres leurs horaires, eux, ne sont pas extensibles, dès qu'il y a une tâche supplémentaire à réaliser, à raison de l'absence d'un collègue secrétaire aide-soignants et autres, c'est à nous de l'assumer, nous affirme l'une d'entre elles, sans compter bien d'autres paramètres comme comme la relation étroite qu'ils et elles entretiennent avec les patientes et l'identification de difficultés nécessitant un accompagnement social de toute urgence, mais pas toujours opérationnel en fonction de l'établissement d'exercice aussi et, pour faire écho au débat précédent sur la proposition de loi constitutionnelle sur la protection de l'IVG et de la contraception porté par notre collègue Mélanie Vogel n'oublions pas le rôle essentiel des sages-femmes a matière de diffusion d'informations fiables et de soins de qualité et disent a fait malgré ces éléments de réflexion annexe à la proposition de loi qui devront inévitablement faire l'objet d'une attention particulière à l'avenir, notre groupe du Rassemblement démocratique et social européen votera à l'unanimité en faveur de ce texte, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Bruno Belin pour. Le groupe Les Républicains et pour cinq minutes chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission madame la rapporteure. Soutien total au texte évidemment Notre collègue, elle se Joseph tout à l'heure, a rappelé la position du groupe en rappelant l'historique, la nécessité de faire évoluer cette profession et donc à mon soutien total, mais 3 vérités 3 vérités : d'abord une nécessité nécessité parce que le volume des compétences exigées de c'est sa femme a évidemment augmenté depuis la dernière réforme du statut de formation qui doit dater de 1000 2011 augmenter je pense notamment à à l'entretien post-natal précoce, je pense, oh quelle heure il calendrier de vaccination qui a fortement augmenté, je pense à des sujets comme l'endométriose sujet totalement tu il y a encore quelques années et puis évidemment, on pourrait penser au au recours croissant sur les besoins de lutte contre un certain nombre d'addictologie donc première vérité mais la mamie c'est cette nécessité d'une année supplémentaire. Mais il y a une 2ème vérité c'est la réalité, la réalité risque d'être le manque parce que, là encore, nous manquons de sages-femmes et nous manquons là encore de candidats dans les écoles, la réalité du numerus apertus c'est plusieurs années je rabâche, j'en ai parlé hier mais c'est que pour l'instant on ne voit pas comment ça va apporter une solution sur un certain nombre de manque de professionnels de santé. Dont celui de sa femme, ça c'est une réalité criante la gynécologie libéral manque sur plus d'une dizaine de départements manque totalement sur d'une dizaine de départements en France, le nombre de sages-femmes est quasiment inexistant en milieu rural en milieu libéral et puis on voit même arriver si j'ai pas entendu dans le débat, un certain nombre de professionnel, je pense à des coaching en natalité ou des doulas qu'on voit apparaître ici et là et là, moi, quand je vois apparaître ça je me dis méfiance et donc cette 2ème vérité c'est cette réalité de terrain qui fait que l'on doit effectivement professionnaliser augmenter le volume de sa il y a une il y a une troisième vérité, c'est évidemment l'urgence. L'urgence de professionnels valoriser le statut parce que si effectivement on n'en veut plus, il faut valoriser ce statut, je vous rappelle, et ça a pas été dit dans les disparités Laurence Cohen, à tout à l'heure parler des questions de salaire mais vous savez qu'il y a une disparité forte chez sa femme entre entre fonction publique quand elles sont par exemple dans un conseil départemental dans une PMI ou en milieu hospitalier, ça dire fonction publique hospitalière, on n'a pas les mêmes grilles de salaires, donc si on veut promouvoir cette profession falloir à un moment donné, maître, tout le monde à la même échelle, ça, c'est effectivement une des urgences, l'autre urgence et que votre gouvernement madame la vraiment ça fait 15 ans qu'on parle des déserts médicaux, vous le savez comme moi, on vit le sujet ben on le connaît par coeur, donc à mon et quand est-ce qu'on se met à apporter des réponses concrètes pour qu'on pallie à toutes ces carences de professionnels de santé sur les territoires, moi je crois que celui la compétence de partage de tâches entendait bien ça madame parce que va falloir à un moment donné, arrêter d'être en tuyaux d'orgue que partage de tâches et notamment avec les IPA avec les sages-femmes avec les pharmaciens puissent permettent d'apporter des réponses, donc c'est un texte que l'on soutient, c'est parce que c'est un message évidemment de soutien à la profession de sage-femme, que l'on apporte en votant ce texte ce soir. Merci beaucoup. La discussion générale est Close, madame la miss, vous souhaitez prendre la parole. Merci madame présidente tout d'abord, madame la rapporteure vous remercie d'avoir porté ce texte salué l'autrice du texte, Annie Chapelier présente la présidente de l'Ordre aussi présente et apporter peut être une réponse à certains d'entre vous, notamment sur évidemment, il y avait urgence à reconnaître le métier des sages-femmes, c'est aujourd'hui chose faite maintenant en charge au texte de continuer sa vie parlementaire et comptez sur moi pour veiller à ce que, ils puissent j'allais dire, arrivé à l'Assemblée nationale et être y être voté et vous dire à quel point le gouvernement se mobilise, puisque le dernier orateur, je sais pas, là, vous avez fait allusion à la capacité à travailler des sages-femmes à travailler avec les autres provient de santé, je vous rappelle que, il y a une semaine jour pour jour, les cet ordre et pas les trois, les sept oui, je sais qu'il est là, mais je regarde là je je sais qu'il est là,

puisque les sages-femmes ont un ordre, elles ont fait partie de, de, de, des signataires et elles seront avec les pharmaciens, les pédicures podologues, les dentistes, les infirmiers aux côtés et les pharmaciens, les équipes pédicure podologue des dentistes, des infirmiers, il m'manque les sages-femmes et les kinés aux côtés des médecins pour apporter des réponses et dégager du temps médical : voilà vous vous avez fait une demande c'est déjà exaucé nous maintenant nous allons travailler sur ce principe. Merci madame la ministre, alors nous passons la discussion du texte de la commission, alors je vais mettre aux voix l'article 1er qui est pour.

Annie Chapelier, qui était à l'initiative de sa proposition qui a été député du Gard de 2017 à 2022 d'encre, comprenez qu'entre parlementaires et de solidarité départementale de dire que ce soir, elle peut être fière du du travail qu'elle a fait dans ce domaine là et je dire avec un petit clin d'oeil il y a quelques il comprendra peut dire dans cet hémicycle que ce soir, elle pourra dire que être parlementaire, ça sert à quelque chose, parce que ça, PPL, Havas et je suis sûr que, après les propos de Madame la Ministre, elle sera inscrite en 2ème lecture à l'Assemblée nationale et que la PPL, elle deviendra loi et ça sera la loi Annie Chapelier. Merci, merci, cher collègue. Alors je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi visant à faire évoluer la formation de sages-femmes qui et pour qui est contre qui s'abstient, il est adopté à l'unanimité, madame la présidente, Catherine Deroche bien entendu. Oui, très rapidement, pour remercier d'abord Raymonde Poncet mon sur le groupe d'avoir inscrit ce texte et la remercier de d'avoir rapporté ce texte en y apportant cette modification importante s'étaient mis d'accord avec l'ordre et avec les étudiantes sur le délai, donc je salue en effet, la présidente de l'Ordre je salue la s', associations d'étudiants sages-femmes et bien évidemment. Annie Chapelier, qui verra. Qui verra son texte, alors je sais que pour certains points, vous souhaitez aller un petit peu plus loin mais qu'il vaut mieux tenir que courir et il nous semblait important, déjà 2 cranté cranté ce qui a été mis dans le texte, maintenant, Madame la Ministre, il n'y a plus qu'à l'inscrire très vite à l'Assemblée nationale, de l'adopter conforme à l'Assemblée nationale et voilà, et le texte sera définitivement. Merci madame la présidente. Alors, mes chers collègues, je vais lever la séance et prochaine séance, le jeudi 20 octobre à 10 heures 30 pour l'examen de la proposition de loi créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales, la séance est levée.